Bonjour mes chers collègues. Bonjour madame, la Première ministre, mesdames et messieurs les Ministres, la séance est donc ouverte. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué, y a-t-il des observations. Je n'en vois pas. Le procès verbal est donc adopté sous les réserves d'usage.---- Madame, la Première ministre, mesdames et messieurs le Ministre, mes chers collègues. L'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement.-- Je vous prie d'excuser tout d'abord le président du Sénat. En déplacement à l'étranger. Je vous rappelle que la séance est retransmis en Direct sur Public Sénat et sur notre site internet.-- Au nom du bureau du Sénat. J'appelle chacun de vous, mes chers collègues. A observé au cours de nos échanges, l'une des valeurs essentielles du Sénat le respect et l'écoute dont vous ne faites pas beaucoup. Preuve en ce moment d'ailleurs, je vous trouve assez dissipée, chers collègues. Ça doit être l'émotion de voir effectivement une vice-, présidente, et non notre président au plateau. Je mais effectivement cela sous le coup de l'émotion.-- Donc une valeur essentielle du Sénat le respect et l'écoute des uns et des autres ou celui du temps de parole. Donc vous savez je suis assez à cheval sur ce temps de parole.-- Mes chers collègues, la parole est à monsieur Martin lévrier pour le groupe du Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. Vous avez 2 minutes chers.-- Merci madame la présidente, madame, la Première ministre Madame et messieurs les Ministres, Monsieur le Ministre de la Santé et de la prévention. Samedi à 21h, le Centre hospitalier André Mignot de Versailles a été victime d'une cyberattaque. Une partie des ordinateurs ont été bloqués et un message des cybercriminels s'est affiché sur les écrans tous vos dossiers importants ont été dérobés et crypté, suivez nos instructions. À la paralyser les systèmes informatiques reportant les actes médicaux perturbant le suivi des malades arrêtant ou faisant dysfonctionner les appareils les plus pointues ces barbares mettent en danger la vie des patients et cette attaque n'est pas sans rappeler celle qui avait touché le centre hospitalier de Corbeil-Essonnes au mois d'août. Je voudrais saluer en votre nom à tous, le sang froid des équipes de l'hôpital André Mignot qui comme l'ensemble du personnel soignant en France était déjà largement éprouvée par la pandémie et les difficultés de l'hôpital public. Aujourd'hui, ils ne peuvent compter que sur leurs crayons leurs papiers et leurs jambes pour prendre en charge un maximum de patients. Tout le personnel est à son poste. Je les remercie.-- Je voudrais également saluer la coordination qui s'est immédiatement mis en place entre la direction du CHU, l'ARS l'AP-HP. Les services du SAMU et tout particulièrement les hôpitaux publics et les cliniques privées du département qui se mobilisent et travaillent en bonne Intelligence. L'intégration de l'établissement dans le parcours de cybersécurité. Sécurité pardon a participé à la réactivité sans pareil de l'équipe de l'hôpital qui en coupant rapidement les communications connexion Internet et services d'interconnexion avec le SAMU à éviter la propagation de cette attaque. Ce parcours de cybersécurité a été renforcée à l'Automne avec une enveloppe supplémentaire de 20 millions d'euros. Pouvez-vous, Monsieur le Ministre, nous dire comment ces crédits supplémentaires et de rond nos infrastructures sensibles à renforcer leur sécurité informatique pour se prémunir de ces attaques de plus en plus fréquentes et virulente et quel sera le support technique apportée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, je vous remercie. Pour vous répondre Monsieur François Braun Ministre de la Santé et de la prévention. Madame la présidente, mesdames les sénatrices messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Laugier. Comme vous je condamne le plus fermement possible. Cette cyberattaque contre l'hôpital André Mignot. Jamais nous ne céderons face à ces criminels à ces actes odieux qui tente de prendre en charge de prendre en otage la santé des Français.-- Je veux moi aussi saluer le sang-froid dont ont fait preuve les professionnels de santé sur place et et l'administration de l'hôpital. Je me suis rendu sur place dimanche, avec mon collègue Jean-Noël Barrot et nous avons pu constater un calme tout à fait relatif mais en tout cas une prise en charge assurée en terme de sécurité et de continuité des soins, malgré les grandes difficultés. Devant lesquelles et ils étaient. L'ensemble des services de l'État sont mobilisés bien sûr aux côtés de l'établissement, notamment via la mobilisation de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ARS mais comme vous l'avez dit, l'AP-HP et dans le sens des hôpitaux du secteur qui ont coordonné à la main du du SAMU local et du SAMU zonal pour la prise en charge de la meilleure des patients. Nous devons renforcer notre capacité collective à faire face aux attaques cyber c'est le sens du plan de 350 millions d'euros, porté par mon ministère en février 2021 pour renforcer les protections cyber et surtout le diagnostic de ces établissements cet été suite à l'attaque. La cyberattaque de Corbeil-Essonnes. J'ai annoncé un complément de financement de 20 millions d'euros pour soutenir cette démarche ce complément vise à renforcer le déploiement du plan et surtout passer. À la phase opérationnelle passer du diagnostic à l'action sur des actions précises et concrètes dans nos capacités de cyberdéfense. Avec mes collègues Gérald Darmanin et et Jean-Noël Barrot, nous allons réunir avant la fin de l'année, une nouvelle fois l'ensemble des parties prenantes, avec les fédérations avec l'Inde. Si avec l'ARS pour renforcer notre stratégie. Je tiens à signaler en plus que cette succession d'attaques nous permet de nous renforcer encore plus à chaque fois en particulier sur les actions immédiates à prendre en compte et ce qui a été le cas à l'hôpital mignon, je vous remercie. Oui madame la présidente. Monsieur le ministre, il s'en est fallu de peu pour que vous supprimiez 14.000 places d'hébergement d'urgence dans le projet de loi de finances pour 2023, c'est seulement sous la pression des associations et des élus que vous avez reculé. Maintenant le froid s'installe et les journaux regorgent d'articles relatant les situations de femmes et de très jeunes enfants de femmes enceintes et de mineurs laissé dehors alors que le 115 ne sait plus où donner de la tête. Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ont été fragilisé par les plans d'économies mises en Oeuvres ces dernières années, la hausse des crédits cette année ne suffira pas à les remettre d'aplomb. La réduction du loyer de solidarité en 2018 a mis un coup de frein aux constructions de logements sociaux par les bailleurs sociaux. Selon la Cour des comptes en 2021 en France près de 300.000 personnes se trouvaient avant même la crise sanitaire sans domicile estimation qui a plus que doublé depuis la dernière enquête statistiques de 2012. Le 93 est emblématique ou par exemple, faute de place. Aucun des 739 appelle traités par le 115, le 28 novembre n'a abouti à un hébergement d'urgence. Mais la crise concerne aussi Lyon, Rennes, Grenoble, Strasbourg, Toulouse et beaucoup d'autres communes il y a les inscriptions budgétaires d'un côté et la terrible réalité que nous rapporte la presse tous les jours et que nous avons de toute façon sous nos yeux. Quelles nouvelles mesures allez-vous prendre.-- Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice. Lubin, je tiens tout d'abord à à redire ici ma confiance et mon admiration pour l'ensemble des personnels des services d'intégration, d'accueil et d'orientation Les SIAO. Ils agissent au quotidien pour écouter et accompagner les personnes. Les plus fragiles, ils auraient été la clé de voûte du 1er logement premier plan logement d'abord. Et vous le savez un deuxième plan logement d'Arbor sera annoncée dans les semaines qui viennent, c'est le souhait de du président de la République et et de la Première ministre, Le gouvernement a a souhaité non pas sous la pression mais sous la réalité de l'urgence sociale maintenir près de 200.000 places d'hébergement d'urgence et nous avons ajouté 40 millions. D'euros sur le PLF, je vous rappelle que ce niveau d'hébergement d'urgence n'avait jamais été atteint dans notre pays et en 2017 il y avait 140.000 places d'hébergement d'urgence, il y en a encore aujourd'hui 198.000. Oui, c'est difficile. Oui, c'est une situation que chaque soir les écoutants du 115, entende écoute et essaye d'améliorer, c'est d'ailleurs pour cela que madame, la Première ministre a souhaité que nous. Mettions en place une prime pour les écoutants du 115, et nous y travaillons. D'arrache-pied pour ce qui est de la situation. Vous le savez avec Charlotte Caubel monsieur comble Ministre Combe. Nous sommes à l'écoute, nous faisons une attention particulière aux familles avec enfants je réunirai encore je crois. L'ensemble des préfets de région pour tenir compte de cette situation, l'ensemble des associations qui sont nos partenaires sur cette situation dramatique sont réunies très régulièrement dans une cellule de crise que nous tenons avec avec la Dial pour que ces situations soit le moins pénible possible et qu'à chaque cas nous trouvions une solution. Rien n'est n'est impossible mais tout est difficile sur une situation aussi dramatique le le la situation géopolitique, vous le savez est particulièrement complexe et un certain nombre de familles en grande urgence sont prises en compte chaque soir en région Île-de-France, par exemple, c'est 45.000 personnes qui sont mises à l'abri et dans l'hébergement d'urgence et nous continuerons à le faire. Merci. Merci, monsieur le Ministre, chers collègues, vous avez 40 secondes pour. Oui, Monsieur le Ministre, vous avez évoqué notamment les les accompagnants du SAMU. Vous avez parlé de confiance mais c'est le Ségur de la santé qu'ils attendent la confiance, c'est bien le Ségur de la santé, c'est encore mieux. Vous avez dressé un tableau avec lequel nous sommes d'accord sur les chiffres de personnes qui attendent. Nous savons qu'effectivement le nombre de places a augmenté depuis quelques années, mais nous savons aussi que la situation s'aggrave pour des raisons que je n'énumère re-pas ici mais que tout le monde connaît et au delà de de ces chiffres que nous vous nous avez annoncé, il est vraiment impératif pour les semaines qui viennent de trouver, voire même pour les jours qui viennent de trouver de nouvelles places d'hébergement. On ne peut pas en France à voir des femmes enceintes et des enfants dehors la nuit.-- Merci cher collègue. La parole est à présent un autre collègue sénatrice Madame Maryse Carrère pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen.-- Merci madame la présidente. Ma question s'adresse à Madame, la ministre Olivia Grégoire et j'y associe ma collègue sénatrice Hautes-Pyrénées Viviane Artigalas. Madame la Ministre depuis désormais 3 ans notre pays traverse de nombreuses crises qui mettent à mal notre économie. Ainsi, après la crise sanitaire dans les collectivités locales et notre économie subissent encore les conséquences. La crise énergétique vient obscurcir le ciel de la reprise au moment de l'année où les besoins en énergie vont être les plus importants. L'intervention de l'État est une fois de plus nécessaire afin de permettre à notre pays de continuer à avancer. Ainsi le 14 septembre, le gouvernement a annoncé le maintien du bouclier tarifaire, puis le 27 octobre il te présenter le dispositif d'amortisseurs, or comme cela s'était déjà produit durant la crise, la crise Covid. Il semblerait que les régies publiques exploite notamment des domaines skiables ou des établissements thermaux ne serait pas éligible à ces nouveaux dispositifs alors qu'elles ont déjà optimiser leur consommation au-delà du soutenable et il est vrai que les régies et notamment les stations de ski verront leurs dépenses triplé et ce ne sera clairement pas supportable. Les régies publiques avait déjà dû faire entendre leur voix durant la crise sanitaire pourrait intégrer dans les mécanismes gouvernementaux de soutien à l'économie et il ne serait donc pas envisageable que cet oubli se répète. Aussi ma question sera simple, la hausse des tarifs énergétiques impactant l'intégralité des consommateurs du pays. Le gouvernement a-t-il bien prévu d'intégrer dans les dispositifs de bouclier énergétique les régies publiques dans leur intégralité et notamment les régies exploitant de remontées mécaniques ou d'établissements thermaux car on ne saurait imaginer qu'en raison de leur statut elle puissent à nouveau être écarté de la solidarité nationale. Je vous remercie. Merci cher collègue. Pour vous répondre madame Olivia Grégoire Ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme.-- Merci madame la présidente, madame la sénatrice Carrère vous évoquez à juste titre. La situation des stations de ski et des stations thermales, dont je sais qu'elles sont comme de nombreux acteurs économiques directement touchés par la crise énergétique. C'est une situation je prends très au sérieux et que je suis au jour le jour avec mon cabinet je ne suis pas étonné que en tant que sénatrice. Vous me posiez la question, sachez que les députés sont aussi très préoccupé, je veux d'abord saluer les efforts de tous et notamment des stations thermales et des stations de crimes de ski en matière de sobriété. On ne le dit pas assez, mais elles ont fait beaucoup d'efforts et aujourd'hui face à la hausse des prix de l'énergie, vous le savez le gouvernement a mis en place tout un type de dispositif d'aide. Je tiens à dire que toutes les structures qui se pose des questions parce qu'il y en a beaucoup et qu'on doit partager l'information tous ensemble peuvent déjà appelé leurs chambres consulaires soit leur CCI ou leur CMA ou alors leur conseiller départemental à la sortie de crise il y en a un dans chaque préfecture de notre pays pour accompagner en matière d'aide aux énergies nos acteurs économiques votre question madame la sénatrice Carrère porte plus spécifiquement sur les aides aux remontées mécaniques et aux stations thermales. Il est prévu que le dispositif d'amortisseurs qui va protéger nos PME et collectivités locales à compter de 2023 sera également ouvert aux régies qui ont la même taille qu'une PME, c'est-à-dire moins de 250 salariés. Je peux totalement vous rassurer, sur ce point je tiens aussi à vous dire que les collectivités locales, vous le savez, bénéficient d'un soutien important avec le dispositif de filet de sécurité qui vient compenser 70% de la hausse des dépenses d'énergie pour les communes, EPCI ou syndicats fortement impacté par la hausse des prix de l'énergie. Les dépenses des régies peuvent être prises en charge dans le cadre de ce filet de sécurité. Et si certaines situations s'avérait mal couvertes. Soyons clairs, je suis à votre disposition pour étudier au cas par cas le cas des régies qui ne rentreraient pas dans le filet pour finir sur une note optimiste. On en a peu, ne nous en privons pas. Le taux d'occupation prévisionnels des stations de montagne pour cet hiver s'annonce supérieure de 7% à celui des des saisons précédentes. Les chiffres des vacances de la Toussaint et les prévisions de Noël nous confirme que nos compatriotes font le choix de la destination France, ce qui est aussi une bonne nouvelle, on a toujours été là, vous l'avez rappelé pendant la crise sanitaire pour les régies les stations thermales et je vous le garantis, madame la sénatrice, nous serons là, je vous remercie. Si Madame la Ministre, chers collègues, vous avez 20 secondes pour répliquer. Merci madame la ministre, votre réponse, ce sera de nature à vraiment rassuré les stations de sports d'hiver, notamment dans les Hautes-Pyrénées, qui ont bondi à, à vue de leur contrat énergétiques multiplié par 3, 60 euros le mégawattheure. En 2021, 170 euros en 2022 au mois de mars 590 euros prévu à cette cette année. Ah au renouvellement. Merci encore pour cette réponse. Merci, cher collègue, la parole est à présent. merci madame la présidente. Ma question s'adresse au ministre du Travail après une concertation de pure forme des partenaires sociaux, vous annonciez récemment une énième réforme de l'assurance chômage avec une réduction de la durée d'indemnité de 25% en période dite favorable la période défavorable qui permettrait de rester aux conditions actuelles d'indemnisation suppose un taux de chômage à 9%, soit un taux que la France n'a pas connu depuis des années cette réforme au prétexte de la cyclicité dégrade donc dès aujourd'hui les conditions d'assurance revenir à 9% supposerait la survenue d'une crise économique majeure, vous annoncez votre confiance dans l'attente d'un taux de chômage de 5% en 2027. Vous devriez en conséquence a minima fixé le seuil au niveau actuel du chômage, soit 7%. La réalité c'est que les prévisions ne valide pas la poursuite de la baisse du chômage et qu'il y a à l'heure à croire, on a possible levier par la baisse de l'assurance. Même en poussant les chômeurs vers des emplois de plus en plus précaire. Pour masquer le véritable objectif de la réforme qui vise à baisser les dépenses re-et réaliser 4 milliards d'économies. Vous affirmez que la contracyclicité permettra le retour à l'emploi de 150.000 chômeurs, quand bien même convenons que cela ne justifierait pas les dizaines de milliers qui perdront leur droit. Mais ma question porte cependant sur ce nombre de 150.000 retours à l'emploi que nous vend votre réforme. D'où vient ce nombre. Monsieur le Ministre, de quel calcul de quelle étude.-- Merci Charles collègue, la parole est à Olivier Dussopt Ministre du Travail, du plein emploi et de l'insertion pour vous répondre. Merci madame la présidente, madame la sénatrice poncer Monge. Permettez-moi d'abord de reprendre les termes de votre question, vous avez dit à l'instant. Pour revenir au niveau de l'indemnisation précédant il faudrait atteindre 9% de chômage, ce que la France n'a pas connu depuis des années. Vous avez raison, la France ne l'a pas connu depuis 5 ans et c'est sous le quinquennat d'Emmanuel Macron que nous sommes passés de 9,4% à 7,3% de chômage. Et vous avez aussi raison de souligner que la politique pour l'emploi que nous menons est une politique efficace qui s'est traduite par la création d'1.700.000 emplois depuis 2017 et encore au 3ème trimestre de l'année 2022 ce sont 84.000 emplois qui ont été créés par l'économie française par les entreprises françaises et parce que je devine que vous allez embrayé si vous me permettez cette expression en disant mais il s'agit de mauvais emplois. C'est la première fois depuis 20 ans que parmi les embauches depuis le début de l'année 2022, plus de la moitié des embauches sont en CDI et c'est aussi la première fois depuis 20 ans que dans le stock d'emplois de l'économie française. Plus de la moitié des emplois sont décédés, donc non seulement année l'économie française crée de l'emploi mais elle crée de l'emploi stable de meilleure qualité qu'il y a maintenant quelques années, c'est aussi le résultat de la politique de lutte contre les contrats courts que nous menons depuis 2019 nous avons porté effectivement une réforme de l'assurance chômage, elle a été adoptée par les 2 assemblées 149 3 je le précise, elle prévoit la contracyclicité. Quel est le principe de la contracyclicité, c'est faire en sorte d'avoir une régime d'assurance chômage qui soit plus protecteur. Quand les choses vont mal et qui soit plus incitatif quand les choses vont bien, c'est ce que nous avons fait, c'est le Sénat qui a introduit la notion de conjoncture économique comme critère de modulation des règles de l'assurance chômage. Nous savons que cette loi, ces dispositions le décret que nous allons bientôt prendre va vont permettre de réduire une part et simplement une part des tensions de recrutement et toutes les études convergent en effet pour dire que, à l'échelle de l'année 2023. Cela peut permettre d'accélérer le retour à l'emploi de 100 à 150.000 personnes. C'est une bonne nouvelle et vous devrez vous en féliciter comme vous devriez vous féliciter du fait que depuis un an, depuis octobre 2021 grâce aux politiques de formation grâce aux politiques de l'emploi, nous avons permis le retour à l'emploi de 300.000 chômeurs de longue durée dans 100 556.000 de très longue durée. Les bonnes nouvelles Madame la sénatrice, vous les oubliez, vous préférez faire peur c'est dommage réjouissent nous avec vous. Monsieur le Ministre. Non le chiffre que vous dites du chômage, vous l'avez trouvé. En 2017, il était là en 2017 effectivement dans la dernière année du quinquennat précédent. Donc c'est pas sous votre mandat que ce chiffre a été atteint. Mais si. De plus, bon vous vous réjouissez. Les chômeurs de catégorie A vous c'est celle que vous voyez mais je termine en disant que de tous ces chiffres, le seul qui est exact, le seul qui est documenté, c'est celui que donne l'Unédic, 4 milliards d'économies faites par cette réforme sur les demandeurs d'emploi. Merci cher collègue. La parole. Est à présent. Un autre collègue monsieur le sénateur Pierre vielle pour le groupe les indépendants République et Territoires pour 2 minutes, chers collègues.-- Merci madame la présidente. Monsieur le ministre de l'Agriculture. Ma question concerne l'influenza aviaire qui continue de sévir dans notre pays et ses conséquences sur la filière palmipèdes avicole cette année d'après ne cesse, c'est une présence endémique du virus ont été victimes la faune sauvage. Alors que les migrations ont à peine débuté la façade ouest et particulièrement touchées, malgré le nouvelles mesures de surveillance inédite. Pensez-vous déjà Monsieur le Ministre, un autre plan, plus protecteur. La filière en raison des abattages massifs évolue aujourd'hui à 30% de ses capacités et les acteurs éprouvent de grandes difficultés d'approvisionnement, même dans les zones indemnes. À la veille des fêtes de Noël, c'est tout un secteur économique qui est plongé dans un profond désarroi. Les aides comme le fonds de mutualisation sanitaire et environnemental s'avère insuffisante et inadaptée à une crise d'une telle ampleur. Alors abattage ou non isolement ou non valorisation ou non, le débat est complexe. Et la seule lueur d'espoir semble venir de la vaccination. Or le vaccin malgré des essais encourageants de laboratoire CEVA et Boehringer n'est toujours pas prêt. Les laboratoires semblent petit peu réticents à investir massivement dans une filière réputée de plus en plus fragiles. Monsieur le Ministre, pensez-vous pouvoir mener une action forte en faveur de la mise en place et du soutien de ce programme de vaccination. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur mais deviennent vous m'interrogez sur la question de la grippe aviaire, qui est un sujet effectivement de préoccupation de préoccupation et de de 13 pour nombre de producteurs. Compte tenu de l'arrivée d'une deuxième vague épidémique puissantes comme celle que nous avons connu en 2022, d'abord vous dire des éléments sur les mesures de gestion qui ont été prises. Vous l'avez rappelé, face à la situation sanitaire dégradée. Des mesures ont été prises, en particulier dans l'ouest. Ce qui est particulièrement touchée en ce moment. Elles ont été regardés. Avec l'ensemble des de la des filières, que je remercie du travail de collaboration qui est le nôtre. Sur ces questions qui sont des questions difficiles ici. Nous avons besoin de renforcer des mesures parfois nous avons besoin et nous pouvons les alléger, nous le faisons à chaque fois que c'est possible, c'est une concertation qui est ajusté chaque semaine pour faire en sorte de faire face à la difficulté des filières 2ème élément. Vous avez parlé. La question des indemnisations. Permettez-moi de dire j'ai j'ai un petit point de désaccord avec vous sur le les montants qui ont été déployés sur l'année 2022 près d'1,1 milliards d'euros qui ont été déployés sur un chiffre d'affaires global de 6,7 milliards d'euros. Je pense que si nous n'avions pas été au rendez vous de ces mesures très puissante. La filière les filières qui sont concernés dans votre région comme dans beaucoup de régions de France aurait tout simplement disparu. C'est vrai que nous sommes en mode encore dégradée qui a un certain nombre de repeuplement qui n'ont pas pu se faire parce que les lieux de la courage ont disparu, enfin vous m'interrogez sur la question de la vaccination. D'abord vous dire que c'est parce que la France a agit que nous avons obtenu une expérimentation et donc tout, tout le monde connaissait le calendrier, le calendrier c'est une expérimentation. Autorisation obtenue en juin expérimentation démarrer en août en particulier sur les palmipèdes en France ces 5 pays qui expérimente, nous attendons la qualification de la vaccination au tournant de l'hiver en décembre et en janvier et sans plus attendre sans connaître précisément encore les résultats de ce vaccin nous travaillons déjà un plan de vaccination qui permettra effectivement de redonner de la perspective à nos éleveurs gérer l'urgence réfléchir au moyen et long terme, c'est bien ce que nous avons à faire et ça permettra aussi que les laboratoires qui seront chargés de produire ce vaccin puis se mettent en situation de le faire dans des conditions de délai qui soit raisonnable pour la saison, évidemment 2023 et donc on est à l'oeuvre sur l'urgence et aussi sur le moyen long terme la vaccination étant l'un des moyens mais pas le seul, vous le savez aussi bien que moi. Merci monsieur le sénateur.-- Merci. Cher collègue, vous avez moins de 40 secondes pour.-- Merci, monsieur le Ministre pour ses réponses sur la vaccination. Bon vous êtes conscient qu'au moment de la fragilité aujourd'hui de la filière donc. Je crois, les aider à tenir jusqu'à la campagne de 2023. On peut se poser des questions sur l'opportunité de de certains abattage à partir du moment où il a interdiction de transport. Je crois que toutes les mesures qui iront en faveur de de de de cette filière pour la faire retenir seront les bienvenues et nous attendent bien sûr des bonnes nouvelles du du côté de laboratoires et si le gouvernement en plus si on peut vacciner de façon anticipée, je crois que ce sera parfait et très bien Merci, cher collègue, la parole est à présent à notre collègue sénatrice Madame Laurence Garnier pour le groupe Les Républicains. Merci madame la présidente. Ma question s'adresse à la Première ministre. Madame la Ministre le 19 février 2020. A été pour vous un jour historique, c'est ce que vous avez déclaré en annonçant tout sourire la fermeture effective de Fessenheim. Quelques mois avant le président de la République, il avait annoncé sa volonté de fermer 14 centrales nucléaires d'ici à 2035.-- Depuis. Vous avez réussi le double exploit d'augmenter. Notre besoin en électricité est de diminuer notre production vous augmentez nos besoins. En achetant des voitures électriques à la Chine. Et vous diminuer notre production en sabordent notre parc nucléaire par vos changements de pieds successifs au gré des arrivées et des départs des ministres écologistes. Madame la Ministre la guerre en Ukraine. Loin d'expliquer la crise actuelle n'a fait que révéler. Vos propres insuffisances et aujourd'hui ce sont les Français qui vont devoir subir une pénurie dont vous êtes responsable. Alors on rouvre. Nos centrales à charbon polluantes. Je pense à Cordemais, en Loire-Atlantique dont la fermeture n'en finit pas d'être reportée. Et puis surtout on prépare les Français au grand bond en arrière en leur parlant. Fermetures d'écoles délestage. Et baisse de tension en moins de 3 ans madame, la Première ministre en moins de 3 ans. Vous avez réussi à remplacer la stratégie énergétique française par un catalogue de bonnes pratiques de doudounes et 2 cols roulés alors Madame la Ministre jusqu'à quand comptez vous infantiliser les Français pour masquer votre impréparation et vos compromissions. Merci. Pour vous répondre, monsieur Roland Lescure. Ministre délégué chargé de l'industrie. Merci madame la présidente, madame. La sénatrice Laurence Garnier. Je suis doublement surpris de votre question. D'abord D'abord parce que vous vous semblait remettre en cause une stratégie de développement énergétique qui dont nous avons une occasion discuter ici au Sénat, dans le cadre d'un débat article 50 tirer hein. Dans le cadre duquel j'avais eu l'occasion de rappeler que la période dans laquelle les centrales nucléaires en France ont été le moins entretenu conduisant du coup à un taux d'occupation des centrales nucléaires, le plus faible historique, c'était sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. J'aimerais pouvoir affirmer que face à un défi historique. Celui de la décarbonation de la France face à un défi historique qui est la guerre aux portes de l'Europe. face à un défi historique qui est oui de restaurer la crédibilité de notre grand opérateur national et de l'amener vers l'avant. Le développement de nouveaux réacteurs. Vous l'avez dit, la fermeture de centrales à charbon difficile dans certains territoires comme le vôtre, nous serions capables de créer de l'unité nationale face à ça, je regrette que nous soyons dans la gestion des peurs. Face à ça, je regrette que nous soyons dans la gestion de la caricature, vous le savez ce gouvernement est extrêmement mobilisés de manière à éviter le pire, le pire, ce serait des délestages sur lesquels nous travaillons jour et nuit avec l'opérateur pour les éviter. J'en appelle à la responsabilité des Françaises et des Français qui le savent et qui réduisent aujourd'hui leur consommation d'électricité pour faire face aux défis. J'aimerais que tout le monde soit aussi responsable que les industriels français aujourd'hui qui depuis des mois réduisent leur consommation d'électricité. Merci. Merci, monsieur le Ministre, la parole. État présent à notre collègue monsieur le sénateur Michel Laugier pour le groupe Union centriste. Merci madame la présidente, madame, la Première ministre et mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question plutôt mes interrogations s'adresse à monsieur Ministre de la Santé à propos d'un sujet déjà évoqué en début de séance au mois d'août dernier, l'hôpital de Corbeil-Essonnes ne subissez une super attaque sans précédent. Samedi soir, c'est l'hôpital de Versailles qui a été victime d'une attaque similaire. Une cyberattaque d'une telle ampleur qu'il a eu des conséquences immédiates sur la prise en charge des patients avec des déprogrammations d'opérations et des transferts vers d'autres hôpitaux. Pendant peut-être encore plusieurs mois, le plus grand hôpital de soins des Yvelines ne fonctionnera au ralenti détériorant l'offre hospitalière et l'accès aux soins de tout le département, confronté à une crise majeure depuis plusieurs années, l'hôpital déjà au bord de l'implosion et qui c'est-à-dire semaine est confronté à l'afflux de malades touchés par les épidémies de bronchiolite Covid et grippe doit dorénavant faire face à des attaques informatiques qui s'apparente, ni plus du moins à du terrorisme. Comment cette attaque d'pas pu être déjoué alors qu'à la suite de plusieurs tentatives. On savait que cet hôpital était visé. Comment cette cyberattaque a-t-il pu se produire après celle de Corbeil-Essonnes visiblement aucun enseignement n'a, n'a été tiré aujourd'hui les patients et les personnels soignants attendent un retour rapide à la normale et la conclusion de l'enquête sur l'identification. Des hackers où en est-on. Plus généralement, quel est le degré de fragilité des administrations françaises au cyberterrorisme. Et quelle est la doctrine gouvernementale face aux demandes de rançon. Enfin quel dispositif allez vous mettre en place pour dissuader toute nouvelle tentative de déstabilisation de notre système hospitalier et plus largement de nos administrations.-- Je l'ai dit, cette attaque et et vous l'avez dit également être ignoble elle tente de prendre en otage la santé des Français. Tous nos hôpitaux plus largement les administrations font face à cette nouvelle menace cette cybercriminalité qui cherche avant tout à s'enrichir en s'en prenant à nos infrastructures essentielles. Les attaques malheureusement évolue au fur et à mesure que des moyens de protection évolue également pour protéger nos établissements.-- Vous avez parlé de rançon éventuelles, je le redis à nouveau avec la plus grande détermination. Nous ne céderons jamais. En ce qui concerne la santé des Français, bien entendu. Le problème est pris plus qu'au sérieux chez rappelé des financements dont nous avons mis en place la coordination qu'il y a entre les différents ministères à ce sujet. À ce jour 150 établissements groupements hospitaliers ont déjà bénéficié sont accompagnés dans le cadre du plan parcours cybersécurité. Je tiens surtout à rassurer nos concitoyens, la sécurité et la qualité des soins sont toujours garanti. Effectivement il y a une déprogrammation immédiate tant qu'on ne connaissait pas l'ampleur de l'attaque. Il y a eu également je vous le confirme mercredi 6 transfert au total à titre préventif pour faire de la place au cas où 3 enfants et 3 adultes vers les autres hôpitaux de l'Île-de-France, en particulier l'AP-HP que je salue ici. En attendant le traitement des patients admis se poursuit bien entendu avec un mot de papier en étant obligé de se déplacer d'un service à l'autre, en particulier en ce qui concerne l'imagerie et et la biologie médicale. Mais en tout état de cause, notre capacité à assurer la sécurité et la continuité des soins est essentiel bien sûr pour protéger nos concitoyens mais aussi pour diminuer l'emprise des pirates en diminuant l'attractivité de nos établissements. La stratégie elle est donc global. Prévenir les cyberattaques bien entendu en renforçant de plus en plus les moyens de protection des établissements mais aussi limiter l'impact de ces attaques pour rendre, je le disais, nos établissements moins attractif. Vous parliez des épidémies qui tape l'hôpital, j'en profite juste très rapidement pour rappeler dans cette assemblée finalement l'importance de la vaccination et du port de masque en notre en endroit clos. Je vous remercie. Merci Monsieur le Ministre, vous avez une poignée de secondes chers collègues pour répondre si vous le souhaitez. Une poignée Il y a quelques semaines et dans cet hémicycle à une question sur la sécurité. Le ministre de l'Intérieur m'avait dit. Et à la fin, c'est toujours la police qui gagne. Le problème c'est qu'on ne voit jamais la fin.-- Merci cher collègue. La parole est à présent au sénateur Pierre Ouzoulias pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en septembre 2020, le président de la République célébrer la France comme le pays des lumières et de l'innovation et raillé ceux qui préféraient le modèle Amish et le retour à la lampe à huile. Cet hiver, la France des Lumières va basculer en mode. Et s'éclairer à la lampe à huile et elle a bougé. notre pays qui était exportateur d'électricité il y a peu, va maintenant dépendre de ses voisins pour tenter de continuer à alimenter en électricité ces transports, ces services publics, ses industries, ses entreprises et cetera. Comment a-t-on pu en arriver là, comment la 7ème puissance économique mondiale a-t-elle pu devenir en si peu de temps un pays en voie de sous-développement. Ces pénuries vont rappeler aux générations les plus anciennes, les privations de l'après-guerre et les tickets de rationnement. Elle frappe d'effroi. Les plus jeunes qui prennent. Ainsi conscience du déclassement. Inéluctable de notre pays. Que les thuriféraires de la décroissance, se réjouissent. Nous y allons à grands pas. La start-up nation n'a plus de jus. Dans la France en pénurie, comme dans le radeau de la méduse. Le gouvernement en est réduit à tirer à la courte paille ceux qui vont être sacrifiés et comme dans la chanson, ce sont les plus jeunes qui ont été choisies ainsi comme vous nous l'avez annoncé dans cet hémicycle. Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale Les écoles pourront être privés d'électricité mais nous sommes rassurés. Les parents seront prévenus par le préfet la veille à 19h. La crise pandémique a durement touché toute la jeunesse de la maternelle à l'université. Monsieur le Ministre. Qu'allez-vous faire pour qu'elle ne soit pas de nouveau la victime de politique qui les ignore. Monsieur le Ministre préserver notre jeunesse. Merci cher collègue. La parole est donnée à monsieur.

Merci madame la présidente. Mesdames, messieurs les sénateurs et sénatrices. Merci pour cet accueil.-- Et Monsieur le Sénateur merci pour votre question. Je Je pense qu'aujourd'hui. Je l'ai dit tout à l'heure avec un ton particulier peut être lié à celui de la question qui m'avait à telle adresse. C'est mais je souhaiterais vraiment vraiment. Sincèrement et solennellement. a appelé à la mobilisation générale. Aujourd'hui, nous le savons. Nous faisons face tous et toutes à une guerre aux portes de l'Europe. nous faisons, nous le savons. Face à un défi de production de la part de notre père international et je voudrais saluer à la fois le nouveau PDG Luc Rémont et à travers lui l'ensemble des salariés d'EDF qui se mobilisent, jour et nuit pour faire en sorte qu'on puisse, comme il nous le dit livrer watts. Hé oui mesdames et messieurs les sénateurs, il se peut que dans des cas extrêmement particulier. Dans un, dans un environnement climatique extrêmement particulier on puisse mettre en place des délestages ciblées. Hé Hé mesdames et messieurs les sénateurs, et monsieur le sénateur, vous le savez. Le plan de prévention a été extrêmement calibrée. L'application EcoWatt permet de prévenir ces délestages bien en avant. Je vous le dis et je vous le rappelle, au cas où la météo deviendrait orange ou rouge. Chacun d'entre nous doit faire les efforts pour limiter sa consommation. Et au cas où très peu probable, les écoles viendrait à en être affecté. Je l'ai confirmé avec mon collègue de l'Éducation nationale. Ce sont bien 3 jours auparavant, que les parents en seront prévenus. Mesdames, et messieurs les sénateurs, les sénatrices. Pour éviter le pire, le meilleur, c'est quand même de s'y préparer. Nous y sommes prêts. Nous l'éviterons merci. Merci, monsieur le Ministre.-- La parole est à présent à notre collègue Madame Jacqueline Eustache-Brinio pour le groupe des Républicains. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre. Armés de machettes coupe coupe ou simplement de tessons de bouteille des jeunes livrés à eux-mêmes font régner un climat de terreur dans le 100 unième département français. Bande violence alcool mains coupées, guerre de gangs caillassage des voitures de police, la liste est longue de tous les fléaux que subissent les Mahorais depuis longtemps. Livrés à eux-, mêmes des milliers de jeunes mineurs isolés sans-papiers Peuple des bidonvilles à Mayotte sans avenir ces jeunes hors la loi n'ont rien à perdre et menace la société tout entière. Sa spirale infernale n'est pas prêt de s'arrêter puisque, sous la pression migratoire. La maternité de Mamoudzou débordé, tout comme le bureau des titres de séjour. On en voit le raid pour calmer la situation, mais il faudrait davantage de moyens pour mettre fin à cette terreur. La politique du pansement ne suffit plus. La vie de tous les Mahorais en danger par cette immigration incontrôlée. Nous ne pouvons pas accepter d'offrir un tel avenir aux habitants de Mayotte, qui ont fait le choix de la France. Monsieur Darmanin va se rendre à Mayotte, à la fin du mois. Pouvez-vous nous garantir que les soit qui seront formulées pour 2023 2 seront pas des voeux pieux. Serez-vous en mesure de garantir aux habitants de cette île. Le respect des lois et principes de la République française en dénonçant clairement les causes de ce désordre et c'est de cette ultra-violence.--

Effectivement.-- Vous l'avez dit, ces actes sont inacceptables. La mobilisation.-- Du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Et totale. vous connaissez les moyens qui sont mis en oeuvre. Au moins, reconnaissez-le. Monsieur le ministre de l'Intérieur se rend. À Mayotte en décembre il confirmera les engagements qui sont pris. S'agissant de la lutte contre l'immigration clandestine. Je voudrais simplement dire que 24.000 étrangers en situation irrégulière ont été reconduits à la frontière l'an passé, soit 78% de plus qu'en 2020 324. Passeur. 324 passeurs ont été présentés injustice. Quatre filières ont été démantelées. La loi sur l'immigration qui sera présentée bientôt au Parlement j'hein La loi qui sera présenté au Parlement répondra à un certain nombre de vos demandes. J'en suis sûr mais ce qui compte, mais ce qui compte, que vous passez sous silence, c'est l'effort extraordinaire que madame, la Première ministre a autorisé monsieur Darmanin et moi-même à mettre en oeuvre sur le développement sur le développement est ce que vous savez que 83 millions d'euros sont dépensés en 2023 sur l'éducation nationale. Est-ce que vous savez que j'ai signé un contrat de 411 millions d'euros sur l'eau avec l'eau de Mayotte. Est-ce que vous savez que Monsieur le Ministre Brown. Il a été et a été ahuri des efforts faits en innovation su en matière de santé, en matière de développement économique. Ce que vous dites madame la sénatrice, ce que vous dites est une. J'allais dire une insulte aux élus de mal de Mayotte qui eux se mobilisent. Merci, monsieur le Ministre.-- Vous avez de 33 secondes pour répliquer, chers collègues. Ah réponse très facile très facile Monsieur Miss. Le préfet du département estime que si on ne fait rien il y aura 750.000 habitants à Mayotte en 2050. Ils sont aujourd'hui 300.000. Alors Monsieur Ministre, êtes-vous prêt à entendre. Que le droit du sol que les politiques publiques en matière d'accès aux soins gratuits et à l'hosto. Les actions des enfants doit être. Mince drastiquement pardon remis en cause sur ce rite sur ce territoire. Je rappelle que 80% des enfants scolarisés à Mayotte ne sont pas des enfants de Lille

Je voudrais juste finir Madame la présidente, madame, la Première ministre Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame, la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national service national universel. Madame le ministre, votre budget 2023 attribue 140 millions d'euros au service national universel, les laissant des crédits dérisoires pour les autres dispositifs du soutien à la vie associative et pourtant, nous savons tous ici, que le service national universel est un échec. Depuis sa création en 2019. En 2022, vous vouliez 50.000 jeunes. Comme les années précédentes. Nous vous avions fait part de notre scepticisme et au final ce sont seulement 32.000 services qui seront réalisés. Il est évident que les jeunes n'adhère pas à ce projet imaginé promue et soutenue par le président de la République qui doit rester aujourd'hui le seul convaincu de son intérêt. Et malgré cela vous augmentez encore ce budget pour 2023, inscrivant 140 millions en espérant 64.000 jeunes, 27% d'augmentation pendant que les crédits du service civique progresse moins que l'inflation alors que c'est un outil très pertinent pour les jeunes et qui aujourd'hui est très recherché, vous le savez madame la ministre, la généralisation du SNU à une classe d'âge sera très difficile, autant pour des raisons budgétaires que pour des raisons d'adhésion. Madame la ministre, il faut savoir tirer les leçons d'un échec. D'autres solutions existent pour l'éducation et la à la citoyenneté de notre jeunesse. Pourquoi ne pas soutenir vraiment le développement du service civique ainsi que les colonies de vacances. Vrai lieu de mixité et de socialisation dès le plus jeune âge et promouvoir le BAFA qui pourrait faire partie d'un parcours d'engagement et de citoyenneté qui se déploierait à bien moindre coût en apportant un vrai soutien à la vie associative dans notre pays. Madame le ministre aujourd'hui, on attend vos propositions. Votre ministère répondre, a-t-il enfin aux aspirations et aux besoins de notre jeunesse. Merci, cher collègue, la parole est à madame Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel.-- Merci beaucoup madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le rapporteur, Mani j'ai la conviction que nous ambitionnons la même chose pour nos jeunesse. C'est-à-dire une jeunesse qui a goût en l'avenir qui est formé qui a de l'espérance et pour ça, monsieur le sénateur, aucune opposition entre les dispositifs le service civique augmente. Il a même, il y a même plus de missions et d'agrément que de jeunes face vos missions proposées. Plus que jamais nous avons investi sur le service civique. Les colonies de vacances. L'éducation populaire augmente vacances à prenante un million de l'été encore dernier le BAFA Installation du comité de filière BAFA financement massif avec plus de 200 euros pour chaque jeune qui le souhaite pour lever le pour lever le frein financier monsieur le sénateur, à aucun moment, ni dans votre esprit, ni dans le mien nous opposons les dispositifs de nos jeunesse par contre ce qui est certain c'est qu'il est nécessaire de construire un parcours de citoyenneté, il ne se décrète pas. Nous avons aujourd'hui une jeunesse qui pour une partie d'entre elles et fracturé. Nous avons besoin d'unité de bilan de santé. Un parcours qui fait que notre abstention recule. Nous avons besoin d'une jeunesse qui retrouve la culture de la défense, nous avons besoin d'une jeunesse formés aux gestes qui sauvent. Nous avons besoin d'une jeunesse à qui on propose un projet pour elle d'abord qu'il l'a fait grandir en complémentarité du projet pédagogique de l'éduquer, de l'éducation civique et morale. Mais nous avons aussi besoin d'une jeunesse qui s'engage et votre famille politique, monsieur le sénateur porte ses engagements qu'ils soient civils ou militaires. Alors avec le ministre de l'Educational, le mystère de la. Le ministre de désarmer sous l'autorité de la Première ministre nous déployons avec beaucoup d'apprentissage, année après année, un grand projet pour notre jeunesse, dans laquelle nous investissons parce que un pays fort un pays uni doit préparer sa jeunesse à répondre aux défis de notre temps le. Guerre en Ukraine aujourd'hui défi climatique majeur, comment les formes face aux catastrophes naturelles. Et puis enfin monsieur le sénateur, un pays uni, c'est une jeunesse qui se parlent et qui partagent des valeurs, et pour ça il faut qu'elle se rencontrent le SNU. C'est pour le, c'est pour eux, pour les autres et c'est pour la France. Toutefois, vous n'avez pas répondu sur ma question du service civique sur du service national universel. Allez-vous continuer, allez vous le réformer. Allez-vous modifier sa façon de se développer. Merci la parole est à présent à notre collègue sénateur monsieur Alain Cadec pour le groupe des Républicains. Ma question s'adresse à monsieur le ministre chargé du commerce extérieur. Tout indique que la Commission européenne va initier rapidement le processus de conclusion formelle de l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur. Et de le faire sur une base juridique qui prévoit une décision à la majorité simple au Conseil après approbation du Parlement européen, sans aucune implication des parlements nationaux.-- La France a longtemps justifié son opposition à cet accord en invoquant l'insuffisance des engagements pris par le Brésil du président Bolsonaro en matière d'action climatique et de lutte contre la déforestation. Mais de ce point de vue l'élection récente du président Lula change la donne et ouvrent la voie à la jonction d'une annexe environnementale à l'accord contenant les garanties exigées par l'Union de la part du Brésil.-- L'Allemagne d'une part et le Brésil. D'autre part, ont de grands intérêts dans l'affaire, la première pour doper ses exportations industrielles vers l'Amérique latine, le second pour obtenir un accès préférentiel au marché agricole de l'Union. Il pousse donc l'un et l'autre pour faire en sorte que l'accord puisse entrer en vigueur dès le début de l'année prochaine. Dans ces conditions, monsieur le Ministre. Que que que compte faire la France pour s'opposer à un accord dramatique pour nos intérêts agricoles, sachant qu'un blocage français à Bruxelles ne pourra bientôt plus être justifié seulement par des arguments environnementaux et qu'il ne sera de toute façon plus possible techniquement compte tenu de la base juridique retenue par la commission. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Olivier Becht, Ministre délégué chargé du commerce extérieur de l'attractivité et des Français de l'étranger.-- Merci beaucoup madame la présidente. Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, Kadek. Oui vous avez raison, l'élection du président Lula est une bonne nouvelle pour la relation bilatérale entre la France et le Brésil et le président de la République l'a saluée comme telle.-- Oui, l'accord du Mercosur. Est en négociations depuis l'année 2000, ça fait donc 22 ans que cet accord est en négociation entre l'Union européenne et le Brésil. Et il n'est à ce jour ni ni fidéliser ni signé et a fortiori pas ratifié. La France a posé des conditions très claires pour la conclusion de cet accord. Elles sont de 3 ordres. La première, c'est la question de la déforestation et il y a lieu de saluer d'ailleurs. La conclusion avant hier dans le cas du trilogue européens du règlement sur la déforestation. Il est hors de question d'importer il y a un seul kilo de boeuf.

derrière la déforestation. C'est le respect par toutes les politiques publiques des pays membres du Mercosur des accords de Paris qui a et la 3ème c'est le respect de l'ensemble des normes sanitaires et environnementales de l'Union européenne et c'est donc dans ce cadre-là que les négociations se poursuivent. Le jour où elles auront abouti et je dis cet accord et se prononcera dans le cadre de la procédure européenne au sein du Conseil de l'Union européenne et le Parlement sera évidemment saisi le Parlement européen dans le cadre de ses pouvoirs ou les, ou les parlements nationaux. Si les accords devaient être scindé, je vous remercie. Merci, monsieur le Ministre, chers collègues, vous avez 35 secondes pour. Je vous ai précisé que la Commission européenne, elle a utilisé l'article 207 du traité et elle ne. Consultera pas les parlements nationaux. Cela étant. Certains députés européens Renaissance dans une lettre au commissaire Dombrovskis. Ont ont prétendu que la procédure choisie par la commission n'était. Était illégal. C'est pas vrai, elle n'est pas illégale, elle est parfaitement légal, et compte tenu de la promo l'approbation requise du Parlement européen. Elle ne peut être qualifié d'outrage démocratique. Donc Monsieur le Ministre. La France est en grande difficulté sur ce dossier et surtout nos agriculteurs.-- Merci cher collègue.-- La parole est à présent à notre collègue Madame la sénatrice Annick Jacquemet pour le groupe Union centriste. Merci madame la présidente. Mesdames, et messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de la Santé. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran est intervenu ce matin à la télévision sur le problème de la tension sur les stocks de Doliprane. Il a tenté de rassurer nos concitoyens en expliquant que la France n'était pas seul concerné que la tension était mondiale. Peut-être mais elle dure depuis quelques temps et touche maintenant les enfants début novembre. Notre collègue Bruno Belin soulever, déjà le problème vous avez alors répondu, prendre la mesure de la situation et vouloir augmenter le volume des stocks et les moyens d'alerte. Aujourd'hui c'est le Doliprane pédiatrique qui pose problème. Alors que le froid est arrivé et avec lui les épidémies saisonnières. Nous sommes en rupture. L'impact est particulièrement problématique car pour le traitement des enfants le Doliprane est le médicament de première intention, il n'existe aucun substitut d'après l'Agence nationale de sûreté du médicament. L'ibuprofène et l'aspirine leur sont contre-indiqués. Le principal fabricant Sanofi en situation de quasi-monopole avec 98% des parts de marché sur la présentation pédiatrique est en grande difficulté, aucun concurrent ne peut suppléer à la baisse de sa production. Toujours selon la MCM ces tension pourrait encore durer plusieurs semaines. On ne peut pas laisser les choses en l'état, car outre les difficultés posées en ambulatoire par ces pénuries. L'effet domino sera inévitable. De plus en plus d'enfants seront orientés vers les hôpitaux en particulier les services d'urgence, alors qu'ils sont déjà saturés. Monsieur le Ministre, à court terme comment votre gouvernement entend-il garantir que nos enfants ne manqueront pas de Doliprane pédiatriques cette hiver à à plus long terme comment comptez-vous éviter que de telles situations ne se reproduisent. Je vous remercie.-- Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Jacques mais je vous prie d'abord d'excuser le ministre de la Santé, qui comme l'a vu comme vous l'avez vu, a dû s'absenter. C'est donc le ministre de l'industrie qui vous répond. Qui vous répond d'abord que. Cette pénurie. Vous l'avez dit et mondiale, elle est liée à une volatilité de la consommation de médicaments en général et de paracétamol en particulier. Extrêmement importantes liées à la crise de la Covid qui a modifié de manière importante évidemment les comportements de consommation à la distribution entre la ville et. L'hôpital. La France a réagi parmi les plus rapidement, liée à un système d'alerte qui s'appelle transmettre, qui nous a permis d'identifier ces tensions réelles que vous mentionnez très tôt qui nous a permis de prendre des décisions notamment l'axe la porte l'interdiction d'exportation le passage privilégié par les grossistes répartiteurs qui permet d'assurer du mieux possible la distribution dans les pharmacies mais qui, vous l'avez dit, dans certains cas particuliers n'empêche pas certaines pharmacies mais j'insiste bien, nous n'avons pas aujourd'hui face à nous une panne une pénurie de Doliprane. Quel qu'il soit d'ailleurs mais c'est dans certaines pharmacies. Il est vrai. Que le Doliprane dont vous mentionnez l'absence être vient à manquer. Et donc, hein. Évidemment j'engage les patients qui cherche du Doliprane pour les enfants aujourd'hui malheureusement à chercher dans plusieurs pharmacies

aux fournisseurs de flacons et de verre sur lequel, on me dit que la situation s'améliore et donc votre réponse de court terme c'est ça s'améliore chercher dans les pharmacies attenante mais on va se sortir du problème à moyen terme, évidemment,

c'est l'entreprise séquence qu'il produira et donc pas l'entreprise que vous mentionnez, monsieur le sénateur, mais nous travaillons pour que à nouveau la France soit un terrain un terrain De consommation et pourquoi pas d'exportation. Un jour de médicaments. Merci. Merci, monsieur le Ministre, la parole est à présent à notre collègue Madame la sénatrice Annick Petrus. Pour le groupe des Républicains. Madame la présidente, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'Économie, des Finances, de la souveraineté industrielle et numérique. La direction générale des douanes et des droits indirects joue un rôle propre pondérant dans la sécurité des Français. En effet, les douanes sont entre autres un acteur majeur de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Elles sont ainsi à l'origine de 60 à 80% de saisie de stupéfiants sur le territoire national. De plus si le rôle de la douane de la lutte contre le trafic de stupéfiants est encore trop souvent sous-estimé. Il est pourtant amené à se renforcer ce trafic est resté dynamique et là et a peu souffert de la crise sanitaire. La menace liée au trafic de stupéfiants ne cesse de s'accroître, augmentation des flux et des saisies. Hausse de la criminalité connexes vulnérabilité de nos ports et aéroports la consommation demeure également très élevé sous le un vrai enjeu de santé publique. La situation apparaît désormais critique en France du fait de des multiples voix d'entrée sur le territoire. Trafic maritime en provenance d'Amérique du Sud mais aussi échange tu restes avec les pays frontaliers feraient postal et Express dans l'ensemble du monde nos territoires ultramarins comme c'est Martins sont donc particulièrement vulnérables, il doit faire l'objet d'une attention spécifique du fait de leur situation géographique à la croisée d'importantes routes maritimes et aériennes vers l'Union européenne c'est Martin, je vous le rappelle, ça situe bel et bien au sein du territoire douanier communautaire malheureusement aujourd'hui sur mon territoire. Il ne nous ne bénéficions d'aucune protection face à ces trafics. Faute d'effectifs, avec seulement 2 douaniers à ce jour un poste sur l'île. C'est un effectif clairement insignifiant pour un territoire de près de 53 km2 et d'une zone économique exclusive de près de 300 km2. Alors ma question est simple, allez-vous laisser la France ouverte à toutes sortes de trafics. Car voyez-vous, Monsieur le Ministre, c'est Martin c'est aussi la France, je vous remercie. Merci cher collègue. Pour vous répondre, monsieur Jean-François Carenco, Ministre délégué chargé des Outre-mer. Madame la sénatrice.-- Madame la sénatrice. Vous savez, le problème n'est pas spécifique à Saint-Martin Saint-Barth. Ni alors ni aux îles de la caraïbe. Le trafic de drogue et partout et le trafic de drogue, le gouvernement essaye de lutter partout notamment en Guyane où je me rends à la demande du ministre de l'Intérieur, la semaine prochaine. C'est une priorité du ministre de l'Intérieur qui s'est rendu en Guyane notamment et à la Martinique mais qui a évoqué l'ensemble des sujets de la caraïbe avec monsieur Attal, le ministre en charge des douanes avec monsieur le ministre de la justice. Ne doutait pas que globalement ce sujet est pris en compte par le gouvernement dans la pratique dans la pratique ça veut dire qu'il nous faut coordonner l'action de l'État en mer sous l'autorité du préfet de zone de la Martinique. travaux sont en cours entre l'ensemble des administrations sur l'autorité de la Première ministre. Globalement, cela veut dire que j'ai demandé pour Saint-Martin pardon spécifiquement. À de renforcer à Saint Barth à Saint-Martin. Les postes de douane qui ont disparu. Il est vrai, il y a quelques années, la discussion est en cours avec le ministre en charge des douanes. Nous avons vous le savez, vous voyez ce bateau telle qu'il ait récemment mis en oeuvre une un bateau des douanes.-- J'en avais jamais vu d'aussi gros et il est désormais et il est désormais complètement à la manoeuvre. Donc, ne doutez pas. Monsieur le ministre Atal répondra j'en suis sûr favorablement à votre demande. Je n'en ai parlé encore il y a quelques jours. Merci, monsieur le Ministre, la parole est à présent à monsieur le questeur Jean-Pierre Sueur pour le groupe socialiste écologiste. Et. Républicain monsieur le questeur fille. Merci madame la présidente, monsieur le garde des Sceaux la surpopulation dans les prisons a atteint un niveau que nous n'avions jamais connu il y a aujourd'hui 1350 personnes qui sont dans des cellules, où il y a 3 détenus et qui dorment sur des matelas par terre la situation est telle que la France a été condamnés pour indignité par la Cour européenne des droits de l'homme. Ma question est très simple, monsieur le garde des Sceaux qu'allez-vous faire.-- Par rapport à cette situation, dans les mois qui viennent.-- Merci monsieur le Keiser la parole. Est à monsieur Éric Dupond-Moretti Garde des Sceaux, ministre de la justice. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs, Monsieur le Sénateur sur. Ça n'est pas la première fois que vous me posez la question. D'abord je voudrais vous dire que c'est la démonstration cette surpopulation carcérale. Que ni la politique pénale, que je conduis, sous l'égide de madame, la Première ministre ni la justice. Contrairement à ce que certains disent qu'en permanence n'est laxiste. Deuxièmement, vous le savez, vous n'êtes pas le seul à être préoccupé par la question. J'ai porté avec beaucoup de force la proposition sénatoriale de Monsieur. Le Président Buffet sur les conditions indignes. Quels sont les leviers que nous avons et je voudrais vous dire d'ailleurs que c'est une gageure de répondre à cette question aussi complexe en 2 minutes. Mais quels sont les leviers rénovation d'abord et de ce point de vue, je voudrais vous dire sans triomphalisme que vous consacriez par 70 millions d'euros rénovation nous consacrons plus de 170 millions par an rénovation construction de places de prison 15.000 places. Elles seront construites, je le dis, nous en avons la moitié en 2024 et nous continuons. 15.000 places mais ensuite il y a bien sûr rappeler aux procureurs généraux la loi peine ce que je fais dans toutes mes circulaire mais également bien sûr développer les peines alternatives, notamment le travail d'intérêt général. Lutter contre la récidive. J'étais hier avec le sénateur Bourgi nous avons inauguré une SAS structures d'accompagnement à la sortie. C'est un établissement pénitentiaire mais c'est aussi une structure qui permet d'éviter la récidive. Et bien sur la prévention. Ce matin j'ai reçu la délégation. la délégation du droit des femmes du Sénat qui m'a remis un rapport absolument extraordinaire sur la pornographie. Et ce rapport a le mérite de mettre cela dans le débat public des enfants de 11 ans, c'est la moyenne d'âge ont accès librement à la pornographie. Hé ben lutter contre ça efficacement c'est naturellement lutter contre la délinquance et si tu aussi régler la question de la surpopulation carcérale.-- Merci monsieur le garde des Sceaux, monsieur le questeur, vous avez un peu plus d'une minute pour répliquer si vous le souhaitez.-- Monsieur le garde des Sceaux, je ne vous ai pas interrogé sur la pornographie qui est en effet un fléau. Monsieur le garde des Sceaux. J'espère que vous avez lu le rapport des états généraux de la justice. Qui a été remis, qui vous a été remis par Monsieur Jean-Marc Sauvé. Vous lirez dans ce rapport que depuis 30 ans. On construit des prisons et la surpopulation 2 décroît pas pour autant. Oui et le rapport dit que la réponse n'est pas essentiellement la mais la réponse elle est dans une régulation. Le mot et dans le rapport. Simplement cette régulation, il faut la penser la réfléchir avec l'ensemble des acteurs concernés et nous aimerions que vous, vous pensiez là-dessus, sur la mise en oeuvre de cette régulation. Ce que pour le moment vous ne faites pas. comme toujours que c'est la faute à avant on connaît et qu'il faut des peines alternatives, l'aménagement des peines et caetera mais on ne sent pas la volonté de répondre au jugement qui condamne la France parce que l'indignité, elle est réelle dans un certain nombre de nos prisons 150% de surpopulation dans 36 d'entre elles, et si on n'agit pas. Fortement dans ce sens, hé bien on ne prépare pas la réinsertion, car cet état d'indignité dans les prisons, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de réinsertion et donc récidive. Chers collègues, merci.-- La parole est à présent à monsieur Guillaume Chevrollier pour le groupe des Républicains. Monsieur le sénateur, vous avez 2 minutes.-- Merci madame la présidente, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse au 1er ministre. Après la COP27 sur le climat, qui n'a pas été satisfaisante. La COP15 sur la diversité biologique est ouverte depuis hier. Apportant avec elle l'espoir d'un possible accord ambitieux permettant d'enrayer le déclin de la biodiversité. Nous le souhaitons tous ici tant le Sénat est mobilisé sur les questions de biodiversité et de climat qui sont liées. Je salue d'ailleurs l'accord européen qui vient d'être trouvé sur l'interdiction d'importation des produits liés à la déforestation. Un enjeu majeur pointés par la chambre haute. Cette COP 15 instaure indique indéniablement un dialogue utile entre les gouvernements en lien avec les citoyens et les entreprises. Face au taux d'extinction des espèces supérieures de 100 à 1000 fois le taux naturel avec des populations de vertébrés qui ont chuté de 69% en moins de 50 ans. Aujourd'hui, plus de un million d'espèces animales et végétales sont menacées à court terme. C'est donc une sur 8. Cette perte massive de biodiversité, a des conséquences directes sur notre économie et concernent de nombreux secteurs, l'agriculture avec le déclin des pollinisateurs la pêche avec la surexploitation et le blanchiment des coraux. Et ainsi que le tourisme impacté par les paysages en souffrance sans oublier l'eau. Le sujet est à la fois international mais il est profondément local nos collectivités les élus ont à coeur de protéger leur territoire. La diplomatie environnementale ne peut pas tout régler. Nous devons continuer d'accompagner de collectivités et de protéger ce sur quoi nous avons une emprise réelle par des solutions fondées sur la nature. l'heure notre pays souhaite porter un message d'exemplarité à l'international, la France nation verte doit se prémunir d'avoir le verbe haut et l'action faible donc madame, la Première ministre quels engagements concrets. La France porte-t-elle au niveau international et qu'en est-il de l'objectif 0 perte nette de biodiversité inscrit dans la loi française.-- Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Christophe Béchu Ministre. De la transition écologique et de la cohésion des territoires. Merci madame. La présidente madame. Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur. Chevrollier, j'aimerais vous remercie pour votre question mais pas seulement pour votre présence. Il y a quelques jours au sein du ministère de la transition écologique pourrait représenter le sénat français pour témoigner de votre attachement à ce que cette COP15 soit un succès, quand avec Bérangère Couillard. Nous avons reçu toutes les ONG qui sont mobilisés et je sais que vous serez personnellement un des acteurs de cette. De cette COP15 qui, qui a commencé à Montréal. Il y a quelques heures.-- L'ambition, elle est simple.-- Vous avez donné les chiffres et ils font froid dans le dos.-- Un million d'espèces menacées, 75% de la surface de la planète qui est altérée par la pollution. 85% des zones humides qui ont disparu. Et ce constat-là. Il nécessite une mobilisation qui était à la hauteur. De ces extinctions de ces menaces en opposant pas le climat et la biodiversité parce que les deux sont liés. Quand le climat se dérègle, il accélère la disparition des espèces il diminue ce que la forêt est capable de piéger en terme de carbone et à l'inverse quand on investit sur des solutions qui sont fondées sur la nature, on se donne les moyens de lutter contre le dérèglement climatique. Nous allons à cette COP 15 à la tête d'une coalition de 112 pays. Avec le Costa Rica et l'Angleterre pour définir et pour défendre le 30 30, la préservation de 30% des Terres de 30% des mères à l'horizon 2030, avec des engagements financiers nous sommes l'un des 3 seuls pays pour le moment avoir indiqué que nous étions prêts à nous engager, il y avait une cohérence lié à la fois à l'annonce d'un One Forest Summit dans quelques mois avec les pays africains pour regarder comment préserver le bassin du Congo et ses réserves de biodiversité. Avec le refus exprimé par le président de la République d'exploitation des fonds sous-marins et avec la perspective de la planification écologique, porté par la Première ministre qui nous permettra de relier tout ça et à court terme. Ce sont 150 millions d'euros. Consacré à la biodiversité qui pourront être dégagés dans le cadre du Fonds Vert. Je salue la sénatrice Lavarde dont je sais l'attachement et le suivi attentif par rapport à ce sujet et qui ne permettront d'accompagner, de manière concrète nos territoires les 1756 territoires concernés par Natura 2000 et la centaine de parcs nationaux maritime ou régionaux dont nous disposons mais mais même. Si Monsieur le Ministre, vous avez une poignée de secondes pour répliquer. Oui, merci Monsieur le Ministre, nous soutenons les 30% d'aires protégées mais on veut une effectivité réelle et le Fonds Vert ne suffira pas de non vraiment les moyens d'avoir de notre souveraineté notamment sur nos nos eaux territoriales et notamment d'outre-mer. Merci, cher collègue, la parole est à présent à madame Brigitte Lherbier sénatrice dans le groupe Les Républicains. Madame la présidente, madame le Ministre. Chers collègues. L'UNICEF a rendu dernièrement un rapport très inquiétant sur la protection de l'enfance en France. Elle constate qu'un enfant est tué par ses parents, tous les cinq jours et que les hospitalisations pour violences physiques commises par les parents ont augmenté de 50%, de 2017 à 2020 la police, la gendarmerie les procureurs nous font régulièrement état de cette violence intrafamiliale particulièrement grave pendant le confinement. Le secrétaire d'État Adrien taquet de l'époque était très attentif et inquiet pour l'avenir. Les violences faites aux femmes sont désormais combattu avec véhémence par tous. C'est devenu une priorité nationale et c'est parfait mais qu'en est-il pour la maltraitance envers les enfants. Si la situation de crise que traverse l'aide sociale à l'enfance est très préoccupante nationalement notamment par le nombre important de mineurs étrangers isolés. Elle est aussi dans mon département du Nord qui est le 1er département français en nombre d'enfants placés. 50% des décisions du juge des enfants concerne les produits, les mesures de protection de l'enfance. La presse locale souligne toutes les semaines des situations préoccupantes où les professionnels du secteur, tire la sonnette d'alarme. Actuellement dans le nord 270 ordonnance de placement ne peuvent être honorées, faute de places d'hébergement pour ses enfants en détresse. Il reste exposée aux dangers qui les menacent chez eux. Le rapport de l'UNICEF est un nouveau signal d'alarme. Un véritable plan national de protection de l'enfant hors de son foyer et de veille à domicile, doit être mise en place par le gouvernement pour épauler les départements une stratégie nationale est nécessaire pour assurer une protection renforcée. C'est un devoir de solidarité nationale a porté au département submergé par la précarité des familles, l'afflux des mineurs isolés et surtout par la violence rencontrée dans tous les coins de France. Merci cher collègue. Pour vous répondre madame Charlotte Caubel Secrétaire d'État chargée de l'an. Merci madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, sénatrice, madame la sénatrice Brigitte Lherbier. Oui, le dispositif de protection de l'enfance étant tension. Oui les signaux de sortie de crise sanitaire sont particulièrement rouge rouge vif, tant sur les violences commises sur les enfants que sur la santé mentale de nos enfants que sur le nombre de placements qui en forte augmentation, plus de 10% sur le département du Nord comme dans bien d'autres départements et dans des territoires particulièrement impacté par les conditions socio-économiques en dépit, vous l'avez rappelé, madame la sénatrice de ce qui a été fait dans le précédent quinquennat, et en dépit de l'investissement très fort qui est fait par les départements sur cette politique prioritaire. C'est pourquoi le président de la République et le gouvernement ont décidé de faire de l'enfance et de la protection de l'enfance une priorité du du quinquennat et à l'occasion du dernier comité interministériel qui s'est tenu autour de la Première ministre 40 actions 50 priorités ont été définies, tous les ministères sont engagés et j'en assurer la coordination il m'appartient aussi, madame la sénatrice, de mettre en oeuvre la loi du 7 février 2022, vous en conviendrez adopté relativement récemment et qui impose une forte impulsion le GIP France Enfance protégée permettra une meilleure coordination des acteurs au niveau national les conseils départementaux de protection de l'enfance permettront une action mais le coordonné au niveau territorial. Il faut plus d'État pas que l'État, mais aux côtés des départements, c'est le rôle de ces comités départementaux qui seront installés à partir du 1er janvier dans les départements prioritaires. Le président du nord m'a dit qu'il installerait ce comité départemental reste bien sûr évidemment la question très complexe des hommes et des femmes qui prennent en charge ces enfants. Vous savez que la politique de revalorisation des travailleurs sociaux est une priorité du des des gouvernements, mobilisés, nous sommes tous mobilisés sur la prise en charge des publics les plus vulnérables, pour les protéger. Pour les accompagner pour leur assurer un avenir et renforcer l'égalité des chances, c'est notre priorité. Vous pouvez compter sur mon engagement. Merci madame la ministre, la parole est à présent monsieur Jean Louis Masson pour la. Pour les non inscrits étant aussi grande que 2 fois la Belgique la région Grand-Est ne permet aucune gestion de proximité. De plus elle étouffe l'ancienne région Alsace dont l'identité est très forte. Tous les sondages montrent qu'une écrasante majorité des Alsaciens souhaite sortir du Grand-Est. Malheureusement, les membres de l'exécutif régional s'accrochent à leurs prébendes et prétendent le contraire. Le sujet du Grand-Est sera inévitablement évoquée lors de l'examen du prochain projet de loi de différenciation annoncée pour début 2024. Auparavant, il faut cependant clarifier la situation. Pour couper court aux controverses politiciennes. Un référendum préalable et non a posteriori je dis bien préalables et donc indispensable pour connaître l'avis des alsaciens de manière démocratique et incontestable. Sans vous prononcer sur l'opportunité d'un redécoupage du Grand-Est. Je vous demande donc Madame le Ministre si vous acceptez le principe d'organiser un tel référendum préalable. Merci, cher collègue, la parole est à présent à Madame Dominique Faure Ministre délégué chargé des collectivités territoriales et de la ruralité pour vous répondre.-- Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Masson. La question du statut de l'Alsace au sein de la région Grand-Est depuis la création de cette dernière a fait l'objet de débats locaux et nationaux que nous avons tous entendu. janvier 2021, donnant naissance à la Communauté européenne d'Alsace, cette évolution institutionnelle qui a été accompagné par le gouvernement et le législateur apporter une réponse consensuelle aux demandes des citoyens et des élus alsaciens. Elle a permis d'adapter l'organisation des collectivités alsaciennes aux besoins spécifiques de leur territoire et de doter la CEA Communauté européenne d'Alsace de compétences supplémentaires justifié là aussi par les enjeux particuliers qu'elle cette collectivité fait face. Notamment en matière de coopération transfrontalière cette organisation différencier existent donc déjà et je crois qu'il est important que nous lui donnions le temps de produire ses effets sur le plan juridique notons ensemble. Que le législateur a prévu que la modification des limites territoriales d'une région ne peut intervenir que par le biais de la loi, soit à l'initiative du gouvernement après consultation du conseil régional et des conseils départementaux concernés soit à la demande du conseil régional et des 10 conseils départementaux intéressé je crois Monsieur le Sénateur, que le gouvernement a déjà largement démontré sa volonté de permettre aux collectivités territoriales d'adapter leur organisation. Il a ainsi notamment voulu faciliter aussi dans le cadre de la loi 3DS, la création de collectivité territoriale unique regroupant la région et ses conseils départementaux ce principe d'adaptation nous est essentiel parce qu'il permet aux collectivités de mieux répondre aux enjeux auxquels elles font face. Alors je crois donc que nous devons d'abord pleinement investir les possibilités que nous offrent déjà la loi je vous remercie. Je suis quand même un peu surpris que vous puissiez dire que tous les Alsaciens sont contents parce que dans ces conditions, pourquoi vous voulez pas faire un référendum. Votre réponse c'est n'importe quoi. Madame le Ministre tout le monde est mécontent en Alsace. Tout le monde est mécontent également dans les autres départements parce que nous sommes victimes d'une région tentaculaire. Alors c'est comme vous le dites Madame le Ministre tout le monde est content en Alsace. Pourquoi vous ne prenez aucun risque à ce moment-là d'organiser une. Un référendum, pourquoi est ce que vous avez peur d'organiser un référendum pour demander l'avis des gens parce que c'est pas votre point de vue de dire que tout va bien, c'est un mensonge de dire que tout va bien si les à chaque référendum à chaque consultation par biais de sondage, on constate que les les Alsaciens sont sont mécontents et qu'il y a également en Lorraine et en Champagne-Ardenne, une majorité de gens qui veulent remettre en cause la taille de la région Grand-Est, alors Madame le Ministre je vous dis une chose, le gouvernement fait ce qu'il veut mais il faut quand même arrêter de mentir.-- Chers collègues. Je vous rappelle que les prochaines questions d'actualité au gouvernement auront lieu mercredi 14 décembre prochain 15h je vais suspendre la séance elle sera reprise à 16h 30 pour l'examen de la proposition de loi visant à protéger les collectivités territoriales de la hausse des prix de l'énergie, la séance est suspendue.

Chers collègues, la séance est reprise, je donne tout d'abord la parole à Monsieur Bernard Delcros pour une mise au point, au sujet d'un vote. Oui merci madame la présidente. Il s'agit des des scrutins, 81, 82 et 84 sur lequel je souhaite voter contre et j'ai été inscrit comme ayant voté pour.-- Très bien. Acte donné de votre mise au point le figurera dans l'analyse politique du scrutin des scrutins concernés ont chers collègues. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte. Sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2023 n'est pas parvenu à l'adoption d'un texte commun. J'informe également le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 ont été publiés ces candidater seront ratifiées si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévue par notre règlement.-- L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi visant à protéger les collectivités territoriales de la hausse des. Prix de l'énergie en leur permettant de bénéficier des tarifs réglementés de vente de l'énergie présenté par monsieur Fabien Gay, mesdames Céline Brulin, Cécile Cukierman et plusieurs de leurs collègues. Il s'agit donc d'une demande du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste dans la discussion générale. La parole est à monsieur Fabien Gay, auteur de la proposition de loi pour 10 minutes, chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre. Monsieur le rapporteur, madame la présidente de la commission. Mes chers collègues. Alors il y a le texte nous allons-y venir.-- Demandant le retour aux tarifs réglementés du gaz et l'électricité pour toutes les collectivités. Et puis il y a le contexte. Permettez-moi de dire un mot d'abord sur le contexte lorsqu'on est un groupe.-- Minoritaires et d'opposition. Nous avons une niche ou de pas en. Et donc il faut évidemment bien choisir son texte. Et dont nous avons 2 solutions, soit parce que nous avons un projet politique à l'opposé de celui de la majorité sénatoriale et donc nous choisissons un texte pour combattre politiquement et marquer des points et nous l'avons déjà fait ici dans cet hémicycle. La renationalisation des concessions autoroutières. On a déjà débattu sur la question de.-- de.-- Interdire toute coupure d'énergie tout au long de l'année on a déjà eu un certain nombre de débats sur le pôle public du médicament. Parfois il nous arrive aussi de marquer des points et que une position minoritaire devienne majoritaire. Je dois noter que la constitutionnalisation de l'IVG continue à faire son chemin et elle était adoptée à l'Assemblée nationale. Et puis la création d'une délégation aux droits des enfants ici au Sénat reviendra demain et nous nous en félicitons et nous espérons qu'elle fera adopter Nous a rejoint, à trouver une position qui rassemble, parce que l'idée a fait son chemin dans la société où dans notre hémicycle. On doit saluer par exemple la question de la rouvert l'utilisation des retraites agricoles portés par mon ami André Chassaigne. Je veux aussi saluer lorsque les APL avaient été rabotée de cinq euros par le Julien d'Normandie. Nous avions réussi ici au Sénat, s'était porté par ma collègue Cécile Cukierman à nous mettre d'accord ou même.-- Pour que nous puissions avoir droit au chapitre sur le sept et. Je dois vous le dire.-- Cette proposition de loi sur le retour des tarifs réglementés du gaz et l'électricité pour toutes les collectivités, nous pensions qu'elle était dans la 2ème catégorie pourquoi.-- Parce que la situation est extrêmement grave pour nos collectivités.-- Bien sûr, on connaît tous pourquoi nous en sommes là. La guerre en Ukraine. Évidemment l'arrêt d'une partie de nos centrales nucléaires nous en avons parlé aux questions d'actualité faisant que nous étions exportateur Net jusqu'à présent et nous sommes devenus importateur Net cette année évidemment la dérégulation. Du marché d'ailleurs. Je pense que nous aurons là aussi.-- À débattre entre nous sur le marché européen de l'électricité. Je vois que là aussi, même les ministres. Bush puisque. Après nous avoir ri, on est. Pendant des années et des années, lorsque nous disions, que ça ne fonctionnait pas. On nous disait que c'était très bon. Et aujourd'hui même, le ministre de l'Économie et des Finances dit qu'il faut le délier le prix du gaz et l'électricité. Tant mieux. Et d'ailleurs il faudra un jour nous expliquer comment un marché sans stock.-- C'est-à-dire peut s'organiser parce que le marché libre. C'est de la production qui rencontre une demande mais là aujourd'hui l'électricité il y a pas de stock et donc, c'est purement de la spéculation et c'est ce que nous vivons et ce que vivent évidemment nos collectivités. Et elles sont toutes, toutes. Face à ce problème. Quel que soit leur couleur politique, leur choix budgétaires ou leur taille. Et comme ici, il n'y a que des sénateurs et les sénatrices de terrain. Vous avez les mêmes discussions que l'ensemble des sénatrices et sénateurs communistes dans mon département en Seine-Saint-Denis. Lorsqu'on discute avec le maire de Noisy, c'est plus 800.000 euros. Le maire de Neuilly-sur-Marne, plus d'un million d'euros. Le président du département 30 millions d'euros. Vous voyez j'ai pris tout l'arc républicain de la Seine-Saint-Denis et dans chaque département. C'est exactement. La même chose, alors évidemment nos collectivités sont inventives sauf que elles sont face à des problématiques extrêmement forte et l'inflation ne touche pas que l'énergie, les matières premières le ça laisse ceux qui gèrent des collectivités, des cantines scolaires voit bien les difficultés à boucler les Budgets et il faut le dire. Les prix de l'électricité ne redescendront pas ceux du gaz non plus et la crise et durable. Alors elles sont face à un dilemme. Soit elles augmentent les impôts mais nous en conviendrons toutes et tous, c'est impossible. 60 d'été.-- Pour faire du fonctionnement ingérable ou alors fermer des services publics. C'est évidemment impensable.-- Alors on demande nos mères de bricoler. Baisser le chauffage dans les écoles ou les EPHAD. Je vous laisse le faire. Ne pas chauffer les piscines en plein hiver. Je connais personne qui a envie de se baigner dans une piscine à 12 degrés ou demander aux usagers des bibliothèques de mettre leurs manteaux pour aller consulter un livre sous peine de ressortir comme un pingouin, évidemment ce n'est pas sérieux. Alors quand il y a une crise, il faut innover. Vous l'avez fait madame la Ministre, avec des dispositifs. Alors si quelqu'un dans cette salle est capable d'expliquer à quelqu'un, le dispositif. Qui a été déjà bricolé 3 fois en un mois et demi. Donc il y a trois critères. Personne ne remplit les 3 critères mais souvent de bref. Demandez à vos préfet de vous expliquer, je vous assure vous passerez un bon moment de rire. Sauf que nos collectivités elles elles doivent gérer alors. Parfois il faut inventer. Oui c'est vrai mais parfois quand on ne peut pas mettre des rustines sur une jambe de bois. Ben il faut se tourner vers passé pas par dogmatisme. Pas parce que on se dit que on est attachés philosophiquement, même nous, vous le savez alors ou nationalisation d'EdF-GDF ce Marcel Paul minus communiste qui a nationalisé inventé les tarifs réglementés avec la promesse que tout le monde aurait accès à l'énergie, ou qu'il soit à un prix raisonnable. Mais parce que pour l'instant les tarifs réglementés sont les plus efficaces, les plus efficaces que nous connaissions. Et nous sommes surpris donc aujourd'hui que la majorité ne veulent pas y revenir, je vous le dis. Pour finir sur la fin des tarifs réglementés du gaz pour tout le monde. Madame la ministre. Vous nous trouverez sur votre chemin.-- C'est le 30 juin prochain Nous mettons à bas les tarifs réglementés du gaz pour tous les usagers, ça va être infernal pour 5 millions de foyers et donc j'espère qu'au moins sur cette question, nous arrivons à nous rassembler. Alors j'en viens évidemment sur. les. Événements sur ce que monsieur le rapporteur, et je veux le remercier ici. Pour la discussion franche, que nous ayons eu à partir des 4 arguments qu'il a développé d'abord les TRV, ça serait très cher, 50 milliards, on nous a dit puis après une étude du Sénat indépendant par montrer que c'était 3 milliards a dit. 3 milliards et demi pour le retrouve le retour des tarifs réglementés du gaz et l'électricité pour toutes les collectivités. Pour l'instant. Chers collègues. Le bouclier tarifaire, le filet de sécurité. La reine supplémentaires l'indemnisation aux acteurs alternatifs. Ces 43 milliards d'euros en une année, 43 milliards donnés aux acteurs alternatifs, contre 3 milliards et demi si nous votons cette PPL franchement c'est le choix entre le privé et le public, c'est le choix entre le racket organisé la gabegie et le choix de l'efficacité. Le 2ème argument c'est que si toutes les collectivités devaient casser leur contrat ils auraient des contentieux mais nous n'avons jamais dit ça. C'est elle qui aurait marché, elles ont qu'à y rester mais nous ouvrons la possibilité à celles qui se retrouvent face à des factures de 30% en moyenne, voire 300% de pouvoir avoir accès au tarif réglementé et on ne demande à personne de casser son contrat. Le troisième c'est que nous serions contraints par le droit européen. Permettez-moi de vous dire qu'il existe des dérogations. Et nous avons déjà des dérogations dans l'énergie puisque les tarifs réglementés pour les collectivités de moins de 10 ETP. Au moins 2 millions le chiffre d'affaires sont déjà en place. Donc c'est possible et puis je vous rappellerai pas que le Portugal et l'Espagne ont obtenu elle aussi une dérogation parce que c'est écrit des entraves à la réalisation des marchés concurrentiels sont possibles, quand elles répondent à un objectif d'intérêt économique général et quand elles garantissent la cohésion territoriale ou quand elles permettent le maintien d'un prix raisonnable. Nous pensons que nous sommes dans cette situation. Enfin, dernier argument.-- On m'a opposé, on m'a dit oui mais on a fait plein de choses pendant le vote du budget. Ici il n'y a ni son ni naïfs. Nous savons que le texte du budget que nous avons voté hier va repartir à l'Assemblée nationale et que la première ministre va redéclencher 1/8ème 49.3 il en restera rien de ce que nous avons adopté alors. Je vous propose que nous passions vote. Et que si il en reste quelque chose tant mieux, mais s'il n'a restauré. Il y aura toujours cette possibilité et comme l'anus du groupe parlementaire communiste à l'Assemblée nationale et au mois de mai on aura tant de faire le point. Enfin, permettez-moi de dire justement. En conclusion, madame la présidente. J'espère que vous aurez été convaincu par mes arguments mais si tel n'était pas le cas. Permettez-moi de citer quelques.-- Il faudra sans doute aller plus loin. Le groupe LR vous prie de revenir sur la suppression des tarifs réglementés. Un véritable bouclier ne doit pas consister en le déversement d'argent public pour les ménages ou dans l'économie. Il y a des décisions à prendre. Or je n'ai pas entendu une seule intervention sur les tarifs réglementés, alors que c'est fondamental. Ces paroles très sage. Ne sont ni de Jaurès.-- Ni moi-même. Elles sont celles du brillant président Retailleau. Le 12 octobre dernier, donc si vous n'êtes pas convaincu la majorité sénatoriale, par tous les arguments du groupe communiste que nous venons de donner au moins respecter la parole du président Roh Tae Young. Je vous en remercie. Merci. Cher collègue. La parole. État présent à monsieur Laurent Somon, rapporteur de la commission des affaires économiques pour 10 minutes, chers collègues. Madame la présidente, madame la présidente de la commission.-- Madame la Ministre. Mes chers collègues. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui a le mérite. D'aborder 2 sujets de très grande importance. La hausse des prix de l'électricité et du gaz et la protection des collectivités territoriales, avec l'objectif louable d'une plus grande régulation. Des marchés de l'électricité et du gaz. Si notre commission partage le diagnostic établi. Elle ne peut souscrire aux solutions proposées.-- En effet, ces solutions sont comme tu l'as dit contraire au droit de l'Union européenne.-- Mais oublié de dire coûteuse pour le le groupe EDF et porteuse d'effets de bord pour les acteurs locaux dont les collectivités territoriales. C'est la raison pour laquelle notre commission a très largement rejeté la proposition de loi lors de sa réunion du 30 novembre dernier.-- L'objectif de la proposition de loi est louable puisqu'il vise à élargir les tarifs réglementés de vente de l'électricité TRV E et prorogé. Les tarifs réglementés du ventre de gaz le TRV G. Depuis la loi énergie-climat de 2019 les TRV sont limités aux collectivités dont la puissance souscrite est inférieur à 36 kilos VA. Le nombre de personnes, a dit qu'est équivalent temps plein et les recettes annuelles à 2 millions d'euros, comme ça vient de nous être rappelé. De plus, en application de cette loi les TRV G ont été supprimés pour les clients professionnels consommant moins de 30.000 kW/h par an, le 1er décembre 2020 et le seront pour les clients résidentiels et les propriétaires ou copropriétaires d'immeubles dont la consommation est inférieure à ce même seuil le 1er juillet 2023. Les évolutions proposées sont effectivement problématique à plusieurs titres. Tout d'abord elle ne tiennent pas compte des dispositifs de soutien tarifaire budgétaires et fiscaux. Que nous venons d'adopter dans le cadre des lois de finances initiale et rectificative pour 2022 et 2023. Je rappelle rapidement que sont prévues pour les collectivités à blocage des TRV G à leur niveau d'octobre 2021, majoré de 15%. Du 1er janvier au 30 juin 2023. Une compensation des TRV eux à leur niveau de décembre 2022 majoré de 15% du 1er février au 31 de décembre 2023. Un amortisseur d'électricité pour les collectivités non éligible au TRV Un filet de sécurité selon les recettes et les coûts des collectivités et une baisse de taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité le tennis faire FE au minimum européen. De plus, un prix de référence du gaz a été adoptée pour servir de base en lieu et place des terres VG dès juillet prochain à l'application des nouveaux dispositifs de soutien. Le coût de ces mesures comme il vient d'être le rappeler a été évalué à 45 milliards d'euros au total et 20 milliards d'euros Net. Il s'agite. Il s'ajoute au relèvement du plafond de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. La reine de 100 à 120 TWh, qui a représenté un coût de 10 milliards.-- Pour Pour le groupe EDF ne l'oublions pas. Plus encore les évolutions proposées ne respecte pas le droit de l'Union européenne ce qui exposerait bien sûr les collectivités un risque juridique et financier. En effet, la directive du 5 juillet 2019 réserve les TRV eux aux clients résidentiels et micro- entreprises auxquelles sont assimilées, les collectivités ne dépensant ne dépassant pas 10 personnes et 2 milliards de millions d'euros de recettes. Elle prévoit aussi une méthode non discriminatoire et notification dans un délai d'un mois.-- De son côté la directive du 13 juillet 2019 requiert la poursuite d'un intérêt économique générale, ainsi que des critères de proportionnalité de temporalité et de non-discrimination. Dans un arrêt du 6 novembre 2019, le Conseil d'État a rappelé la nécessité de restreindre les TRV eux aux consommateurs domestiques et petits professionnels et de respecter ce qui est très important, une méthode d'empilement des coups. Dans un arrêt du 19 juillet 2017, il a considéré que les Terres VG ne remplissent pas un objectif d'intérêt général. Ni la garantie de prix car pour l'été. Hervé G ils doivent couvrir les coûts des fournisseurs ne respecte non plus la cohérence territoriale car le gaz est substituables son prix et peu harmonisés et sa desserte peu étendue. Ni enfin la sécurité d'approvisionnement qui n'entrent pas dans l'émission des fournisseurs.-- Ce cadre européen a été modifiée par le règlement tout récent du 6 octobre 2022 qui autorise à appliquer les TRV aux PME qui ne dépasse pas 250 personnes et ont des recettes entre 46 et 50 millions d'euros. Une indemnisation des fournisseurs et un examen des mesures sont toutefois nécessaires.-- S'agissant des TRV VG seule est autorisée, l'institution d'une contribution de solidarité non des tarifs réglementés. La proposition de loi et donc directement contraires à ce cadre européen.-- Hervé eux, elle ne respecte aucun critère d'éligibilité ne prévoit ni indemnisation ni notification. De plus elle supprimerait la reine qui, si elle doit à terme être réformé garantit la conformité du marché national de l'électricité avec le cadre juridique européen. Pour les terres VG aucune base législatives ou jurisprudentielles ne les autorise d'autant qu'il ne serait pas seulement maintenu mais aussi élargi.-- Autre point les évolutions proposées ne répondent pas forcément aux besoins des collectivités. Tout d'abord les TRV les terres ne protège en tant que telle. Les collectivités des hausses de prix car leur niveau doit couvrir l'ensemble des coûts des fournisseurs cette fameuse mode de calcul par empilement. Ce sont donc plutôt les dispositifs tarifaires budgétaires et fiscaux liés à ces tarifs qui viennent d'être adopté par le Sénat qui assure cette fonction protectrice. En outre, un grand nombre de de collectivités ayant souscrit des offres de marché souvent via des groupements d'achats de leurs syndicats d'énergie une résiliation anticipée de ces offres les obligeraient à indemniser leurs fournisseurs. Ce qui les fragiliseraient contractuellement et les pénaliserait financièrement. Plus largement. Appliquées aux collectivités des tarifs réglementaires contraires au cadre européen les exposerai de fait à un risque de contentieux et de remboursement. Ne reproduisons pas les erreurs du passé.-- On se souvient tous ici plus certain que d'autres des contentieux sur la contribution au service public de l'électricité le CSPE. Ou sur le relèvement du plafond de la reine. Au reste, la vingtaine d'organismes sollicités collectivités comprise l'ont bien rappelé. Enfin les évolutions proposées sont de nature à déstabiliser les fournisseurs d'énergie. Pour l'électricité. Le groupe EDF seraient contraints d'acquérir des volumes non anticipés dans des proportions importantes dans des délais serrés sur les marchés de gros de l'électricité ou auprès des concurrents. Compte tenu des prix de l'électricité cela exposerait de fait la société un risque financier très élevé. Pour le gaz, le groupe Engie devrait se réorganiser à six mois de l'extinction des TRV G 7 tarifs ayant cessé pour les nouveaux contrats en 2019 et les clients professionnels en 2020. Pour notre commission le coup d'une application des TRV eux été AVG aux communes seraient a minima, comme ça a été dit de à 2 5 milliards d'euros pour 2023. Dans les 2 cas les fournisseurs alternatifs serait évincé au profit de ce historique au mépris du principe constitutionnel de libre concurrence.-- Au total. Si notre commission reconnaît la nécessité. À une évolution des TRV et des TRV VG. Elle ne pourrait être réalisé que dans le strict respect du cadre constitutionnel et du droit européen. Dans le cas contraire, ce serait exposées les collectivités un grave risque juridique et financier, ce qui ne serait pas responsable. Pour autant. Je me félicite que l'examen de cette proposition de loi avec son promoteur ou ses promoteurs. Soit aussi l'occasion de mettre le gouvernement face à sa propre responsabilité.-- Car le gouvernement a agi de manière tardive et timorée face à une crise énergétique dont les fondements ont été connus et rappelé. L'an dernier encore on nous disait que la hausse des prix était passagère que le risque de délestage hypothétique. Je rappelle qu'il a fallu attendent le conseil des ministres du 29 novembre dernier pour que le gouvernement présente un plan sur la préparation risque d'approvisionnement électrique hivernaux. notre commission s'est inquiété de la flambée des prix des énergies et du décalage du programme d'arrêt de tranche dès son rapport de la crise Covid 19 de juin 2020. Nous avons été aussi les premiers à nous pencher sur les conséquences de la guerre russe en Ukraine et du phénomène de corrosion sous contrainte dans notre rapport sur le risque de Black-out de février 2022. Nous avons enfin appelé à garantir notre sécurité d'approvisionnement dans notre plan de notre rapport sur la relance du nucléaire de juillet 2022. Plus concrètement, c'est la Cena qui encadrer les coupures d'électricité et les offres de gaz faciliter les projets de biogaz. Évaluer la situation des collectivités dès la loi pouvoir d'achat d'août dernier. On ne peut pas dire que le gouvernement n'a pas été prévenu. Il aurait dû et pu réagir plus précocement et plus fortement. Notre commission attendons du gouvernement une évolution du cadre européen au-delà de celui national et bien sûr du marché de gros. Outre celui du détail. Rappelons que la France, comme ça a été dit, n'a toujours pas obtenu un découplage du prix de l'électricité, celui du gaz. Contrairement au Portugal et à l'Espagne. Il y a encore beaucoup à faire. Dans ce contexte ne contre notre commission continuera d'être attentive à la régulation des marchés du gaz et d'électricité à la protection des consommateurs et en particulier des collectivités locales dont nous aurons forcément un replay reparler dans les prochains projets de loi à la fois sur l'électricité nucléaire et à la fois dans le cadre du de la programmation pluriannuelle de l'énergie.-- Merci monsieur le rapporteur. La parole est à présent à à Madame Dominique Faure Ministre délégué chargé des collectivités territoriales et de la ruralité.-- Merci madame la présidente. Monsieur le rapporteur, madame la présidente de la commission mesdames et messieurs les sénateurs. La proposition de loi que vous nous présentez aujourd'hui suggère la mise en oeuvre de 3 dispositions. La première, la modification des règles de calcul des tarifs réglementés de vente de l'électricité. Hervé eux pour qu'ils soient calculés en fonction du coût de production du mix électrique français. La seconde, l'extension des TRV à toutes les collectivités et leurs groupements et la troisième le rétablissement des tarifs réglementés du gaz au bénéfice des collectivités locales et des particuliers. Alors vous le savez, le gouvernement est pleinement engagée en soutien des collectivités territoriales et des Français face à la crise énergétique. Il a déployé plusieurs outils, en ce sens au cours des derniers mois, les plus petites collectivités sont assimilés à des particuliers le bénéficiant cela du bouclier tarifaire de l'électricité. Les critères à respecter sont les suivants, moins de 10 moins de 2 millions d'euros de recettes et une puissance souscrite inférieure à 36 KV à. Toutes les autres collectivités bénéficieront à partir de janvier 2023 de l'amortisseur électricité mis en place par le PLF 2023 qui viendra limiter la hausse des prix de l'électricité. Le bouclier tarifaire sur l'électricité et l'amortisseur s'applique, quel que soit le contrat de fourniture d'électricité qu'elles ont souscrits, les collectivités ont donc nul besoin de sortir d'un gros contrat groupés pour être protégée, elle bénéficie à ce titre d'une aide de l'État équivalente à celle dont bénéficient les clients à titre individuel au tarif réglementé ou en offre de marché. Je rappelle que les collectivités les plus fragiles peuvent également bénéficier du filet de sécurité budgétaire mis en place en 2022. Les discussions parlementaires sur le projet de loi de finances pour 2023 ont conduit à étendre ce filet de sécurité aux départements et aux régions. À eux de l'amortisseur électricité le filet de sécurité représente 2, 5 milliards de soutien de l'État aux collectivités, nous avons entendu les préoccupations dont les parlementaires se sont fait l'écho pour la mise en oeuvre de ces dispositifs et, comme l'a annoncé la Première ministre une simplification du filet de sécurité sera proposée dans la version finale du projet de loi de finances pour 2023. Tout cela s'ajoute aux mesures générales dont bénéficie l'ensemble des collectivités depuis 2022. Je pense en particulier à la baisse de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité la TIC F. E. A. sont minimal légal soit un coût de 8 milliards pour l'État et cette mesure est prolongée en 2023. Aux côtés de ces mesures visant à modérer les dépenses d'énergies. Le gouvernement a également proposé des hausses de recettes ainsi la dotation globale de fonctionnement sera augmenté de 320 millions d'euros en 2023 pour la première fois depuis 3 ans, 200 millions d'euros seront fléchés sur les communes rurales. Par ailleurs, les bases de la fiscalité locale seront indexés sur l'inflation. Ce qui générera des ressources supplémentaires dans le respect de l'autonomie financière des collectivités. Par ailleurs, le gouvernement ne peut souscrire à vos propositions qui seraient non opérationnels car contraire au droit européen, comme monsieur le rapporteur. La extrêmement bien expliqué. S'agissant de l'électricité. Monsieur le sénateur, le droit européen. L'article 5 de la directive de 2019, la directive 944 réserve en effet strictement les TRV sur l'électricité aux consommateurs résidentiels et aux professionnels de taille TPE. D'où les moins de 10 salariés les moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, comme cela a été rappelé par monsieur le rapporteur. Tout à l'heure, cela permet aux petites collectivités, comme vous l'avez dit vous-même monsieur le sénateur. Cela permet aux petites. Collectivités d'être éligible au TRV eux l'application du TRV un périmètre plus large. N'est juste pas possible en vertu du droit européen. S'agissant de l'électricité, toujours la même directive encadre strictement les conditions dans lesquelles les tarifs sont établis. Le droit européen prévoit en effet que les tarifs doivent être établies selon des modalités qui garantissent l'égalité de traitement entre tous les fournisseurs et dans un cadre concurrentiel m'exprimer. J'entends pas ce que vous dites mais on pourra en parler tout à fait. Après un prix calculé sur la base des coûts du mix français ne permet pas une concurrence effective en ce qu'aucun de fournisseurs français. Si ce n'est. EDF ne serait capable de proposer une offre à ce prix. J'entends en revanche et le gouvernement également qu'il est nécessaire de travailler à une réforme structurelle du marché de l'électricité en Europe, sujet sur lequel le président de la République s'est déjà exprimé très clairement s'agissant du gaz les tarifs réglementés de vente du gaz TRV j'ont été jugés non conformes au droit européen par le Conseil d'État en juillet 2017. C'est pour cette raison qu'ils disparaîtront au 1er juillet prochain Et a fortiori les étendre seraient donc strictement contraire à cette décision de justice et aux droits européens. Pour autant. La fin d'été. V. j'ai ne constitue pas un obstacle à la mise en place de mesures de soutien et d'accompagnement ciblé comme le filet de sécurité et qui lui concerne toutes les énergies. Alors vous l'avez compris, même si l'objectif poursuivi est louable, monsieur le sénateur. Comme l'a dit monsieur le rapporteur. Toutes ces raisons et surtout la non-conformité au droit européen, amène le gouvernement à être défavorables à cette proposition de loi, tout en rappelant qu'il active activera tous les leviers nécessaires pour protéger efficacement nos concitoyens ainsi que toutes les collectivités, contre la hausse des coûts de l'énergie. Je vous remercie.-- Merci, madame la Ministre, dans la suite de la discussion générale. La parole est à madame Guilaine Pantel du groupe RDSE. Et vous avez 4 minutes, chers collègues. Madame la présidente. Madame la ministre, monsieur le rapporteur, madame la présidente de la commission économique chers collègues. Dans un 1er temps, nous souhaitons remercier nos collègues sénatrices et sénateurs du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste pour avoir impulsé ce débat de la protection des collectivités territoriales face à la hausse du prix de l'énergie.-- Ces derniers temps il ne se passe pas une semaine sans que je sois interpellé par des élus locaux l'rien à l'image du maire de Moissac française qui constate une augmentation de la facture de 46% sur l'éclairage public et de 55% sur des bâtiments publics et je me doute que vous êtes toutes et tous dans le même cas, quel que soit votre département. En effet, pour bon nombres de collectivités et notamment celles qui anticipent le plus le cycle budgétaire annuelle pour le prochain exercice est déjà entamée, nous connaissons le mécanisme avec la tenue d'une série de réunions de préparation et d'arbitrage durant lesquelles on fait des heureux, mais où l'on éprouve aussi beaucoup de frustration face à une épargne nette souvent trop maigre pour la réalisation des lotissements patiemment. Aujourd'hui, et notamment à l'occasion du congrès des maires et présidents d'intercommunalité nous recueillir les témoignages de plusieurs personnes à la tête d'exécutifs locaux qui nous expriment leur grande prudence dans ce contexte.-- Depuis la fin de l'année 2021 et encore plus depuis le début de la guerre en Ukraine, les collectivités territoriales subissent de plein fouet l'impact de l'inflation, en particulier sur les dépenses énergétiques. Par conséquent pour éviter un bis répétita hein se faisant surprendre par des événements difficilement prévisibles. Les ambitions des collectivités sont redimensionné à la baisse. Ceci entre autres dans l'optique de limiter l'adoption de décision modificative ouvrant des crédits nouveaux.-- L'autre risque majeur que l'on voit poindre, pardon c'est la disparition ou a minima, la dégradation de certains services publics locaux délivrés par les communes les épaisses les EPCI, les départements et les régions. Or, dans la mesure où le service public, c'est le Patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Nous pouvons craindre le fait que nos concitoyens les plus fragiles en paient les conséquences. Et c'est le cas de dire si le choix est fait de confier à des entreprises privées toutes au parti d'une activité qui jusqu'alors était assuré directement par l'administration et de même. D'un souvent un nouveau coup pour les usagers.-- Et si Madame la Ministre. Que diraient les habitants de votre ville de coeur de Saint-Orens de gamme ville si la municipalité que. Contrainte de réduire la programmation de l'espace culturel. Ou de raboter le financement de l'Epad Augustin la bouille. Il s'agit naturellement d'une question rhétorique, puisque nous sommes d'accord pour reconnaître le caractère essentiel de ces structures pour l'épanouissement de chacun de la petite en face au grand âge.-- La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui a le mérite de mettre en évidence ces difficultés. Mais elle permet également d'exiger la sortie des collectivités d'un système de réglementation tarifaire qui est une véritable.-- Que cela soit sur les tarifs réglementés de vente d'électricité ou sur les tarifs réglementés de 22 grâce, l'État doit pouvoir reprendre le contrôle sur un marché qui expose les demandeurs à des risques tout bonnement déraisonnable.-- Néanmoins, tout comme monsieur le rapporteur. Le groupe RDSE a pleinement conscience de la primauté du droit européen sur le pardon du droit européen sur le droit national d'ce. C'est la raison pour laquelle nous partageons pleinement l'intention de travailler sur une proposition de résolution européenne évoqué en commission par notre collègue Franck Montaugé. En conclusion, le groupe RDSE est pleinement mobilisée pour avancer sur ces sujets et votera en partie pour cette proposition de loi, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à présent à monsieur Patrick Chaize du groupe les républicains pour cinq minutes. Madame la présidente, madame la présidente de la commission des affaires économiques. Monsieur le rapporteur. Madame la Ministre, mes chers collègues.-- Chacun de nous le constate avec une vive préoccupation. Les collectivités sont confrontées à une hausse sans précédent des coûts de l'énergie.-- Pas une semaine sans qu'un maire ne nous alerte ici sur une piscine qui n'est plus possible de chauffer là sur une salle des fêtes dans l'alimentation en électricité pèsera lourdement sur le budget communal. Les qui nous remontent sont alarmants. Le prix de l'électricité sur le marché du gros est passé de 49 euros le mégawattheure en 2021. À plus de 1000 euros fin août 2022, soit une multiplication par 20. Les prix du gaz ont quant à eux évoluer d'un niveau particulièrement faible en 2029 euros. En moyenne à des pics de 114 euros fin 2021 et jusqu'à 300 euros en août 2022.-- Les associations d'élus sont elles aussi grandement préoccupés. L'Association des Petites Villes de France note que les dépenses énergétiques de certaines communes ont bondi de 50%. Pour l'AMF et la Fnccr. Ces hausses varieraient entre 30 et 300%. Ce que rappelait récemment le président Larché doit nous interpeller. Les communes françaises ont consommé au 31 juillet la totalité de leur budget énergie prévue en 2022 et non pas de visibilité pour 2023.-- Face à cette situation alarmante. Le groupe communiste nous propose une solution nationale consistant à élargir le bénéfice des tarifs réglementés de vente d'électricité à toutes les collectivités et à maintenir au-delà du 30 juin 2023. Les tarifs réglementés de vente de gaz.-- Mes collègues l'ont rappelé. Nous partageons la préoccupation du groupe communiste. Nous partageons l'urgence à agir pour soutenir les collectivités. Nous partageons les propos du président Retailleau. Sans aucun doute. Mais nous souhaitons sur ces sujets, trouver des solutions efficaces solide juridiquement et protectrice pour les finances de nos communes. Or les dispositifs proposés. Font courir de nombreux risques que notre rapporteur Laurent Somon a énuméré. Gardons-nous des fausses bonnes idées qui exposerait nos collectivités à des contentieux juridiques nombreux et un risque de pénalités financières. Pousser les collectivités a opté pour l'été. Hervé eux c'est les condamner pour la moitié d'entre elles a résilié prématurément un contrat ce qui a un coût. C'est également leur promettre l'assurance d'une électricité moins cher. Ce qui n'est pas démontrée.-- Maintenir les tarifs réglementés de vente de gaz c'est favoriser une Fonda sincérité juridique alors que l'ensemble des communes et des particuliers a été avertie que ceux-ci s'étendrait au 30 juin prochain. Veillons enfin à ne pas pénaliser les fournisseurs d'électricité et de gaz qui serait contraint avec les dispositions de la PPL à se procurer en urgence des volumes conséquence d'énergies carbonées pour le gaz et souvent indisponibles pour l'électricité.-- Comme notre rapporteur l'a mentionné le Sénat et puis perdu la commission des affaires économiques n'ont pas été inactifs sur le sujet des coûts de l'énergie depuis plus d'un an. Nous l'avons encore démontré ces dernières semaines lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2023, en améliorant considérablement le filet de sécurité, énergie. Nous pouvons encore aller plus loin en soutenant la renaissance de notre parc nucléaire et on en envoyant un message très clair auprès de l'Union européenne pour une refonte des marchés de l'électricité. Nous accueillons le texte proposé par Monsieur et ses collègues comme un appel à agir et nous nous y associons bien volontiers. Mais compte tenu des trop nombreuses fragilités juridiques que je viens d'évoquer le groupe Les Républicains ne pourra pas voter cette PPL en l'état, je vous remercie. Merci. Je demande maintenant à Jean-Pierre Grand. Prendre la parole au nom du groupe les indépendants pour quatre minutes, chers collègues.

le titre de cette PPL et et d'actualité. Nous sommes sollicités de manière constante sur le sujet depuis le début de la guerre en Ukraine et ses conséquences énergétiques comme les ménages, les entreprises nos collectivités. Ça a été dit j'irai pas plus loin, souffrent de la hausse des prix de l'énergie et ce après après la crise du Covid, qui les a déjà beaucoup fragilisé. Nous entendons souvent les questions de chauffage dans nos écoles, collèges, lycées, nous aussi, les fermetures d'équipements et services dans nos communes. Les craintes des élus locaux. Je pense en particulier aux maires sur la santé financière des collectivités ne peuvent pas être prise à la légère. Si l'idée de cette PPL est intéressante. Je suis surpris par sa méthode comme l'a souligné dans son analyse précieuses le rapporteur. Les articles de cette PPL sont contraires à notre droit national et au droit européen en plus ils sont en opposition totale avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et celle du Conseil d'État. En commission des affaires économiques. Vous avez expliqué qu'il s'agissait en quelque sorte d'une PPL d'appel.-- Pourquoi pas. Nous participons au débat que vous proposez. Mais permettez-moi de dire qu'il y avait d'autres véhicules qu'PPL pour débattre du sujet. La crise énergétique de place face à nos choix antérieur et à nos faiblesses stratégiques, nous avons voté récemment dans cet hémicycle à une grande majorité le projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables nous serons mobilisés sur celui qui arrive. Concernant le nucléaire. Les temps forts énergétique ne sont pas terminés en 2023, nous devrons démontrer leur efficacité a décidé un avenir énergétique souverain. Quand il s'agit des tarifs de l'énergie et je pense que l'échelon européen est incontournable mais rajoute de la complexité. Les Européens sont divisés. Le Conseil européen de la semaine prochaine sera de la plus haute importance. Nous espérons que les résultats concrets des résultats concrets et pas une énième En effet, qu'il s'agisse de l'achat d'électricité sur le marché européen. La fixation du prix de gros, ou le découpage des prix de l'électricité et du gaz. Ces sujets sont trop importants pour attendre. Les tarifs réglementés. De vente reste le sujet majeur des débats. Et nos débats le prouve. Je soutiens l'idée que nous devons ici au Sénat, à avoir une réflexion plus approfondie dans toute sa dimension et, en particulier européenne. Ce débat commence dès, dès, dès aujourd'hui, mes chers collègues. Pour les raisons de non conformité aux jurisprudence. Au droit français et européen. Le groupe les indépendants ne peut s'associer et de s'associera pas à cette CPL merci. Merci cher collègue. J'appelle maintenant monsieur Daniel Salmon du groupe écologiste à intervenir pour 4 minutes,

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, monsieur le rapporteur, madame la présidente. L'augmentation du prix de l'énergie était déjà perceptible en 2019 mais depuis plus d'un an. De nombreux facteurs ont concouru à sa hausse exponentielle déclenchement de la guerre en Ukraine et la fin de la baisse des approvisionnements en gaz russe, auquel il faut ajouter l'indisponibilité d'une bonne partie des réacteurs nucléaires en France et la faible production hydroélectrique dû aux conditions climatiques. Mais cette crise n'est pas seulement conjoncturel, le manque d'anticipation des gouvernements successifs sur la nécessaire sobriété et le développement des ENR le choix de la libéralisation du secteur de l'énergie le tout alimenté par le mythe d'une énergie bon marché ont créé les bases de cette situation et ce manque d'investissement criant que nous devons rattraper aujourd'hui dans l'urgence avec pour résultat un MWh d'électricité qui a dépassé les 1000 euros cet été, ça a déjà été dit, soit 20 fois plus que le son prix début 2021 une crise sociale particulièrement rude pour nos concitoyens et une contrainte financière inédit sur les dépenses de fonctionnement des collectivités locales dans un contexte déjà très tendu en matière de finances locales. Ses factures d'électricité et de gaz ont été multipliés par 3 par 4 voire par 6 elles atteignent des proportions qui leur est souvent impossible d'absorber. La Fnccr a d'ailleurs évalué à 11 milliards d'euros ce surcoût pour les collectivités lié à la hausse des prix de l'énergie en conséquence non de de missions de service public sont menacés comme cette proposition de loi le souligne justement dans l'exposé des motifs. C'est pourquoi il est indispensable de soutenir l'ensemble des collectivités pour faire face à cette crise et limiter autant que possible une répercussion sur nos concitoyens avec à la clé des hausses d'impôts ou une baisse de l'offre des services publics. Nous saluons certains des dispositifs adoptés dans le cadre des récentes lois de finances, je pense à l'amortisseur électricité et l'électricité et à la reconduction en 2023 du filet de sécurité même si nous n'avons pas encore une vision très claire de ces mesures, ni une réelle visibilité sur les collectivités qui vont être directement concernés. Sur le bouclier tarifaire, cela a été dit, seuls les collectivités de petite taille peuvent encore avoir accès aux tarifs réglementés de vente. Au final, nombre de collectivités passeront à travers ces dispositifs et auront recours à des offres de marché sur des contrats d'un à 3 ans et seront donc soumises au prix du marché de l'énergie. C'est pourquoi nous souscrivons aux objectifs de cette proposition de loi, à savoir l'élargissement du TRV eux à l'ensemble des collectivités et le maintien des tarifs réglementés de vente pour le gaz, dont la mise en extinction est prévue pour le 30 juin 2023. Des dispositifs qui nous paraissent en effet bien plus lisible pour les collectivités et dont l'efficacité n'est pas à démontrer. Il permettrait de préserver dans tous les territoires, les services publics et les investissements locaux essentiels à la reprise économique et à la transition écologique.-- Nous entendons les alertes du rapporteur sur les problèmes d'application, liées au droit européen mais il me paraît important d'adopter ce texte pour envoyer un signal politique notamment auprès de la Commission européenne et de rappeler la nécessité d'une baisse structurelle des prix de l'énergie à l'échelle européenne et plus largement à réformer le marché européen de l'énergie. Permettez-moi cependant de rappeler que pour nous si les exonérations et autres tarifs réduits sont indispensables dans l'urgence qu'ils sont utiles pour panser les plaies, ils ne sont pas tenables dans la durée et très coûteux et parfois même inadapté face à la nécessaire bifurcation écologie. Ils peuvent encourager la consommation d'énergies fossiles comme le gaz, c'est pourquoi nous continuerons à défendre les indispensables mesures structurelles pour accompagner au mieux les collectivités dans la durée et leur permettent une vision budgétaire pour planifier sur le long terme.-- Ces outils nous les connaissons très bien, ce sont ceux qui enclencherait allemand la transition énergétique, la sobriété et l'efficacité énergétique. Une rénovation thermique des bâtiments plus rapide, le développement des énergies renouvelables. Nous avons. Des choses dans la boîte à outils, il faut les mettre en place au plus vite mais. Nous adhérons à cette proposition de loi de groupe CRCE et donc nous la vôtre. Même. Si la parole est à présent à notre collègue Monsieur Bernard buis du groupe RDPI.-- Vous avez 4 minutes, chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la commission des affaires économiques. Monsieur le rapporteur. Mes chers collègues.-- L'objectif de la proposition de loi présentée par notre collègue Fabien Gay mérite toute notre attention. L'impact de la hausse des prix de l'énergie sur les consommateurs que sont les collectivités territoriales, est en effet considérable. Sans trop m'avancer au lendemain du congrès des maires et des présidents d'intercommunalités. Je crois pouvoir dire que nous sommes tous, nous en sommes tous conscients dans cet hémicycle. l'urgence de la situation attire notre attention elle attire aussi et surtout celle du gouvernement car malheureusement je crois que nous ne réglerons pas la situation avec les dispositifs de cette proposition de loi. Monsieur le rapporteur. Vous l'avez suffisamment rappelé. Le mécanisme du présent texte sont contraires au droit européen. De surcroît, au delà des risques juridiques et financiers. Les collectivités ne serait pas pleinement protégés. En réalité, mes chers collègues, nous réglerons les difficultés actuelles lorsqu'au niveau européen, nous arriverons à décorrélés le prix de l'électricité du prix du gaz et surtout lorsque notre pays sera souveraine d'un point de vue énergétique aujourd'hui dans l'urgence. Notre groupe considère que l'État doit soutenir les collectivités les plus impactés. Et à ce propos, je considère que le gouvernement est au rendez vous. Si l'on prend en compte l'ensemble des dispositifs adoptés pour protéger des collectivités. Je vais citer le bouclier tarifaire pour les plus petites amortisseurs d'électricité généralisée. Peu importe la taille, le filet de sécurité, 2023 pour 2 5 milliards d'euros. La charte d'engagement des fournisseurs. La publication des niveaux de prix de référence par la Commission de régulation de l'énergie sans oublier bien sûr l'augmentation historique de la dotation globale de fonctionnement de 320 millions d'euros. Après des années de baisse, puis de stabilisation la DGF augmente pour la première fois depuis 13 ans. Tout ceci dans un contexte où la dette publique s'élève à 115% du PIB de notre pays. Contexte qui nous rappelle l'impérieuse nécessité de maîtriser notre dépense publique. Mes chers collègues. Dire que l'État peut compenser la totalité de l'augmentation de la facture des collectivités. Dire cela, ce serait mentir aux élus locaux. Le choc énergétique impose que tout le monde fournissent des efforts et je sais à quel point les élus locaux en fournissent beaucoup innove pour réduire leurs dépenses en matière de dépenses énergétiques et nous devons tous se saluer la sobriété énergétique. De nombreux élus y travaille déjà depuis longtemps.-- Pour trouver une solution pérenne. Nous devons réformer le marché européen de l'énergie. La Commission européenne doit présenter d'ici la fin de l'année une feuille de route en ce sens le bouquet énergétique des 27 pays membres est très hétérogène. Raison pour laquelle à trouver un consensus européen s'avère indéniablement difficile et là en effet le découplage du prix du gaz et de l'électricité que nous demande la France coûterait cher à d'autres pays, nous devons arriver à trouver un mécanisme qui puisse nous être favorable mais sans porter atteinte à ceux qui produisent beaucoup d'électricité avec du gaz. Nous devons ainsi créer un nouveau cadre stable européen et pérenne. Plutôt que d'appliquer des pansements nationaux non concertée avec nos alliés. L'Union européenne est un collectif, un gage de stabilité de paix de protection, une puissance économique et stratégique qui nous rend plus fort et plus attractif, soyons-en fiers pour toutes ces raisons. Si nous partageons vos inquiétudes et comprenant les raisons de ce texte. Notre groupe ne pourra pas s'associer au vote de cette proposition de loi.-- Merci, cher collègue, la parole est à présent à monsieur Jean-Claude Tissot du groupe socialiste et vous avez six minutes, chers collègues.

Madame la présidente Madame la Ministre, mes chers collègues. Tout d'abord je tiens à remercier les auteurs. De cette proposition de loi qui nous permettent une nouvelle fois de débattre et d'échanger sur les difficultés rencontrées par les collectivités territoriales pour faire face à l'explosion des factures énergétiques. Cette crise énergétique sur laquelle nous pourrions revenir à chaque débat à deux a des origines multiples et n'est pas seulement une conséquence de la guerre en Ukraine à l'illustre aussi l'échec du marché européen de l'énergie ou la course aux profits, a trop longtemps remplacé l'idée de souveraineté énergétique et de défense de l'intérêt général. La période difficile que nous traversons, que ce soit pour les ménages, les entreprises ou les collectivités est également symbolique des erreurs du modèle énergétique français avec une multitude de choix trop tardif pour des enjeux de long terme. N'oublions pas que le retard de la France en matière de développement des énergies renouvelables va nous coûter plusieurs centaines de millions d'euros pour ne pas avoir fait répondu aux objectifs contraignants de l'Union européenne.-- À ce propos, les divergences entre les États de l'Union européenne retarde fortement la prise de décision sur les enjeux stratégiques pour le marché de l'énergie, que ce soit sur le plafonnement du prix du gaz, les achats en commun ou le découplage entre le prix de l'électricité et celui du gaz. Face à tout cela. Madame la ministre des collectivités territoriales, garante du bon fonctionnement de leur territoire et de leurs services publics se retrouve acculés par des factures augmentant entre 30 et 300% pour le gaz et l'électricité. Certaines communes vont même se retrouver avec un coût annuel supplémentaire pouvant aller jusqu'à plusieurs millions d'euros par rapport à leur budget prévisionnel et la seule réponse dont disposent les collectivités et particulièrement les communes est de restreindre ou de limiter les équipements et les services publics locaux. Mes chers collègues, nous avons tous malheureusement connaissance de communes qui font le choix de fermer des locaux municipaux ou faire pour faire face aux dépenses énergétiques directes sont aussi à craindre sur le traitement de l'eau et la gestion des déchets qui sont des missions de service public particulièrement énergivores, mais indispensable à la vie en collectivité, il paraît inconcevable que les collectivités territoriales et leurs habitants subissent de manière aussi importante les erreurs stratégiques de l'État et du gouvernement. Alors oui, Madame la Ministre vous nous répondrez très certainement et vous l'avez déjà fait dans votre propos liminaire, que le gouvernement a pris toute sa part pour alléger les difficultés rencontrées par les collectivités. Dans ce contexte inflationniste, et nous ne vous donnerons pas totalement tort mais malheureusement ces mesures sont souvent trop limités, notamment par des critères pour pouvoir bénéficier du bouclier tarifaire et ont, de manière logique des dates prochaine d'arrêt, ce qui nuit à la visibilité budgétaire des collectivités. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui répond à cette logique de long terme, en permettant l'accès au tarif réglementé de vente de l'électricité et du gaz dans les périodes de crise, mais aussi lors des. Retour à la normale dans l'objectif.-- De répondre aux préoccupations des collectivités. Nous avons collectivement obtenus lors de l'examen. Lors de l'examen de ce projet de loi de finances, ceux de 2020 pour 2023 que nous venons de terminer et malgré les fortes réserves du gouvernement un élargissement du filet de sécurité pour les collectivités, même si nous aurions pu le souhaiter plus ambitieux l'amortisseur électricité qui entrera en vigueur au 1er janvier 2023 pour les collectivités non éligibles DE est une bonne nouvelle malgré que les seuils et les montants couvert aurait pu être plus large, selon nous, notamment pour les prendre notamment pour les premiers mois de l'hiver 2023 toutefois au sein de mon groupe socialiste, écologiste et républicain. Nous pensons que les tarifs réglementés de vente peuvent apporter une réponse plus. Et plus durable pour les collectivités territoriales en mettant un retour en permettant, pardon, un retour à la finalité du première déterré la protection des usagers et de tous les usagers et nous rejoignons les propos présentés dans l'exposé des motifs de ces propositions de loi. La réglementation des tarifs symbolise parfaitement la nécessité d'une intervention publique dans le secteur hautement stratégique que représente l'énergie et le nécessaire engagement de l'État pour préserver les collectivités territoriales. Ainsi, lors de l'examen de ce texte nous soutiendrons l'élargissement du bouclier tarifaire à l'ensemble des collectivités territoriales par l'accès à un tarif réglementé de vente de l'électricité décorrélées des prix du marché. Comme évoqué précédemment. C'est une mesure qui répondra à l'urgence de la crise énergétique en permettant un accès au bouclier tarifaire, le temps de son application mais aussi une réponse de long terme pour que les collectivités n'aient plus à subir la vôtre la volatilité extrême des prix du marché de l'énergie. est également une mesure de bon sens en proposant le rétablissement des tarifs réglementés de vente du gaz dans le contexte actuel. Nous savons tous. Il est inconcevable que les collectivités territoriales ne puisse plus conclure de nouveaux contrats au tarif réglementé de vente de gaz et que l'extinction définitive des TRV. prévu le 30 juin 2023 s'applique pour les collectivités, dont le contrat est toujours en cours. Alors bien sûr, lors de l'examen de cette proposition de loi en commission des affaires économiques du Sénat, nous avons parfaitement entendu les remarques. Formulées par le rapporteur sur la non-compatibilité de ce texte avec le droit européen toutefois au sein de mon groupe socialiste, écologiste et républicain. Nous soutiendrons cette proposition de loi car nous considérons qu'elle peut permettre de lancer un appel et un nouveau rapport de force au sein des négociations européennes sur le sujet de l'énergie. En effet, il est indispensable que l'énergie sont considérées comme un bien de première nécessité un bien commun dans l'organisation ne peut être laissée aux seuls marchés pour cela l'énergie doit être reconnu comme un service public ou dans le langage de la Commission européenne, un service d'intérêt économique général qui suppose une maîtrise publique de la politique tarifaire ainsi mes chers collègues. Comme vous l'avez comme vous avez pu le comprendre. Le groupe socialiste, écologiste et républicain soutiendra cette proposition de loi. Si cher collègue, la parole est à présent à Madame Marie-Noëlle Lienemann du groupe. Communiste pour quatre minutes, chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre. Monsieur le rapporteur, chers collègues. Certes, la pandémie du Covid. La situation géopolitique, on a cru la crise énergétique qui a aggravé la flambée des prix. Mais elles étaient prégnante auparavant car les causes sont structurel, la libéralisation, la dérégulation du marché européen aboutissent à des hausses régulières et forte des prix, en particulier celui de l'électricité et conduisent aujourd'hui n'a pas ce total. Accrochés à leurs dogmes ni les institutions européennes, ni les dirigeants français nous ont voulu écouter les arguments de ceux qui contestaient cette logique anticipait les dégâts et font mine aujourd'hui de découvrir ce qui pourtant était prévisible. Avec la dérégulation du marché européen et la mise en cause du monopole public a été décidée l'extinction progressive des tarifs réglementés et on envoie les graves conséquences. Les collectivités territoriales affronte donc aujourd'hui des augmentations de 30 à 30 300 % pour l'électricité, comme pour le gaz. Cette crise explose en plus au pire moment puisque vous le savez, les marges de manoeuvre budgétaires de nos collectivités leur autonomie fiscale et la capacité à maîtriser les recettes n'ont jamais été aussi faible. C'est donc tout le sens de cette proposition. Donner aux collectivités locales des soutiens pérenne que ne leur garantit ni le le bouclier tarifaire ni l'amortisseur ni le filet de sécurité. Alors, Sir collègue. On ne peut pas présenter nos intentions comme louable pour ensuite proposer un plaidoyer d'impuissance. Selon notre rapporteur cette proposition de loi ne serait pas conforme au droit européen. C'est d'ailleurs les mêmes. Qui aujourd'hui nous disent qu'on ne peut rien faire. Et qui nous disait hier. Vous allez voir la dérégulation, ça va faire baisser les prix par la concurrence. Les mêmes qui n'ont pas voulu écouter le vote de notre peuple qui se méfiait de la concurrence libre et non faussée dans le secteur des services publics et qui nous disent aujourd'hui, on peut rien faire. Or. Justement. On a vu avec la crise sanitaire. Que la certitude. Les règles européennes. Ont volé en éclats.-- Ont pu voler en éclats. Et que toute une série de règles qu'on croyait intangibles ont été du jour au lendemain. Mise en cause et transformé. C'est ce que nous proposons aujourd'hui au regard de la crise énergétique. Il est possible d'obtenir des dérogations. Il est possible d'obtenir des bifurcations dans les choix européens. Je vais donner quelques exemples. Vous nous dites les dérogations, c'est pas possible. Pourquoi l'Espagne et le Portugal obtiennent des dérogations parce qu'ils sont déterminés, ils trouvent leurs arguments. Je vous donner d'autres exemples, 200 milliards d'aides publiques de l'Allemagne à ces entreprises. Vous croyez qu'ils se sont perturbés parce que ce n'était pas conforme aux règles européennes, ça ne l'est pas. Le groupe or laine en Pologne a le monopole, tenez-vous bien, le monopole du gaz, de l'électricité et de l'approvisionnement en pétrole en Pologne une seule entreprise. Ça ne pose pas de problème de règles. De concurrence européenne. C'est tout récent. Personne n'a rien dit. Parce que face à la crise énergétique. Les pays doivent pouvoir faire prévaloir est leur intérêt général et une vision d'avenir pour l'Europe, c'est ce que nous vous proposons aujourd'hui avec ce texte. Alors vous dites, le coût est élevé. Oui le couvert. On peut on peut chipoter si je puis dire sur le chiffre, mais enfin ce sera jamais les 50 milliards. Qu'on a déjà dégagé. Pour faire face à cette crise énergétique mais surtout. Ce système de colmatage budgétaire au jour le jour.-- Qu'est-ce qu'on peut-on prévoir pour l'avenir.-- Comme les prix de l'énergie vont certainement continuer augmenter. On va mettre à la pelletée des sommes budgétaires. Au coup par coup sans avoir essayé d'introduire un système qui soit maîtrisée. Elle ce principe des tarifs réglementés. C'est ça. C'est pourquoi nous pensons que c'est une bonne solution. Nous avons aussi évidemment l'argumentaire vous conviendrez monsieur le rapporteur. Qu'il est peu crédible. De dire de faire croire que le groupe communiste est défavorable à l'avenir d'EDF et ben la fragiliser.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, madame la présidente de la commission des affaires économiques. Mes chers collègues, mes chers collègues. Chauffage, des écoles, fermeture des piscines. Appel à la sobriété énergétique nos collectivités sont aujourd'hui en première ligne dans cette crise et subissent de plein fouet les conséquences de l'explosion de la facture. Énergie. À ce titre je souhaite saluer l'initiative de nos collègues du groupe communiste et salue également le travail de notre rapporteure. Il est primordial de mettre en lumière les difficultés éprouvées joué par nos collectivités à accéder à l'énergie au prix compétitif dans notre assemblée. Je crois que nous. Partageons tous, c'est ce qui moi. Tous les Costa des auteurs de cette proposition de loi depuis le printemps 2022 et le déclenchement de la guerre en Ukraine, les prix du gaz et de l'électricité sur le marché. Connaissent une hausse record.-- Atteignant des niveaux inédits pénalisante directement l'ensemble des collectivités territoriales. En effet, l'onde de choc provoquée par la crise internationale et amplifié par notre dépendance au gaz russe à toucher les particuliers, les acteurs économiques associatifs mais également nos collectivités.-- Entré. De plain-pied dans cette économie-d'externalités que décrivait récemment Jean Pisani-Ferry. Nous ne pouvons rester muet.-- Si d'importantes dispute dispositifs d'aide ont été mises en place par l'État, à l'image du récent amortisseur électricité le contenir pas totalement. Mes chers collègues. Nos collectivités. Tire la langue avec une augmentation des prix comprise entre 30 et 300% pour l'électricité, comme pour le gars. Une explosion de la facture qui n'est tout simplement pas tenable pour des finances locales souvent fragile parfois.-- Les Les élus locaux sont démunis.-- Dans cette crise énergétique notre soutien dans nos collectivités doit être totale et l'État doit prendre ses responsabilités pour accompagner face aux répercussions néfastes de ce choc exogène. Si nous partageons donc le diagnostic établi. Nous ne souscrivons pas aux propositions que les auteurs de cette proposition de formule. En effet.-- L'extension de l'éligibilité du tarif réglementé de la vente de l'électricité à l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que le maintien du tarif réglementé de vente du gaz pour les mêmes acteurs sont un non-sens à la lecture du droit de l'Union européenne au regard notamment de la jurisprudence. Constante de la Cour de Luxembourg. Où la réalisation d'une Union européenne de l'énergie et plus que jamais nécessaire pour assurer notre souveraineté énergétique. Et la sécurité de l'approvisionnement en énergie. Il serait opportun. D'aller à rebours de celle-ci.--

Le découplage des prix de l'électricité, du gaz doit ainsi être notre priorité. En effet aujourd'hui.-- Le prix de l'électricité produite est le sur celui du gars conduisant conduisant à gonfler artificiellement le prix de l'électricité produit par les autres sources d'énergie au 1er rang desquels figurent le nucléaire et les énergies renouvelables. Cela ne peut durer. La finalisation du mécanisme de plafonnement du gars à l'échelle européenne, s'appuyant notamment sur la bourse TTF et une autre perspective que nous devons exploserait rapidement afin de contrôler l'envolée des prix. C'est un agissant collectivement avec l'ensemble de nos partenaires européens que nous réussirons à aider nos collectivités.-- En plus de l'importance d'agir structurellement au niveau continental. Cette proposition de loi. Voit se dresser devant une telle une série d'obstacles constitutionnels EDF et par exemple le seul fournisseur. À pouvoir proposer le TR EVE qui des fournisseurs alternatifs et de l'effectivité du principe de libre concurrence. Consacré par le juge constitutionnel. De plus, le calcul des tarifs réglementés pour un en compte l'ensemble des coûts fournisseur. La hausse des coûts de production et d'acheminement de l'énergie serait. Répercuter directement sur le tarif réglementé. Proposé.-- Chers collègues mais faut méfions-nous donc des miroirs Alouettes. Cette à ce titre que je salue la proposition formulée par notre collègue Franck Montaugé et le groupe socialiste en commission de déposer une proposition de résolution européenne visant à alerter le gouvernement sur l'urgence d'agir au niveau européen pour réformer le marché de l'électricité et du gaz.-- C'est pour ces raisons. Qu'avec la majorité de mes collègues du groupe centriste sans idéologie. Ni dogmatisme. Et à nous méfiant des remèdes miracles nous ne voterons pas en faveur de cette proposition de loi. Madame Catherine MacGregor PDG d'Engie hier devant la commission d'enquête visant à établir les raisons de perte de souveraineté d'indépendance énergétique de la France, déclaré à l'Assemblée nationale la souveraineté énergétique doit aussi être penchée penser pardon à l'échelle européenne. Nous devons être pragmatique et trouver une réponse adaptée et efficace aux défis de la facture énergétique afin d'accompagner nos collectivités. C'est sûr que l'ampleur du défi qui ne nous a pas je vous remercie.

Madame la présidente. Monsieur le rapporteur, madame la présidente de la commission, madame la Ministre, nous sommes assis sur une bombe, une bombe énergétique prête à exploser prête à emporter les marges de fonctionnement et d'investissement de nos collectivités locales prête à emporter des pans entiers de nos économies locales des industries électro-intensives ou dépendante du gaz comme l'était la faïencerie de Digoin obligé de fermer ses portes après 2 siècles d'histoire. Faute d'avoir pu maintenir son approvisionnement en énergie.-- Sans oublier nos artisans boulangers, bouchers pâtissiers saisi d'effroi à la vue des tarifs d'énergie pour 2023. Dans un tel contexte, je remercie le groupe auquel je suis rattaché le groupe des Républicains de m'offrir la liberté de vous exprimer ce que j'ai sur le coeur et de dire publiquement au-delà des nuances politiques ou idéologiques, le mérite que je reconnais à cette proposition de loi déposée par notre collègue Fabien Gay.-- Cette PPL qui vise à protéger les collectivités territoriales de la hausse des prix de l'énergie. Ah, d'abord le mérite d'ouvrir le débat sur les tarifs réglementés.-- Depuis plusieurs semaines des questions me semble devoir être posée sur le fonctionnement de ses tarifs sur le passage par exemple des tarifs de marché aux tarifs réglementés pour les éligible sur la définition des éligibles à ces tarifs pour desserrer par exemple les critères des 2 millions et 10 équivalents temps plein voir intégrer toutes les collectivités. Mais aussi sur le critère de la puissance installée, les fameux 36 qui avait à qui ne figure pas dans la directive européenne mais qui semble le fruit d'une sur-transposition à la française que l'on pourrait revoir pour le plus grand bien de mon boulanger.-- Le PLF pour 2023 me semblait donc être le vecteur le plus opérationnel malheureusement mes amendements ayant ont été frappé de la foudre de l'article 34 de la loi organique redéposer pour compléter cette présente, proposition de loi. Les voilà foudroyée par l'article 40, le droit d'amendement et parfois un vrai combat à défaut d'être une lutte finale. Alors oui, cette proposition de loi le mérite de pouvoir débat d'une question qui est dans beaucoup de têtes en particulier des élus locaux. Pourquoi, pourquoi cette inégalité cette inéquité pour ne pas dire cette injustice entre nos différentes collectivités entre celles qui bénéficient des tarifs réglementés du bouclier tarifaire qui leur est appliqué et celles qui sont livrés aux joies au loi de la jungle, pardon la jungle du marché de l'énergie. Je remercie le rapporteur Laurent Somon sensible, tout comme nous au sort des collectivités à qui revenait la lourde tâche de nous rappeler la réalité derrière l'espoir que pouvait représenter ce texte. Il nous a livré une analyse aussi poussé qu'attentionné du sujet. Il a bien deux décrit le cadre juridique de ses tarifs réglementés sous le contrôle intraitable de la jurisprudence européenne et du Conseil d'État français voter la PPL c'est sans nul doute se mettre en contradiction avec le droit européen actuel et risquer d'exposer nos collectivités à des contentieux que pourra engager par exemple des fournisseurs d'énergie, comme ils l'ont fait par le passé en responsabilité ce risque réel de contentieux individuel ou collectif dissuadera un certain nombre d'entre nous de voter ce texte, dont pourtant nous apprécions. L'objectif est l'égalité qu'il rétablira entre nos collectivités. Pour autant, le débat ne saurait s'arrêter là. Madame Luminaire. La ministre et c'est donc vers vous que nous nous tournons il y a urgence, urgence de qui clarifier rapidement les mesures de soutien. Le Sénat a jouer tout son rôle en faisant des propositions pour améliorer le soutien aux collectivités ou la de l'amortisseur qui pourrait diminuer les de de d'énergie de 25% quel filet de sécurité allez-vous retenir dans le texte final du 49 3 ce qu'il y aura égal accès à ce filet aux discriminations à l'entrée. Quelle année de référence. Allez vous prendre 2021 août 2022. Quel montant de l'aide, est-ce que finalement ce sera un filet un filet ou une Nasse dans laquelle les collectivités se retrouver bloqué garderez-vous notre proposition de quatrième étage avec le fonds de sauvegarde énergie pour les situations les plus désespérés.-- Il faut également clarifier les mesures de soutien pour les TPE, les PME puisque la ministre Pannier-Runacher nous disait que les collectivités les. Entreprises pardon aurait droit et à l'amortisseur et aux aides de guichets et la communication gouvernementale dit désormais le contraire. Finalement, quelle est la position du gouvernement français sur le marché de l'énergie puisque le droit européen nous contraint le gouvernement a-t-il la volonté de changer ce droit pour nous permettre la préservation et l'extension des tarifs réglementés, y compris le maintien des tarifs réglementés du gaz aux particuliers, cet été, la France va-t-elle vraiment se battre pour obtenir le découplage des prix de l'électricité du marché du gaz et, finalement, ne faut-il pas changer notre logiciel et revenir au bon sens, un système électrique, c'est un réseau et des centrales de production au regard des investissements nécessaires il ne saurait y avoir de concurrence possible sur les réseaux ni sur les centrales de production. L'enjeu est plutôt d'obtenir un équilibre parfait entre la consommation et la production indispensable pour ne pas aller au Black Out et la libre-concurrence n'est pas forcément la meilleure solution pour y parvenir pour conclure madame la présidente. Revenir sur les dogmes européens semble donc difficile mais la crise énergétique rebat les cartes et Louis Aragon ne disait-il pas qu'il y a toujours un rêve qui veille pronos donc cette PPL pour un rêve éveillé qu'il nous appartiendra de concrétiser ensemble dans les mois qui viennent, je vous remercie. Merci. Mes chers collègues la dit. Question générale est Close, la commission n'ayant pas élaboré de texte. Nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi initial article 1er, nous avons une demande d'explication de vote de madame Merci madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente des affaires économiques. Monsieur le rapporteur. Lors du débat sénatorial sur la politique énergétique de la France, du 12. Dernier j'avais déjà fait part de mon intérêt quant quant à l'éventualité d'un rétablissement des TRV pour l'électricité le Guess la considérant pertinentes pour nos collectivités. Au vu du contexte inflationniste du prix à la fois de l'électricité et du gaz sur les marchés. En effet, alors que la transition écologique les mais déjà aux prises avec un mur d'investissement colossal. Je crois qu'il est nécessaire de faire en sorte que leur capacité d'investissement ne soit pas obéré par leurs dépenses énergétiques. Je suis évidemment consciente des efforts déjà fournis par le gouvernement pour venir en aide à nos collectivités par le biais du bouclier tarifaire et de l'amortisseur électricité le Sénat est allé encore plus loin en votant un filet de sécurité dans le PLF 2023 à la fois élargi et simplifié. Ce qui était indispensable. Cependant, ces mesures vont avoir un coût considérable pour nos finances publiques et ne peuvent donc être pérenne aussi la solution du retour au TRV m'apparaît tel approprié pour prendre le relais sur le moyen terme, bien sûr, je comprends que la constitutionnalité de cette proposition de loi ou sa conformité au droit de l'Union européenne puis tête questionné pour ma part, je n'en suis pas convaincu car il me semble que l'énergie n'est pas une marchandise comme les autres, mais un bien public, de première nécessité. C'est pour cette raison que je voterai ce texte. Je vous remercie.-- Merci cher collègue. Demande d'explications de vote. Par notre collègue Madame brûle hein. Merci madame la présidente Madame la Ministre, mes chers collègues.-- Madame la ministre, vous nous avez révoqué tous les disques, enfin les dispositifs gouvernementaux pour aider les collectivités à faire face à la crise énergétique et aux sommes colossales qu'elles sont obligées de dépenser aujourd'hui. Revenons à la réalité dans un département comme celui de la Seine Maritime. À ce stade, le filet de sécurité ne concerne que 99 communes sur les 708 et donc considéré ici que les dispositifs gouvernementaux certes amélioré par le Sénat serait de nature à faire face au mur financier face. Auquel elle se trouve est une erreur. Ensuite, mes chers collègues. Certains d'entre vous. Nous explique que. Finalement, ce serait pas très bon. Ce retour aux tarifs réglementés de vente pour les collectivités. Mais alors pourquoi dans toutes les communes de France aujourd'hui sont adoptées d'émotion initiée notamment par l'Association des maires de France qui précisément demande ce retour aux tarifs réglementés de vente. Est-ce que le Sénat est-ce que la majorité du Sénat, la chambre des territoires va ce soir dire à tous ces maires que ce qu'ils demandent ce qu'ils votent à l'unanimité de leurs conseils municipaux n'est vraiment pas une bonne idée. Au point que nous là vous rejetez ici. Je pense que ce serait là aussi une grave erreur et enfin de nombreux exemples ont été donnés de possibilités. Que nous avons utilisées de déroger au droit européen, dans une période récente Nona notamment en raison de la crise sanitaire. Moi je mets en garde. Les coupures d'électricité. Donne le sentiment à nos concitoyens d'un très grand déclassement de la France. Dans ce contexte dire nous n'y pouvons rien. À cause de l'Europe. Je pense que ça pourrait avoir des conséquences politiques sociales en terme de cohésion extrêmement grave et de ce point de vue c'est aussi une erreur.

Nous n'obligerons aucune collectivité à souscrire au tarif réglementé à casser des contrats qui les placerait dans une situation juridique et économique très complexe, nous permettons à des collectivités qui se voient proposer des nouveaux tarifs à 30% d'augmentation en moyenne voire à du racket organisé puisque lorsqu'on nous on propose 300% d'augmentation de pouvoir souscrire au à nouveau tarif réglementé, ça laisse qui sont contents de leur contrat. Très bien. 2ème chose.-- Ça coûterait EDF. Oui, nous le redisons et ces chiffres maintenant, 3 milliards et demi. Mais on a entendu, personne ici lorsque la ministre de l'énergie a demandé 20 TWh supplémentaires au mois de février à EDF et lorsque ça a coûté 8 milliards R4 personne est venu ici pleurer. Donc on en est à 43 milliards entre le filet de sécurité l'amortisseur le bouclier tarifaire. On ne sait quoi donner au privé et on préfère nous donner 3 milliards et demi à EDF pour qu'ils puissent. Redonner accès à l'ensemble de nos collectivités. Et leur permettre le tarif réglementé et la dernière chose c'est sur l'Union européenne. Permettez-moi de vous dire madame la ministre, on a eu un bon cours mais l'article 26 du traité de l'Union européenne et la Cour de justice de l'Union européenne a aussi a fait des arrêts. Je le redis que sur une mission d'intérêt général et de service public, il peut exister des dérogations et on vous a redonné un certain nombre d'exemples et déjà au niveau énergétique nous même, la France a ayons.-- Des dérogations puisque un certain nombre de nos collectivités les plus petites y ont déjà accès les 200 milliards d'euros. Du Parlement. Si c'est pas une dérogation et ce que vient de redire aussi Céline. Donc il est possible évidemment de bouger et donc si nous disons que nous sommes pieds et poings liés. C'est pire que tout, c'est qu'ici, nous ne pouvons rien bouger. Si nous pouvons bouger des choses mais ce sont des choix politiques et vous voulez pas le faire. Merci la parole est à présent au président Laurent pour explication de vote.-- Oui, je voudrais donner un ou 2 arguments supplémentaires sur la question européenne. Comme le vient de le dire. Fabien, d'abord en droit c'est possible.-- Deuxièmement, nous vivons de depuis maintenant, depuis le début du Covid dans une situation où les gouvernements européens passent leur temps à inventer des règles qui n'existaient pas avant, et qui soit disant ne pouvait pas exister. nous, nous nous sommes entrés dans une situation exceptionnelle et là, à nouveau, nous sommes dans une situation exceptionnelle je cite un autre exemple sur l'énergie. Nous sommes en conflit avec la Commission européenne depuis des années sur l'hydroélectricité. La terre ne s'est pas arrêté de tourner parce que nous n'acceptons pas d'ouvrir à la concurrence les barrages hydroélectriques et heureusement que nous ne le faisons pas parce que là sinon les délestages ça serait encore pire. Donc nous ne respectons pas cette demande là il y a une discussion avec la commission européenne et rien de et le monde ne s'écroule pas. Donc arrêtons d'employer ces arguments. J'ajoute qu'hier nous étions en discussion sur le débat préalable au conseil européen et que nous a dit la ministre à propos de la discussion sur la réforme du marché de gros. Parce que vous nous dites oui mais attendez on va, on est en train d'entamer une discussion c'est que au mieux au mieux. En ayant des dispositions adoptées au Conseil européen de mars prochain. Tout ça n'entrerait en vigueur qu'à l'hiver 2024 au mieux, et encore on ne sait pas ce qu'il y aura dans la réforme du marché de gros. Donc ça veut dire que dans les 2 années à venir et les 2 hiver qui se présente, il va falloir vivre dans cette situation-là. Hé bien, si nous ne prenons aucune mesure nous allons mettre à genoux les collectivités locales avec des conséquences sur leur investissement public en général et sur leur investissement en matière de transition énergétique qui seront catastrophiques pour le pays. Donc, nous allons perdre sur tous les tableaux et enfin dernière chose, 45 milliards de bouclier tarifaire Madame la Ministre déjà aujourd'hui. S'il faut tenir 2 ans comme ça ça va coûter combien le coupe le bouclier tarifaire pas 45 milliards d'euros, soit on lâchera tout le monde en rase campagne, soit ça va coûter 150, 200 milliards au bout de 2 ans, ça va être ça l'addition. Alors par rapport à ce que nous proposons, il y a pas photo. Donc je crois qu'il faut prendre nos responsabilités et voter cette PPL.-- Merci monsieur Piednoir, vous avez demandé la parole pour explication de vote.--

la situation énergétique de notre pays, on a eu l'occasion de le faire, on a eu des questions au gouvernement tout à l'heure. Et il me semble que les uns et les autres ne sommes pas satisfaits des réponses du ministre-Lescure tout en esbroufe tout à l'heure qui nie. Les difficultés notamment sur le parc nucléaire et qui ne sont pas dues uniquement à des questions d'entretien, mais bien à des choix. Non stratégiques, j'allais dire des gouvernements successifs. Depuis, depuis le gouvernement Jospin, Voynet en 97. C'est le 1er point, donc on a des points de convergence avec le groupe communiste sur la nécessité d'avoir. Dans notre mix LR énergétique dans notre mix électrique plus précisément de la production nucléaire là-dessus. Nous sommes d'accord mais quand j'entends à brûle. Évoqué les raisons fallacieuses pour lesquels on on se on compte au contraire mes collègues tout à l'heure dans la discussion générale ont clairement exprimé les raisons pour lesquelles on on allait voter contre ça, mais on n'est pas loin de la manipulation de d'opinions et de de nos grands électeurs des des élus locaux. Lorsque vous évoquez ce que vous dit tout à l'heure en refusant cette de voter cette PPL là nous on s'inscrit en faux parce qu'on a proposé dans le PLF des dispositifs qui conviennent tout à fait aux communes qui conviennent aux élus locaux. Il appartenait il appartenait aux élus communistes de voter lorsque le groupe LR auquel j'appartiens faisait ses propositions. Il me semble que là dessus vous n'avez pas été alignée sur cette position. Donc c'est un peu le le le le chien qui se mord la queue, si j'ose dire. Vous n'êtes pas cohérent avec vos, vos prises de positions précédentes et je voulais le juste le faire remarquer.-- Madame Cukierman pour explication de vote. Merci madame la présidente, madame la ministre. Je crois que. Il faut savoir garder raison dans les arguments et donc qu'on ait des désaccords, c'est une chose. Mais l'avantage des débats que nous avons ici c'est qu'il y a les retranscriptions. Et donc. Les débats sont publics.-- puisque vous faites référence je vous invite à reprendre. De mémoire hein. Il devait être une heure et quart du matin Kant. Dans la première partie du projet de loi de finances. L'amendement proposé d'ailleurs par le rapporteur général membre du groupe LR jusque là je pense que nous sommes d'accord. A proposé effectivement la mise en place du filet de sécurité. je vous inviterai à revoir et compris ce qu'a dit mon collègue, Pascal Savoldelli, donc une heure et quart, 10 minutes après il était à peu près 1h25 en disant effectivement que nous prenions acte et que même si nous avions proposé quelque chose de plus large, nous allions le voter parce que nous pensions qu'il y avait besoin de convergence. Je vous inviterai également à reprendre mes propos lors de l'intervention générale la semaine suivante toujours un mercredi. Au moment du budget de la mission collectivités territoriales ou je saluais ce qui avait été déjà acté dans la première partie et donc proposé que nous avions voté. Donc là je crois, mon cher collègue que très sincèrement nous pourrons restons sur le fond politique sur la capacité à voir ou à ne pas avoir la volonté de remettre en cause des politiques européennes de prendre ou pas. La décision de voter ici ce soir le retour aux tarifs réglementés pour les collectivités territoriales nous avons et nous l'avons toujours eu ici, la capacité à travailler en toute Intelligence avec tous les groupes politiques et votée quand ça va dans l'intérêt général et dans le sens attendu par les élus locaux, un certain nombre de dispositifs sans aucun sectarisme de notre part, je vous remercie et donc je souhaite que ce soit bien éléments notifié pour que cela reste aussi dans la nos mémoires collectives.-- Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres demandes d'explications de vote. Madame Lienemann. Je vous invite à méditer. Sur l'évolution.-- De la richesse de la France. En Europe. Depuis 20 ans. Vous verrez que non seulement l'Europe et déclassé au niveau international. Mais la France ne fait que reculer. En termes de PIB. En termes d'industrie.-- Et même en termes globalement économique. Chaque fois. On a avalisé désaccord. Donc on nous disait qu'il était pas très bon. Mais qu'on avait pu éviter le pire.-- Une fois qu'on avait avalisé ces accords. C'est le cas des directives de dérégulation de l'énergie. Chaque fois qu'on a déjà avalisé ces accords. On nous dit après au bout quelques années on se rend compte que c'est pas bon. On nous dit il faudrait que ça change. On va se battre en Europe pour que ça change. Et puis ça change pas ou ça change tellement peu. Qu'on continue notre déclin par rapport aux autres puissances européennes. On n'est pas les seuls c'est plutôt vrai de l'Europe du Sud. La c'est bien beau de nous dire, on va revoir les règles du marché européen des règles européennes pour pouvoir avoir les tarifs réglementés. Rappelez-vous la taxe Gafam.-- Heureusement que les Américains avaient bougé on n'arrivait pas à l'avoir, on allait à la voir l'année prochaine. On l'a jamais eu quasiment. Regardez les les super profits. On peut rien faire parce qu'il faudrait que ce soit européen. Et puis il se passe toujours rien. Un an 2 ans 3 ans 4 ans je me rappelle aussi la taxe carbone au fond aux frontières pour éviter les importations etc. Il se passe rien. Il se passe, il y a aussi. Parce que la France ne cherche pas jouer un rapport de force, pas seulement au nom de son intérêt national ce qui en soi est légitime mais aussi dans une certaine idée de ce que pourrait être le la TVA européen réguler le trafic de l'électricité elle les tarifs aussi pour qu'il n'est pas dit yo-yo et qu'on sache que les investissements d'avenir sont rentabilisé en termes de décarbonation sans ses tarifs réglementés. L'Europe va globalement fragilisé et la France plus que tout autre en votant cette PPL, c'est un acte politique envoyé aux institutions. Et gouvernement pour qu'on revoie stratégiquement cette politique. Avant de donner la parole aux rapporteurs saumon je voudrais vous dire que j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par la commission sur cet article 1er monsieur le rapporteur. Vous aviez des précisions à nous donner.-- Oui, profiter de la discussion sur cet article. je ne mets pas davantage Madame Lienemann en doute le groupe CRCE du souci de protéger le l'entreprise d'EDF. Bien entendu, pas plus que je l'espère. Vous ne mettait en doute notre volonté, notre autre souci commun de protéger les collectivités territoriales et quel que soit le choix que l'on fasse par rapport à cette proposition de loi que l'on respecte cette équivalence d'intérêt pour EDF comme pour les collectivités territoriales. Mais le règlement en place des des TRV eux qui est basée néanmoins sur la ça n'échappe à personne. Coûte à l'entreprise avec uniquement l'augmentation de 100 à 120 TWh. Je vous le rappelle quand même 10 milliards d'euros. Donc c'est quand même une difficulté pour l'entreprise. À l'heure où elle a besoin d'énormément d'investissement pour remettre à niveau je dirais déjà le parc actuel et demain pour les investissements à faire, tels qu'ils sont annoncés. On attend d'ailleurs pour ce qui a été dit sur le coup que ça représentait. C'était Hervé que toutes les collectivités, on l'a évalué on va dire entre 2 5 et 3 milliards d'euros, on attend quand même parce que ça c'était fait, j'allais dire en interne on attend l'évaluation de la creux qui n'a pas pu nous la fournir et c'est important d'avoir la vie de la crue à ce sujet. Encore une fois on ne conteste pas et je pense que je partage complètement à 300%. Les propos de Fabien. Et la et de la ville de Digoin, bien sur. La nécessité de réviser la fixation du prix de l'énergie sur le le le le prix du enfin le taux marginal qui est basé, lui-même sur le prix du gaz tant qu'il était bon marché, tout le monde s'est retrouvé, une fois effectivement qu'il est élevé. Il y a de grandes difficultés et c'est la crise que nous connaissons aujourd'hui. Mais on doit le faire et on est tous d'accord là-dessus pour c'est que on doit le faire d'une manière sécurisante à la fois financièrement et juridiquement pour l'ensemble des collectivités locales, ne l'oublions pas. Et bien sûr on ne peut pas échapper au contexte tels qu'il est aujourd'hui c'est un contexte de libéralisation que chacun pourra juger en âme et conscience. Voilà j'en dirai pas plus, mais faire croire que la solution la panacée. La solution ultime, c'est de revenir aux tarifs réglementés. Je voudrais quand même cité la Fnccr qui représente aussi les collectivités territoriales qui distribue.-- Je la cite le retour au TRV d'énergie ou de gaz ne permet donc pas de garantir à lui seul des niveaux de prix économiquement raisonnable et socialement acceptable pour les consommateurs.

La présentation un peu rapide et qui paraît tellement séduisante qu'elle est simple mais qui va être très coûteuses et très risqué pour les collectivités locales.-- Merci Madame la Ministre, vous avez demandé la parole pour des précisions également.-- Merci madame la présidente. Donc, juste quelques mots. Pour dire que en fait. Il y a 3 phrases que j'ai noté et je voudrais juste m'inscrire en faux au niveau du gouvernement, je n'ai jamais dit je ne crois pas que le rapporteur et dit qu'on ne pouvait rien faire. Je ne crois pas avoir dit nique le rapporteur et dit qu'on ne pouvait rien bouger, je ne crois pas avoir dit que nous souhaitions d'une façon ou d'une autre mettre à genoux les collectivités locales et je ne crois pas qu'. On puisse dire qu'il ne se passe rien c'est quand même juste de 5 milliards d'euros qui sont investis. Pour essayer de faire en sorte que les collectivités parce cette crise énergétique. Ensuite je voudrais pas de d'interprétations hâtives non plus pas de procès d'intention. Si vous le voulez bien. Et dire que le Sénat qui cette chambre des territoires comme vous l'avez dit. Mesdames. Dire que même ceux qui voteront contre. Votre PPL dont j'ai dit que, elle était intéressante en soi dans les objectifs qu'elle poursuivait. il ne faut pas. Stigmatiser dans cette assemblée, ceux qui ne souscrivent pas parce que s'ils ne souscrivent pas comme le gouvernement, c'est tout simplement pour des raisons juridiques, comme cela a été dit il y a d'autres façons de faire bouger l'Europe sur ces sujets, je crois que le président démontre qu'il aimait beaucoup d'énergie et de talent pour pour essayer de faire changer les choses. C'est juste pas le moment aujourd'hui, même si c'était le moment pour vous au niveau de de votre niche Monsieur le Sénateur merci.-- Merci. J'ai donc été saisis comme vous je voulais préciser d'une demande de scrutin public par la commission. Il va être procédé à ce scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est donc ouvert.

Le scrutin est donc clos.--

merci. 96 sur l'article numéro de compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordé par les sénateurs, groupes politiques et notifié à la présidence. Nombre de votants, 343 Nombre de suffrages exprimés, 330 pour l'adoption, 98 contre 232, le Sénat n'a pas adopté l'article 2. Nous allons passer à l'article de. Je vois qu'que si cet article 2 n'était pas adopté, il n'y aurait donc plus lieu de voter sur l'ensemble de la proposition de loi, puisqu'elle est constituée, seulement de 2 articles. Dans la mesure.-- Où est-ce. Suivant, comme je vous le dis, ces 2 articles seraient supprimés il. Pas donc d'explication. De vote sur l'ensemble de la proposition de loi. Donc si vous avez une demande de parole d'explication de vote. C'est maintenant, chers collègues. Après le sujet serait clos.-- Donc. Avant de mettre aux voix cet article de.-- Pour lequel il a été demandé un scrutin public par la commission. Y a-t-il des explications de vote, monsieur Guy.--

D'ailleurs on n'a pas dit ça. C'est des choix politiques. Qui sont pas les mêmes face à une situation. Donnée. Nous, nous prenons l'efficacité. Et le public et il y a un choix qui est fait, on, on verra l'efficacité de donner beaucoup d'argent public à des acteurs alternatifs. Pour des résultats. Par exemple, ça a coûté des milliards pour imposer le bouclier tarifaire à 4%. Résultat. 5,4%. C'est-à-dire que donc. Il y a des acteurs alternatifs qu'ont pris l'argent public pour imposer un bouclier tarifaire qui n'ont pas respecté. Est-ce que par exemple. L'État va demander le remboursement de cet argent public. Deuxièmement, puisque nous sommes sur le gars. Nous vous le redisons l'extinction pour tous les usagers. Du gaz au 30 juin est une catastrophe en plein moment où le prix du gaz est en train de s'envoler et son approvisionnement n'est pas sécurisé. Est ce que nous nous mettons d'accord pour prolonger les tarifs réglementés du gaz pour l'ensemble des s'usagers c'est une question, elle va nous être posée. Et donc nous nous mèneront la bataille dans les 6 prochains mois qui nous reste, parce que nous pensons. Au delà des collectivités. On a entendu et à juste raison les TPE-PME. Les commerçants, les boulangers qui. Manifesteront le 23 janvier prochain et nous serons à leur côté, qu'il y a besoin sur cette question là de nous mettre d'accord.-- Vous voyez bon bé nous vous remercions de nous avons déposé nous aussi. Un scrutin public sur cette question et quoi qu'il arrive. Du vote du Sénat. Au final, nous continuerons à porter évidemment ce combat politique, notamment sur la question des temps à effet réglementé, mais aussi pour un monopole public et une entreprise publique qui a les capacités d'investir 10 nommé et évidemment. De répondre. Aux défis du XXIe siècle, notamment sur la question de la précarité énergétique. Je vous remercie.

Oui, rapidement. Merci la la présidente. Je souhaite intervenir parce que c'est le dernier moment pour, pour le faire parce que je crois que chaque fois que nous pouvons saisir une occasion, une opportunité de faire remonter ce qui se passe sur le terrain, c'est absolument indispensable et c'était l'un des mérites, je l'ai déjà dit de cette PPL il y a pas forcément qu'une différence de choix politique. Il y a aussi. Une sorte de prudence à ne pas. Faire croire aux. Aux responsables de collectivités locales qu'il suffirait qu'on vote ici un texte pour que tout soit résolu et je crois que dans ce moment de crise que nous vivons et qui va aller qu'en s'amplifiant. Nous avons besoin de faire très attention aux paroles publiques qui sont les nôtres mais puisque je parle de parole publique. Je voudrais redire Madame la Ministre que. Sur les soutiens, je je conçois tout à fait que nous avancions un peu dans le brouillard. Dans le brouillard bien sûr des dispositifs qui ne sont encore pas précisé dans le brouillard également de la réalité des collectivités locales puisque même les aides 2022 on aura une vision très claire de la situation qu'au vote du compte administratif, c'est-à-dire à la mi-année 2023 ce qui ne facilite pas l'adaptabilité des dispositifs pour 2023 et je pense que, à l'été 2023, nous aurons certainement remettre peut-être. La la copie sur le métier pour vraiment adapter les dispositifs mais puisqu'on vient de parler des boulangers. Je rappelle quand même que lorsqu'on lit votre le communiqué de presse de de vos collègues qui donne le cas type Inde de la boulangerie, on nous explique très bien qu'il y a un certain nombre d'aides qui vont. Pouvoir s'appliquer en particulier l'amortisseur mais le boulanger, il va rester quand même avec 75% de l'augmentation de sa facture à payer, et c'est ça aujourd'hui qui inquiète beaucoup la population c'est que certes il y a des il y a des soutiens l'amortisseur c'est 25% mais il reste des sommes considérables l'énorme énorme à payer les collectivités bah il y aura effectivement toujours l'état ou pour être derrière, mais moi. Notre crainte, c'est que vraiment un certain nombre d'acteurs économiques disparaissent disparaissent dès le début de l'année 2023 et je je rejoins Fabien Guez sur l'inquiétude de nos concitoyens qui sont au tarifs réglementés du gaz qui reçoivent ces quantités de courriers où on leur dit c'est fini allez voir les les entreprises dans le contexte actuel c'est excessivement anxiogène.-- pour explication.-- Chers collègues, voilà je vais y arriver. D'abord moi, je voudrais remercier le goût pour le débat qu'on a eu aujourd'hui. Vraiment et remercier tout particulièrement Fabien gay dont chacun connaît l'engagement sur les matières. En la matière énergétique sur le la sauvegarde d'EDF et donc je ne fais de procès à personne ici dans les effets de bord de la PPL qui sont déposées et que chacun à notre place nous apprécions à à leur valeur. Je voudrais vous remercier parce que c'était un débat et je voudrais répondre à, à Jean-Pierre Grand lui disant le débat commence pas aujourd'hui le débat il a commencé depuis des

il faut attendre maintenant la crise pour peut-être y aller encore plus fort, mais en tout cas je veux dire à notre collègue Jean-Pierre Grand, que le débat évidemment ne commence, mais il ne s'arrêtent certainement pas aujourd'hui et je prends évidemment la proposition de notre collègue Franck Montaugé sur la proposition de résolution européenne sur laquelle nous allons travailler dès cet après-midi. Je voudrais dire qu'ici, personne n'a le monopole de la défense des collectivités territoriales et que contrairement. À mon collègue Fabien Gay. Dont chacun sait voilà que je l'apprécie pour la clarté de ses convictions qui sont pas forcément les mêmes que les miennes mais peu importe. Que que chaque. Aucun. Ce n'est pas un problème politique, je crois que ce n'est pas aujourd'hui un problème politique. Nous cherchons tous à protéger les Français, notre économie et les collectivités territoriales de ce qui est en train de se passer sur l'énergie et notre différence entre nous et vous c'est peut être la méthode, vous avez une méthode aujourd'hui qui est audacieuse qui est forte et que nous nous considérons comme dangereuse pour les collectivités territoriales et présentant des risques, nous pouvons avoir des écarts de de nuances et de de d'analyse sur ce sujet mais je crois que la la la différence entre les groupes n'est pas une différence politique, elle a une différence de méthode. Voilà, alors maintenant je me retourne vers vous Madame la Ministre de la balle est chez vous. Nous nous donnerons tous nos efforts pour donner les forces nécessaires au président de la République pour aller négocier en Europe la modification de l'architecture. Du prix de de l'énergie car il n'y a que cela. Qui peut nous aider et nous protéger. Il n'y a que cela, donc nous y allons nous y allons en bon ordre et nous y allons avec force et nous attendons vraiment du gouvernement et du président de la République des résultats et des résultats qui soient plus rapides que ceux qui nous ont été annoncées hier soir dans le débat, c'est une question de survie pour notre pays et de survie pour notre rang, comme le disait Marie-Noëlle Lienemann tout à l'heure.-- Merci madame la présidente. J'ai donc été saisie de.-- Oui, chers collègues. Allez-y. je vais juste dire quelques mots on en serait peut-être pas là si honorée. Rester à la nationalisation. De certains services publics. Je pense que on on on serait pas arrivé là on a dit aux gens allez. On va prendre du privé ça ira mieux, vous verrez il aura la concurrence on aura des meilleurs prix. Le résultat on le voit aujourd'hui.-- Tim madame la sénatrice. Je mets donc aux voix. Ayant été saisi de de demande de scrutin public par la Commission et par le groupe CRCE. Le scrutin est ouvert.

Résultat du scrutin numéro 96 sur l'article numéro de compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordé par les sénateurs, groupes politiques et notifié à la présidence. Nombre de votants, 343 Nombre de suffrages exprimés, 330 pour l'adoption, 98 contre 232, le Sénat n'a pas adopté l'article 2. En conséquence, la proposition de loi n'est pas adopté. Je vais suspendre la séance quelques instants pour permettre à chacun de s'installer pour l'examen du prochain point à l'ordre du jour. La séance est suspendue, chers collègues.

La séance est ouverte. Bonjour monsieur le Ministre bonsoir. L'ordre du jour appelle donc l'examen de la proposition de résolution. Pour le développement du transport ferroviaire présenté en application de l'article 34 1 de la Constitution par monsieur Gérard Lahellec Madame Marie-Claude va. Et plusieurs de leurs collègues. Il s'agit d'une demande du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste dans la discussion générale. La parole est à notre collègue monsieur le sénateur Gérard Lahellec auteur de la proposition de la résolution. Et vous avez 10 minutes chers collègues pour vous exprimer. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues. Et tout le. Il n'y aura pas de transition écologique sans le train.-- Il n'y aura pas de train sans que notre pays le décide. Enfin de financement fortement accru et garanti sur le long terme. Nous faisons notre cette formule de Jean Rottner, président de la région Grand-Est et il est vrai que la, le ferroviaire et la colonne vertébrale de la mobilité verte. Tout le monde sans exception s'accordent pour dire qu'il faut défendre le transport ferroviaire qui constitue la Pierre angulaire de la stratégie du développement des transports des personnes et des marchandises. Dans le cas du débat de la semaine passée. Se rapportant donc à la loi de finances pour 2023. Les 3 rapporteurs spéciaux de la commission des finances, ici. Et notre collègue. Rapporteur de la communication, aménagement du territoire et développement durable. N'ont pas manqué de pointer. Je les cite la trop grande faiblesse des moyens accordés au développement du ferroviaire. Et nous n'avons d'ailleurs pas manqué de voter ici. Des amendements et singulièrement un amendement consistante à augmenter la part a consacrés au ferroviaire.-- Le gouvernement s'est également montré confiant et c'est d'ailleurs engagé à apporter des financements en conséquence. Une fois des études complémentaires réalisés pour je cite. Faire mieux. Plus et plus vite. Fin de citation. Et les déclarations récentes de monsieur le président de la République en faveur du développement des TER métropolitain ou RER dans les métropoles de France. Ne constitue au fond. Que la confirmation des ambitions qu'il convient de nourrir pour la desserte de nos territoires et de nos villes. Ce développement doit être un développement solidaire harmonieux et. Nous savons que le mode de transport retenu sera le mode ferroviaire. Mais ça ne peut en aucun cas être un type d'aménagement. Qui opposerait ville et campagne qui opposerait l'urbain à la ruralité. Il ne faudrait pas que demain nous ayons. Le rail des villes et de l'autre côté le rail des chants. Comme le disait en d'autres temps. Un beau slogan prix publicitaire. Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous, Pour y parvenir, nous avons besoin de changer de paradigme et de nourrir une grande ambition publique sans laquelle rien ne sera possible et nous ne pourrons y arriver sans le soutien de l'État à l'ensemble des autorités organisatrices de mobilité et je et je pointe au passage tout de même les dispositions qui ont été annoncés hier évidemment auxquels nous ne sommes pas insensible. Le ferroviaire qui est donc le mode de transport écologiquement le plus vertueux et le seul mode qui paie l'intégralité de ses coûts et le cas pour En ce temps de crise de l'énergie, réaffirmant que le faire et plus résiliant que l'aérien et la route et il serait d'ailleurs légitime de reconnaître les experts et les externalités négatives des autres modes quand il s'agit d'aborder le coût réel du ferroviaire. La transition sera aura aussi des incidences une incidence sociale qui peut s'avérer positive et il faut pour cela que les tarifs du train soit attractif. Quand on sait que un véhicule individuel avec l'assurance d'entretien de carburant coûte en moyenne de 5000 euros par an aux automobilistes. Le transport ferroviaire n'est pas seulement écologique. Il est donc aussi un soutien majeur au pouvoir d'achat des Français, à condition que nous nous en donnions les moyens. Alors malgré la reprise de la dette. Les 35 milliards de la dette de la SNCF réseau. Les fonds de relance vers le fret et les trains de nuit. Nous savons qu'il manque au moins au minimum 1 milliard d'euros par an aux gestionnaires d'infrastructures pour envisager un maillage équilibré, donc du territoire et offrir une alternative de mobilité à nos concitoyens. Et comme nous raisonnons sur le long terme. Il lui était raisonnable de commencer tout de suite. Ce fut d'ailleurs je le dis au passage. Un des amendements que nous avions soumis au débat initial vendredi dernier en séance publique ici même. Nous savons que notre réseau vieillit. 29 ans de moyenne d'âge, contre 17 ans en Allemagne. Accélérons donc la régénération et sa modernisation pour augmenter la sécurité et les fréquences sur décision avec une vraie stratégie qui n'est pas aujourd'hui suffisante. Nous ne pourrons donc pas nous contenter de considérer. Que 7 ans. Se contentant d'ouvrir cette activité à la concurrence que leur répondra aux besoins de modernisation du réseau au développement des territoires et au sauvetage des petites lignes ferroviaires. Du reste, on remarquera que les initiatives locales et solidaire et autres coopératives ferroviaires qui ont émergé. Dans des dites des territoires qui nourrissent des ambitions de réouverture de certaines lignes se heurte aussi à des difficultés résultant d'une insuffisance de moyens affectés à la réhabilitation des infrastructures. Il y a donc cet enjeu industriel favorable à l'emploi que nous devons soutenir par la relance et la pérennisation de filière utiles à notre économie, enfin. Pour mesurer les limites du Paris de l'ouverture à la concurrence. Il suffit de se référer à ce qui s'est passé dans le fret ferroviaire pour constater que il y a loin de la coupe aux lèvres. Aujourd'hui tout le monde s'accorde pour reconnaître que si rien d'exceptionnel n'est fait au plus vite des objectifs annoncés pour 2030 ne seront pas atteints. Ni pour le fret, ni pour le transport des voyageurs. Des petites lignes risquent d'être. Des réseaux ne seront pas entretenues. Donc, les objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre seront également manqué. Plus près de nous dans le cadre du débat autour de la loi climat résilience et dans le cadre d'une mission d'évaluation conduite par le Sénat. Des pros qui des préconisations ont été retenus dans la perspective de la reconquête du transport ferroviaire, qu'il s'agisse du fret tous des voyageurs d'ailleurs. Pour aller dans ce sens depuis le débat sur le projet de loi modificatifs 2022 toutes les composantes politiques du Sénat sont intervenus pour pointer cet objectif. Ce fut encore le cas la semaine passée lors du débat sur la loi de finances pour l'année 2023. La présente. PPR nous dodo. L'occasion d'y revenir. Et l'argument de la reprise de la dette ne doit pas être utilisée pour s'interdire de nouveaux investissements ni pour s'interdire le nécessaire développement du ferroviaire en France comme en Europe. La résorption de la dette doit maintenant se conjuguer avec le développement du mode ferroviaire et telle est bien l'ambition que se fixe cette PPR. Merci de votre attention.-- Je voudrais avant que nous commencions la discussion générale vous rappeler que les interventions des orateurs dans la discussion générale Val. Explications de vote pour votre groupe.-- Donc nous allons poursuivre par cette discussion générale. La parole est à monsieur Didier Mandelli du groupe les. Républicains. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je me réjouis que nous puissions parler une nouvelle fois du transport ferroviaire, dans cet hémicycle. La proposition de résolution du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste met en lumière des enjeux. Et les enjeux du rail en matière d'aménagement du territoire d'approvisionnement notre chaîne logistique de mobilité des personnes et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le transport ferroviaire mais est en effet chacun le sait ici 9 fois moins de CO2 à l'attendre à la tonne transportée, que la route. Ce n'est pas mon éminent collègue Philippe Tabarot rapporteur du budget transport qui me contredira. Il le confirmera sans doute tout à l'heure bon la dernière intervention de ce, de cette discussion. On ne parle jamais assez du rail. Cependant, comment ne pas être dubitatif en entendant les annonces du président de la République sur la construction du nouveau RER quand on sait sur ces bancs qu'il manque des financements importants pour l'entretien du rayon France. De la vie de tous les acteurs du secteur, les montants prévus en matière de régénération du réseau par le nouveau contrat de performance entre SNCF réseau et l'État sont très insuffisants, ils ne permettront. Même pas d'enrayer la spirale de dégradation de ce réseau. Où sont passés les engagements d'investissements voter dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités, dont j'étais le rapporteur. et la perspective d'une enveloppe quinquennale en progression à 14,3 milliards d'euros sur la période 2003 2023 pardon 2027. Qu'en est-il. Nous avions choisi de ne pas voter la CMP qui n'avait pas donc été conclusive en raison de l'absence. Des financements nécessaires notamment pour pour les AOM qui prenait la compétence. Le temps nous a donné raison, nous en sommes là aujourd'hui à l'horizon 2040 et faute de moyens, les ralentissements sur le réseau structurant classique risquent d'augmenter de plus de 50%. Combien de fois faudra-t-il tirer la sonnette d'alarme pour être entendu, faudra-t-il attendre. D'être au au pied du mur, comme en matière de nucléaire. Pour réaliser l'erreur de ne pas avoir accordé les fonds suffisants au moment où il a fallu faire. La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable là toujours portée avec constance des ambitions fortes en faveur du développement du transport ferroviaire. Notamment à travers le rapport d'un fonds mation sur le transport de marchandises face aux impératifs environnementaux avec l'idée de lancer un plan d'investissement massif en faveur de la régénération et du développement des réseaux faire ferroviaires et fluviales par la même occasion. De même.-- La loi climat et résilience, dont l'article 131 entendus en commission par.-- Le même Philippe Tabarot fixe l'objectif de doubler la part modale du fret ferroviaire aujourd'hui de 9% d'ici à 2030. Je me satisfait donc de voir que sur ce sujet. Tous les groupes partagent les mêmes constats forcément et les mêmes préoccupations et les mêmes objectifs. La proposition de résolution reprend notamment plusieurs points que nous portons régulièrement comme la réduction du taux de TVA sur l'achat de titres de transport. D'ailleurs dans ce projet de loi de finances. Le soutien en train de nuit et aux petites lignes et surtout la nécessité de réviser le contrat de performance est à SNCF. Réseau que je viens d'évoquer. Le texte que nous étudions aujourd'hui n'aborde néanmoins pas de points que sont l'ouverture à la concurrence et la nécessaire gestion des conflits et revendications salariales comment inviter les Français à choisir massivement le rail. S'ils sont régulièrement méprisé par les organisations syndicales qui les utilisent comme boucliers aux monnaie d'échange. Ce qui est une nouvelle fois le cas en cette fin d'année si cher au coeur des familles de France. L'absence de ses 2 points dans cette proposition ne nous permettra pas d'y donner une suite favorable. Notre groupe s'abstiendra avec la plus grande bienveillance. Chers collègues, je vous remercie.-- Merci la parole est à présent hein. Monsieur Jean-Pierre Grand. Pour le groupe des Indépendants pour 4 minutes, chers collègues.-- Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. D'emblée, je, je souhaite. Préciser que nous sommes tous en faveur du développement du transport ferroviaire dans le pays. Mais cette pépère. Il faut politique. Ne répond pas à l'objectif que nous partageons. Le ferroviaire et l'une des solutions clés pour l'écart Bombet efficace par le transport je rappelle les engagements internationaux, européens et nationaux pris en la matière. Pour pour la neutralité carbone à l'horizon 2050. Nous avons aussi noté des évolutions importantes dans le dernier projet de loi sur la question du ferroviaire et notamment du fret et de l'intermodalité, je pense en particulier à la loi climat résilience. Le président de la République, le gouvernement a récemment fait des annonces sur le ferroviaire ceci et d'ailleurs dans l'exposé des motifs. je pense à l'annonce du lancement d'un projet de 10 RER dans les grandes métropoles si je salue cette annonce beaucoup de questions se posent. Certaines villes en désaccord région métropole déjà avancé comme Strasbourg, Bordeaux, je crois savoir que Toulouse il travaille également sur le Ministre vous comprendrez que je vous signale particulièrement la métropole de Montpellier.-- Particulièrement.-- Qui souhaitent légitimement être incluse dans ses projets compte tenu de ses efforts massifs, un investissement d'investissements Cependant on ne peut pas avancer sans faire un inventaire précis des disponibilités techniques par métropole à nouveau. Je prends l'exemple. Dans mon département. Qui dit RER multiplication des stations D halte TER et RER et des gares intermédiaires. Mais quid des sillons. Nos lignes sont déjà terriblement sollicités avec des conséquences techniques que nous connaissons pour le trafic. Nous devons être précis sur nos besoins en infrastructures intermédiaires. Aussi j'en profite pour vous rappeler toute l'importance de la ligne à grande vitesse Montpellier Perpignan pour accélérer les projets simplifier les procédures comme bien d'autres acteurs de terrain j'imagine sur ce sujet, Monsieur le Ministre, comme sur d'autres, comme sur d'autres j'imagine une grande loi d'accélération comme a su le faire la Ve République, quand elle l'estimait d'intérêt national.-- Les besoins sont là et les exigences climatiques aussi on ne peut pas attendre 20 ans pour sortir On ne peut pas attendre 20 ans, ce sur n'importe quel projet d'infrastructure c'est plus c'est plus possible aujourd'hui. Cette PPR aborde le prix du billet de train à la crise énergétique a mécaniquement des conséquences sur les prix de transport, Monsieur le Ministre, le groupe les indépendants. Vous avez posé le mois dernier les questions sur le sujet du prix de vie, Mon groupe avait relevé l'absurdité de constater que le sang sport en commun le moins carbonée est aussi l'un des plus cher ce sujet mérite des réponses comme pour les multiples annulations des trains qui est perdu qui perturbent la vie quotidienne des des Français quand on parle de développement de transports ferroviaires. Nous devons aussi examiner des options concernant la modernisation et l'extension des infrastructures pour gagner un maillage territorial et en sillons c'est essentiel

le ralentissement mécanique et que cela induirait hein. Dans pour les lignes à grande vitesse et et le et les trains du quotidien. Depuis la mise en service de la première ligne de chemin de fer de France en 1827, le rail rythment la vie des Français aujourd'hui fidèle à cette belle histoire. Soyons les révolutionnaires du rail. Mais cette révolution en ce début de 21 siècle est trop sérieuse pour la confier à notre à cette seule PPL.-- Je vous remercie, cher collègue, la parole est à présent à monsieur Jacques Fernique du groupe écologiste et vous avez 4 minutes, chers collègues. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, chers collègues. Le ferroviaire est une réponse à beaucoup d'enjeux, la mobilité, d'abord la réduction des ségrégations spatiale, la fin des énergies fossiles, le pouvoir d'achat. La reconquête industrielle, il est un vecteur. Ça a été dit de la transition écologique. Notre groupe salue donc cette initiative de nos collègues du groupe communiste et la votera sans un changement de braquet. Les prochaines années seront marquées par un déclin inexorable de la performance du réseau. Ce n'est pas moi qui le dis c'est SNCF réseau aujourd'hui votre politique globale des transports est loin d'apparaître structuré pour parvenir à l'objectif ambitieux de doublement de part modale d'ici 2030. Autant pour les voyageurs que pour le fret. Pour le fret. Atteindre cet objectif de doublement nous permettrait juste il faut le noter, de rejoindre la moyenne européenne actuelle, c'est-à-dire 20% sachant que l'objectif européen pour 2030 et de 30%. Alors certes, votre gouvernement a commencé à répondre au manque d'investissement criant ces dernières décennies mais le contrat de performance avec les 2, 8, 9 milliards d'euros par an pour SNCF réseau dont une bonne part, il faut le noter, dépend de la hausse forte programmée des péages ferroviaires déjà parmi les plus chers d'Europe. C'est de 9 milliards d'euros par an, c'est insuffisant. Il faudra aller plus loin. Vous le dites vous-même mais on sait un tiens vaut mieux que 2, tu l'auras bien sûr le tant attendu rapport du conseil d'orientation des infrastructures sera déterminant, outil de référence pour qu'une loi de programmation ferroviaire planifie l'effort et pour que nos collectivités en concertation planche sur la définition, la déclinaison et le déploiement de projets structurants pour nos territoires le redéploiement.-- D'un véritable réseau de trains de nuit en France et vers l'Europe devra être intégrée à cette programmation pluriannuelle. On ne peut en rester pour les trains de nuit à de lignes. La Commission européenne vient d'ailleurs de donner le feu Vert à l'interdiction en France des liaisons aériennes inférieures à 2h 30 mais non sans relever que sur les 6 liaisons qui pourraient. Être dans ce cas trois seront exclus du Champ de la mesure du fait de l'absence d'une alternative ferroviaire adapté sans changement urgent de braquet, de nombreuses lignes risque de dépérir en 25 ans, nous avons perdu l'équivalent du réseau ferroviaire suisse en France le réseau ferroviaire, on le sait est vieillissant et pour sa modernisation pour garantir une offre de transport équilibré structuré aucun modèle de financement durable n'a vraiment été défini. On paye ici d'une certaine façon le renonce le renoncement historique à rééquilibrer la concurrence rail route par la redevance pesant sur les donneurs d'ordre du fret routier c'est pourtant là un des leviers des réussites de transfert modal. Ailleurs en Europe. Au lendemain de nos débats budgétaires aucun basculement d'ampleur, je le disais, vers le ferroviaire ne se lit de façon précise à ce titre puisqu'il n'a pas été politiquement possible d'actionner le levier du versement mobilité le vote visant à réduire le taux de TVA à 5 5 pour les titres de transport. En soutien à la hausse des coûts de l'énergie à laquelle les opérateurs doivent faire face doit absolument devrait passer on qu'on le voudrait à la CNP. Il est vital de prendre des mesures exceptionnelles pour maintenir ses services publics essentiels des transports en commun du quotidien pour éviter le signal désastreux qu'aux aides au carburant des autos soliste correspondent les hausses des tarifs des transports en commun dans ce sens l'aide qui vient d'être annoncée de 300 millions d'euros, 200 pour Paris sans pour les régions va dans le bon sens. Assurément, car sans soutien au secteur ferroviaire. C'est la part du train qui s'érodera en rayon cette dérive construisant avec les a ôter avec les territoires, les stratégies et les moyens du choc du ferroviaire. C'est la voie ouverte par l'euro métropole et le Grand-Est qui en mettant en service ces jours-ci leur réseau Express métropolitain réalisent le potentiel de développement ferroviaire et intermodal rendue possible par le renforcement d'infrastructures obtenue par feu la région Alsace et et coproduit par l'Europe, l'État et la région en disant que cette ténacité cette coopération positive puisse inspirer la que l'action publique nationale et décentralisé pour construire dès maintenant ce renouveau ferroviaire. Merci cher collègue. La parole est à présent à monsieur Michel Dagbert pour le groupe RDPI et vous avez 4 minutes, chers collègues.-- Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Ce texte est un appel à une ambition forte dans le domaine des transports ferroviaires que nous partageons très largement il est en effet nécessaire d'avoir un engagement important dans ce domaine, les enjeux étant à la fois écologiques, économiques et sociaux. Je voudrais tout d'abord rappeler que la France est le pays de l'Union européenne qui a le taux d'investissement le plus important en matière de ferroviaire. Dans le projet de loi de finances pour 2023, plus de la moitié des crédits alloués pour l'ensemble des transports sont affectés au ferroviaire, ce qui représente pas moins de 6 milliards d'euros et que 85% des crédits inscrits au programme 203 Infrastructures et services de transport sont consacrés au ferroviaire.-- Le budget de la FIDE quant à lui a été revalorisé à hauteur de 150 millions d'euros. Cette résolution insiste sur la nécessité d'assurer la régénération du réseau. Nous ne pouvons que partager cette ambition là encore mais le contrat de performance signé entre l'état et SNCF réseau prévoit un investissement en augmentation pour atteindre 2,9 milliards d'euros pendant. Les 10 prochaines années, ce qui constitue un effort sans précédent et il faut en prendre acte. S'agissant du fret ferroviaire. Celui-ci doit sans aucun doute être soutenu comme le préconise le texte proposé pour cela. Je rappelle qu'une stratégie nationale a été d'ores et déjà établi il y a un peu plus d'un an et il est prévu un milliard d'euros d'investissements jusqu'en 2027 des aides. Différentes. Aides ont été mises en place également. Je pense notamment à l'aide sur l'Eawag 11 isolés, ils sont prévus jusqu'en 2024 pour un montant de 170 millions d'euros par an et le gouvernement vient d'annoncer qu'ils seront chez elles seront prolongées jusqu'en 2027. L'État porte ainsi la volonté de doubler la part du transport de marchandises via le ferroviaire en le faisant passer de 9% en 2019 à 18% en 2030 pour atteindre 25% à l'horizon 2050. Pour les transports de voyageurs les transports du quotidien et les petites lignes des protocoles d'accords ont d'ores et déjà été signés entre l'État et 8 régions pour investir dans près de 6000 kilomètres de voies afin de les les préserver les entretenir, voire même parfois les rouvrir. J'en veux pour preuve l'inauguration lundi prochain de la réouverture de la ligne Gap-Grenoble. Depuis février 2020, date du premier accord 550 millions d'euros ont été déployés par l'État pour les petites lignes auxquelles s'ajoutent les financements régionaux bien sûr les financements consacrés aux petites lignes ont donc triplé depuis 2020 et ces dernières seront de nouveau présentes dans les contrats de plan État-Région 2023 2027 vous le voyez ce chantier se poursuit dans un dialogue constant et étroit avec les régions. Quant aux trains de nuit là aussi. Des initiatives ont été prises, plus de 100 millions de crédits sont prévus au budget pour 2023 et des commandes de voitures sont programmées l'année prochaine nous nous félicitons par exemple du retour de la palombe bleue qui rouvre. qui retrouvera nos plaines landaise et nos vallées du Pays basque. Tous les jours en 2024 mais il nous faut souligner que pour répondre simultanément à 2 injonctions contradictoires, à savoir le développement du fret et des trains de nuit et la régénération d'autre part du réseau nécessitant des travaux ceci s'effectue justement bien souvent la nuit. La proposition de baisser le taux de TVA sur les billets de s'apparente à une fausse bonne idée car il n'est pas certain que les AOM décisionnaires la répercute en totalité. De plus, elle entraîne un coût conséquent pour les finances publiques jusqu'à un milliard d'euros selon certaines estimations, collègues, vous le voyez si cette PPR a vocation à nous unir autour d'une ambition forte pour le ferroviaire. Alors oui nous le la faisons nôtre et puisque nous sommes nombreux à aimer le train et qu'il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour au-delà de tout ce que je viens de rappeler, s'il fallait une raison supplémentaire. Je me bornerai à rappeler la reprise de la dette à hauteur de 35 milliards d'euros. Pour conclure, si les objectifs visés par cette PPR sont louables, celle-ci ne nous apparaît pas d'autant qu'une nouvelle programmation pluriannuelle, pour le ferroviaire va être établi sur la base du prochain rapport du conseil d'orientation des infrastructures. Le groupe RDPI s'abstiendra donc sur ce texte. Merci, cher collègue, la parole est à présent à madame Martine Filleul du groupe socialiste.--

au début des années 90, la SNCF reprenez fièrement cette citation d'Aristote pour slogan publicitaire et pourtant aujourd'hui à l'heure où le développement du rail s'impose comme une arme incontournable pour limiter nos émissions de carbone et éviter la congestion du réseau routier des voyageurs partout dans notre pays vivent au rythme de la galère des transports, cette France qui se lève tôt et qui arrive en retard, la France des trains à l'arrêt dans ma région des Hauts de France, les mêmes cette se répète quotidiennement pour les usagers du TER, dans les salles devenues des salle des pas perdus. Ceux-ci craignent chaque matin de découvrir que leur train a été supprimés faute de conducteurs de contrôleur ou de matériel en quelques années à peine, la situation s'est dégradée à tous les étages. Partout en France, trains régionaux, TGV, aucun n'est épargné. Le taux de régularité que la SNCF tente de maintenir difficilement tous les jours est un exploit au regard de la vétusté de notre réseau. À la lumière de ce constat, nous pouvons affirmer que oui. La SNCF est en voie de clochardisation. Pour autant, les Français ont envie de trains, 12 millions de billets ont été vendus pour le seul. Été 2022, un record, alors même que les billets étaient hors de prix pour une partie de nos concitoyens et que les trains pris d'assaut affiché complet en cette période où les prix de l'essence se sont envolés, le train et la promesse de concurrencer au mieux la voiture. Les Français sont au rendez-vous tant que le service et de qualité et abordables ayant de l'ambition. Il est plus qu'inadmissible que nous soyons aujourd'hui rendu à abaisser la vitesse commerciale d'exploitation parce que le réseau n'a pas été entretenues ou moderniser. Nous sommes à Los alors qu'en parallèle, nos voisins européens se lancent dans des dispositifs innovants comme la digitalisation de leurs réseaux. Opérant une maintenance prédictive, par le biais de capteurs pour intervenir avant que le matériel ne casse et ne mettent à l'arrêt le réseau en outre la réalité du réchauffement climatique met à rude épreuve nos infrastructures ferroviaires, les équipements doivent être adaptées et homologué. Face à ces changements. Alors oui, quand on voit que la SNCF est déjà à la peine pour entretenir son réseau en en raison pardon du manque de soutien de l'État. J'entends qu'il vous paraisse inconcevable de mettre en place des dispositifs innovants de développer ou de redévelopper le train de nuit le fret l'inter modalité prenons pour exemple l'abandon de de plateforme tri-modale connecté au réseau ferré pour le projet de canal Seine-Nord. Que d'argent public et de possibilités de développement économique gâcher. De façon plus globale, Jean-Pierre Farandou, que nous avons. Et auditionné plusieurs fois dans le cadre de la commission du développement durable évalue les besoins de la SNCF à 100 milliards d'euros d'euros sur 15 ans, une grande loi de programmation ferroviaire de planification et d'évaluation des besoins annuels au long cours est une nécessité. Au lieu de cela avec le contrat de performance. 2021 2030. Le gouvernement a renforcé la règle d'or de SNCF réseau qui contraint sa capacité d'endettement et l'oblige à réaliser des efforts de productivité inatteignable. Faute d'un niveau d'investissements suffisants et dans un contexte d'ouverture à la concurrence, il risque d'affaiblir la SNCF et de générer chez les usagers une hostilité accrue. Nous refusons de voir cette stratégie menée à une privatisation. L'erreur serait majeur le rail a historiquement besoin de subventions publiques, que ce soit ici ou chez nos partenaires européens qui n'hésitent pas y recourir. C'est dans ce sens que mon collègue Olivier Jacquin a déposé en juillet dernier une proposition de loi visant à libérer SNCF. Réseau de ce carcan de règles d'endettement et de performance qui ne permet pas aux rails de répondre aux urgences écologiques. Également les socialistes au Sénat ont déposé un amendement au PLF visant à renforcer le soutien au ferroviaire à hauteur de 3 milliards d'euros, un montant certes important mais néanmoins indispensable à l'impératif de régénération et de modernisation du réseau, ce même amendement déposé par les députés socialistes a été d'ailleurs largement adopté en séance publique pour ne pas finalement être retenue par le gouvernement suite à l'application de l'article 49.3. Dès lors, le groupe socialiste ne peut que saluer cette proposition de résolution relative au développement du transport ferroviaire il votera pour. Il est grand temps de renverser la vapeur. et faisons le pari du train afin que les Français retrouvent confiance dans leur réseau ferré à l'heure de l'impératif climatique. Je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à présent à monsieur Pascal. Savoldelli du groupe communiste et vous avez 4 minutes, chers collègues.

Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. C'est un pan de nos politiques publiques.-- Parce que nous trouvons à un tournant en matière de mobilité et nous devons en avoir conscience. Cette proposition de résolution vise à à donner tort à un dicton.-- Ce dicton. C'est la seule façon d'être sûr de prendre un train c'est de manquer le précédent.-- Car la mobilité est un droit universel et qui devrait être accessible à tous et toutes. C'est écrit hein c'est présent dans l'exposé des motifs je cite se déplacer c'est pour aller étudier travailler, faire vivre des relations sociales amical, familial, c'est accéder aux soins, c'est pouvoir partir en vacances.-- Mais ce droit à la mobilité est mise à mal. D'un côté, il faudrait mieux se déplacer en réduisant la consommation d'énergies fossiles. C'est le moins qu'on puisse faire quand on voit les ravages de la pollution sur notre santé et notre environnement. De l'autre côté, on ne trouve pas suffisamment d'alternatives efficaces à la voiture et de transports publics, on devient un moyen de transport par défaut, alors qu'il devrait être un choix consenti. Permettez-moi ce pléonasme. J'en veux pour exemple la situation catastrophique dans les transports d'Île-de-France. L'attendent des bus, les suppressions, les retards de RER de métro sans parler des suppressions de postes et aussi de la criminalisation des syndicats de cheminots depuis des années maintenant depuis des années. Monsieur le Ministre. D'abord pénible. La situation est devenue insupportable. Nos collègues élus dans la région du groupe Gauche communistes, écologistes et citoyennes ont initié stoppe la galère et lancé une pétition pour demander des moyens et refuser la hausse du prix Navigo. Ce matin il y avait de nombreux élus et citoyens rassemblés en ce sens devant le conseil régional et à raison. Le service s'est dégradée rétrogradé même avec un entassement des passagers qui vont désormais devoir payer. On le sait depuis hier soir, presque 10 euros supplémentaires pour cette expérience scandaleuse et ce malgré votre annonce d'hier soir, des 200 millions.-- Le seul changement c'est donc 10 euros supplémentaires à la place de 15 euros. Oui et ce prix il est excessivement cher et il faudrait en plus se considérer comme des privilégiés. Comment être privilégiée quand les lignes sont surchargées avec des fréquences réduites et aléatoire et du matériel roulant, des fois vieillissant, hé bien ailleurs, il n'y a plus de services en un siècle, la moitié du réseau ferré français a fermé. Monsieur le Ministre, les gares sont venus des reliques des fois parfois transformée à d'autres fins, parfois même abandonnées et contribue au sentiment d'oubli de certains de nos concitoyens vivant dans la rue à la ruralité. Le transport de marchandises en partie aussi en pâtit aussi et ne représentent que 9% du secteur face à 89% pour le transport routier, plus coûteux pour l'environnement et vous reconnaîtrez notamment mes collègues vous recadrer très d'ailleurs mon engagement pour le maintien du train des primeurs entre Perpignan et Rungis. Rappelez-vous ces séquences ici dans l'hémicycle le transport ferroviaire né au niveau nulle part. Nous avons tous entendu des engagements pour rattraper le retard de la France notamment par rapport à nos voisins allemands, les engagements pris dans le contrat de courte performance d'abord avec la part du ferroviaire qui doit doubler d'ici 2030, les engagements du gouvernement sur les trains de nuit et c'est vrai il y a quelques lignes qui rouvre. Pour l'instant, elles sont encore en nombre insuffisant et loin des performances attendues pour un pays comme le notre qui a le moyen pourtant d'avoir de belles autoroutes privées. Et qui pourrait en retour, avoir des transports publics de qualité, enfin il y a l'engagement du président de développer digne de réseau Express régional de RER en métropole. On attend des précisions. On attend des financements et on attend aussi des garanties pour que le transport soit public et des Serbes, des territoires afin d'assurer le droit à la mobilité et non pas pour apporter sur un plateau un nouveau secteur lucratif au prophète de la privatisation des transports dans tout ça, il y a 2 catégories de responsables politiques, ceux qui parlent des transports et ça incontournable d'en parler, pour faire connaître cette situation lamentable et il a ceux qui agissent, hé bien maintenant il faut agir. Cette proposition de résolution fait un pas vers la transition des mobilités et agir. Mes chers collègues. C'est la voter. Merci. Cher collègue. La parole est à présent à monsieur Jean-François Longeot du groupe Union centriste pour. Six minutes. Bien, madame la présidente, monsieur monsieur là elle est hauteur de la à PPR, mes chers collègues, je suis très heureux d'être devant vous aujourd'hui pour exposer la position du groupe Union centriste sur la résolution présentée par nos collègues du groupe CRCE. À la tête de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Je n'ai eu de cesse de rappeler l'impérieuse nécessité du développement ferroviaire dans notre pays. Le secteur du transport et le plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. En France, or une tonne de marchandises transportées par voie ferroviaire émet 9 fois moins de CO2 que par la route le développement massif du ferroviaire pour le fret, comme pour les personnes représentent donc un levier considérable de décarbonation à l'échelle de notre pays. Lors de l'audition du président directeur général de la SNCF comme celle comme celle du ministre des transports, il y a quelques semaines devant la commission. J'ai souligné la nécessité absolue de faire croître le secteur ferroviaire dans notre pays tout en rappelant que les moyens. Mis sur la table n'était pas conforme à nos ambitions. Si nous souhaitons atteindre l'objectif. D'ici à 2030 d'un doublement de la part modale du rail à 20% pour les voyageurs et à 18% pour le fret. Il nous faut investir massivement dans notre réseau et ce sans plus perdre de temps. Afin de par parvenir à ce doublement de la part modale du ferroviaire, la proposition de résolution invite à réduire la TVA sur les titres de transport en commun. Partageant ce souhait. Je suis très heureux de vous rappeler mes chers collègues. Que l'amendement visant à baisser la TVA à 5 5 % sur les titres de transport porter au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable par Hervé Gillet et Philippe Tabarot a été adopté lors de l'examen du PLF je suis donc parfaitement face avec les auteurs de cette résolution. Le plan de relance avait alloué, plus de 4 milliards d'euros supplémentaires à SNCF réseau donc 2,3 milliards pour les investissements en faveur de la rémunération du réseau afin d'aider le secteur. Pour autant, le nouveau contrat de performance entre l'état et SNCF et réseau qui faisait l'objet de très fortes attentes.-- Constitue une occasion, une occasion manquée, tant il déçoit par son manque d'ambition. Seuls 2 9 milliards d'euros par an sont prévus pour le réseau sur la période 2021 2030. Une enveloppe très insuffisante pour assurer la régénération des infrastructures. En outre, ces crédits seront majoritairement issus des fonds propres de SNCF réseau, en particulier, du produit des péages dont le montant en France est déjà le plus élevé en Europe. Cette déception est d'autant plus grande que l'inflation grève les marges d'action de SNCF réseau à hauteur de 500 millions d'euros en année pleine perte non compensée dans le projet de loi de finances. À moyens constants. Cette situation risque de conduire à un resserrement du périmètre d'investissement de cet acteur. Des inquiétudes. Portent sur l'état des petites lignes ferroviaires, parent pauvre du réseau national dont le Sénat avait souligné l'importance lors d'examen du projet de loi 3DS et dont le maintien représentent des enjeux financiers considérables. Selon le rapport Philizot de février 2020 40 % de ce réseau de proximité et menacée faute de régénération. Le rapport estime nécessaire des investissements de l'ordre de 7,6 milliards d'euros d'ici à 2028. À ce titre, on peut se réjouir de l'absorption du Sénat d'un amendement déposé au nom de la Seat TDD visant abondé de 150 millions d'euros supplémentaires. Les crédits alloués à la régénération des petites lignes ferroviaires, n'est-ce pas. Cher Philippe Tabarot. Dans ce contexte des tensions budgétaires et et de nécessité d'accélérer rapidement nos efforts. La proposition de résolution par porté par nos collègues me semble tout à fait intéressante et puis la bienvenue. Je souhaiterais présent à aborder avec vous, chers collègues. Mon analyse. De 2 objectifs avisé afin d'atteint dans le doublement de la part modale du transport ferroviaire. Il existe, à mon sens un double enjeu, la régénération des petites lignes. Et des lignes d'équilibre du territoire, d'un côté et le développement des lignes urbaines voire métropolitaine de l'autre. Bien sûr, en tant qu'ancien maire et conseiller départemental. Je ne peux qu'être sensible aux arguments avancés par nos collègues quand ils expose à à raison que la moitié du réseau. Ferroviaire a fermé depuis 1930. Partout sur nos territoires. Nous avons constaté la déprise ferroviaire qui a eu lieu avec son lot de fermeture de petites lignes et de gars. Il faut donc briser ce cercle vicieux et donner une nouvelle dynamique dynamique puissante aux lignes locales qui font l'objet d'un engouement considérable de la part de nos concitoyens. La 2ème priorité impérieuse à laquelle nous devons adresser une réponse puissante et le besoin de transport ferroviaire dans les grandes métropoles françaises. La densité du réseau ferroviaire en Île-de-France fait figure d'exception parmi nos grandes villes, il faut et poursuivent les travaux d'agrandissement du réseau qui sont en cours. Le Grand Paris Express. Le projet Eole la prolongation des lignes de métro existence et la finalisation du du vaste réseau de tramway franciliens ces projets permettront de décarboner sur le long terme les mobilités au sein de notre région capitale. Quant à nos métropoles régionales que sont Marseille, Lyon, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Toulouse et d'autres encore elle mériteraient de bénéficier d'investissements d'ampleur dans les réseaux afin d'y permettent l'éclosion de véritables réseaux de trains de banlieue, à l'image des S-Bahn allemands qui sont présents dans de très nombreuses villes. Je salue l'annonce du président de la République de doter ces métropoles de réseau Express métropolitain car le potentiel de décarbonation au sein de ces zones est énorme tant les mobilités par vous automobile ils sont courant. Espérons que les moyens budgétaires seront à la hauteur de ses engagements. Le groupe Union centriste est en phase avec cette proposition de résolution.-- Et les objectifs de cette PPR ce groupe votre mon groupe votera donc en faveur de ce texte. Merci, cher collègue, la parole est à présent à monsieur Henri Cabanel pour le groupe RDSE. Vous avez 4 minutes, chers collègues. Madame la présidente, monsieur le ministre et chers collègues. Nos concitoyens subissent des hausses de prix sur tous les fronts et en particulier sur l'énergie, l'alimentation et les transports inflation galopante qui durable d'un côté endettement aggravé de l'autre et tout cela dans un contexte d'urgence climatique. Cette équation insoluble ne peut susciter tôt ou tard que l'explosion sociale. La politique ferroviaire, grande oubliée des dernières décennies a fait l'objet d'un regain d'intérêt relativement récent, nous payons aujourd'hui au prix fort l'inertie qui a été celle des gouvernements qui se sont succédé. La régénération et la modernisation du réseau quand elle progressive sont bien moins coûteuse qu'un coup d'accélérateur porté sur des elle fera que. Culture pardon dont l'âge moyen et d'une trentaine d'années, ce qui se traduit par un prix des péages 2 fois plus élevé par rapport au reste de l'Europe. Sur les trains de nuit après sur le simple abandon en 2016. Il aura fallu que nos voisins européens s'y intéressent, pour finalement décidé de les relancer. Cependant les moyens engagés ne correspondent pas actuellement aux besoins, soit 800 millions d'euros dans les 5 prochaines années. Nous payons le choix d'avoir favorisé les métropoles, la concentration des richesses au détriment du reste du territoire. 47 ans après le plan annoncé par Valéry Giscard d'Estaing. Le Massif central n'a toujours pas été désenclavée par le train. Au XXIe siècle les pans entiers du territoire se retrouvent mal desservies. Ah mais que les sages du droit à la mobilité. Nous avons aussi nos grands projets aux procédures interminables comme ça été le cas de la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan décidé dans les années 80 abandonné puis relancer. Un espoir se dessine avec le vote de nouveaux financements à loi de finances et Monsieur le Ministre, je voudrais remercie. À ce qui concerne le transport de marchandises il s'effectue essentiellement par la route d'un autre pays. Le plan de soutien au fret ferroviaire si les bienvenus et malheureusement arrivé un peu tard pour être jour compétitif le ferroviaire doit être performant efficace le système européen de gestion de trafic, des trains et la commande centralisée du réseau doivent impérativement être mises en place. Enfin comment inciter au rapport Mauroy modal ça me protéger l'usager de la hausse des prix. L'alternative à la route doit être crédible et pas demain. Soutenu par l'État. Or non seulement le transport ferroviaire n'est pas suffisamment compétitifs mais il devra subir 1,7 milliards d'euros de surcoûts liés à la flambée du prix de l'énergie. On n'hésite pas à instaurer un bouclier tarifaire énergétique de manière aveugle et coûteuses. Que sur la situation économique aux professionnels des ménages, il est logique que cet effort soit poursuivi en matière de transports collectifs. nous soutenons donc la proposition visant à ce que des dispositions exceptionnelles soient prises pour contenir l'incidence du prix de l'énergie sur les finances de la SNCF réseau et sur les autorités organisatrices de transport. Ainsi que la baisse de la TVA sur l'achat de titres de transport votée tous les ans au Chénois au Sénat à loi de finances. S'il faut améliorer le maillage ferroviaire du territoire, nous devons également ralentir l'étalement urbain et mieux réfléchir à l'organisation spatiale. Que de temps perdu que nos gouvernants que le gouvernement s'efforce de rattraper et je le salue. Il y a eu bien des progrès en termes de. Si seulement nous ne pouvons pas le nier. Lors de l'examen du projet de loi de finances. Monsieur le Ministre des transports a évoqué plus de 6 milliards d'euros investis en 2023 de la politique ferroviaire. Si les sommes paraissent désormais considérable et que nous nous situons dans la trajectoire établit par la nous pouvons faire davantage car la décarbonisation du secteur du transport repose pour beaucoup sur le monde ferroviaire. Nos voisins allemands Bicanic ou suisses ont récemment mis la main au portefeuille. Alors que le réseau est un est un bien meilleur état aussi. Nous vous invitons le Gouvernement aussi les ambitions françaises, notamment pour les petites lignes. Pour toutes ces raisons, le groupe RDSE qui partage l'ensemble des constats établis par les les auteurs et la quasi-totalité des propositions avancées bien sûr soutiendra la présente proposition de résolution, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est enfin monsieur Philippe Tabarot du groupe Les Républicains et vous avez 5 minutes, chers collègues. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, cette résolution a l'Avantage de porter le débat sur une passion française, celle de La Vie du rail. Avec notre étendard le TGV le rail est une fierté française en même temps qu'un instrument de notre cohésion nationale. Plus encore que la prouesse technologique il représentait c'est l'engouement du public pour un moyen de transport confortable massifier sur peu polluant qui fait du train, une grande réussite nationale le train c'est une carte de France qui se dessine et le témoignage de notre Patrimoine coréen comme aurait pu le dire, Marc Laménie, le train, c'est un défi. Qui coche les cases de notre temps, la nécessaire décarbonation notamment pour le fret aussi je partage bien volontiers les constats de cette PPR dans la droite ligne de nos travaux transpartisans de commission cher président Longeau avec notamment notre collègue Lahellec. Il n'y a pas un train de gauche et une rame de droite. Nous avons le devoir de nous hisser au dessus pour prendre des décisions. Nous partageons ce sursaut qui doit naître sur les mobilités ferroviaire qui doivent prioriser de futurs projets, comme le Grand Paris Express comme les accès du Lyon-Turin ma chère Martine Martine Berthet mais aussi la sauvegarde des petites lignes vitrine une France périphérique trop souvent laissé de côté. Nous sommes tous sur ces bancs, un peu amer que les transports soient continuellement les grands absents des campagnes présidentielles et de ces débats. Et malgré cela le train Trust l'actualité devient un élément pivot de réponse aux crises de notre temps. Et pourtant l'acuité médiatique du train demeurent inversement proportionnel au PIB injectés chaque année dans le financement du transport public, le retard pris est si grande que les investissements de régénération permettent tout juste de stopper la dégradation du réseau le montant d'investissement par habitant est ridiculement bas, seulement 40 euros en France quand il est de 395 euros en Suisse, 95 en Italie. Ce sous-investissement chronique c'est dernièrement manifesté par son nouveau totem, vous l'avez dit chers collègue le contrat de performance. Ce document encadre fait courir un risque majeur à nos infrastructures. Il prévoit des investissements de renouvellement notoirement insuffisant et fait l'impasse sur la modernisation du réseau pour traduire l'ambition du train et le retour des Français dans les rames, il faut investir davantage pour rattraper le temps et non pas dépenser le temps de l'action décision. En cohérence. Vous l'avez dit, nous avons fait voter ici pour le PLF 2023 150 millions d'euros supplémentaires à la régénération du réseau. Monsieur le Ministre, sans vous cacher éternellement derrière le CO donnant les mêmes chances au ferroviaire au moins équivalente à celle octroyée aux filières automobile et aéronautique sans pour autant les opposer nos attentes sont vivaces car elle porte une existence rehaussé équilibrée. Elle ne se tourne pas vers la facilité des annonces solennelles aux pieds d'argile, comme celle du président sur les RER métropolitains qui pour l'instant sont remisés aux ateliers de maintenance sans aucune trajectoire financière. Je suis conscient de la complexité de notre demande et des capacités limitées de SNCF réseau. En cela, nous ne pouvons nous cantonner aux seul sirènes de 7 PPR elle porte de grandes ambitions affichées. Sans jamais y adjoindre les pistes de solutions pour y arriver. Performance, productivité. Trajectoire de l'État en très forte révision lutte contre le poison des péages ferroviaires. Je ne peux également validé totalement la portée tant elle cache mal en arrière boutique une opposition plus dogmatique que réaliste et une certaine complaisance l'opposition dogmatique. Tout d'abord dans le fait de rejeter en bloc le Champ de l'ouverture à la concurrence à votre différent j'y crois car elle responsabilise et ne se complaît plus dans les travers du monopole. La concurrence ferroviaire ce doit être pour moi une offre accrue de train et à terme des péages ferroviaires plus accessible, une complaisance ensuite celle de ne jamais porter un regard objectif voire quelquefois critique par idéologie sur le Champ social miné. Avec une reprise de la dette. Ça a été dit 35 milliards, une recapitalisation. Les contribuables français ne cachent plus leur crispations envers les grèves à répétition qui ruinent nos efforts collectifs, les efforts de satisfaction de l'opérateur à des moments importants et souvent festives de leur vie. Et je fais bien la distinction entre certains syndicats et entre certains cheminots dont beaucoup restent attachés à la qualité du service et à l'amour de leur travail alors fidèle à mon héritage politique qui n'est pas prisonnier de ses vieilles lunes dogmatique, je crois au ferroviaire par conviction. Notre groupe cher Didier Mandelli sonores ainsi de réclamer un effort de rattrapage de modernisation et de performance ferroviaire mais il s'abstiendra sur cette proposition qui part des constats bienveillant que je partage reste prisonnière d'une idéologie quelques fois un peu trop politique sur les deux sujets que je viens d'évoquer.-- Merci, cher collègue, la parole est à présent à monsieur Clément Beaune Ministre délégué chargé des Transports.

Merci beaucoup madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Lahellec je vous remercie. D'avoir porté ouvert ce débat sur, comme l'a dit à l'instant le sénateur Tabarot une passion française qui est je crois les interventions successives en témoigne en tout cas s'il y a un point commun. Avec. L'orateur qui désormais s'exprime au nom du gouvernement, c'est que cette passion et. Que la volonté de faire du ferroviaire une grande priorité est également partagée mais permettez-moi avant de revenir sur. Quelques points prioritaires de la politique en matière de transport et ferroviaire singulièrement de réagir à quelques propos que j'ai trouvé pour être très sincères excessif. Je pense notamment Madame Filleul n'est plus dans l'hémicycle propos qu'a tenus la sénatrice ce filleul. On ne peut pas parler de clochardisation du système ferroviaire français. Ce n'est ni juste ni vraie et je m'indigne contre ce genre de propos. Je crois que ça ne fait pas avancer le débat, il ne figure pas, d'ailleurs je m'en félicite. Dans le texte. La proposition de résolution.-- On ne peut pas traiter notre système ferroviaire de cette façon. Bien sûr et j'y reviens dans un instant nous devons évoquer la galère que vivent beaucoup de Français nous devons évoquer les difficultés qui sont évidentes et auxquelles nous devons répondre et prendre nos responsabilités peut-être nous aurons des désaccords. J'y reviendrai dans un instant aussi on ne veut pas partir de ce constat qui est faut biaiser et outrancier. Je ne m'y résous pas car ce serait une autoflagellation collective. Un SNCF bashing. Si vous me permettez cet anglicisme auquel je ne m'associe en rien il y a des difficultés dans le système ferroviaire. Oui. Mais partons quand même de ce qui fonctionne aussi et qui fait la vie quotidienne des salariés du secteur public ferroviaire et des usagers qui, malgré les difficultés recours aux transports publics utilisent le train, j'ai beaucoup voyagé en Europe car les hasards de la vie on fait qu'avant d'être mis sur les transports. J'ai été mis chargé des affaires européennes. Et ça n'est pas vrai que l'herbe est verte ailleurs et que tout serait sombre et noir de notre pays. Il y a des succès français le sénateur Tabarot et plusieurs autres monsieur Dacbert notamment l'ont rappelé à l'instant qui sont de vrais succès partagé d'ailleurs je ne cherche pas me les attribuer aucunement qui sont portés par les collectivités locales, toutes sensibilités politiques confondues par les gouvernements successifs. La politique du TGV qui l'est aujourd'hui commode et commun de dénigrer a été une grande politique d'aménagement du territoire, le développement économique et de succès industriel et ferroviaire français, soyons-en fiers et d'ailleurs plusieurs ont réclamé aussi je pense sénateur grand qui nous a quitté ses quelques instants, qui a défendu l'idée qu'on doit ouvrir à certains endroits où il y a un manque de compétitivité un désenclavement un besoin d'attractivité économique des lignes ferroviaires, il faut sans doute les financer autrement le soutien du Sénat et le vol de trois amendements qui est sur les projets GPSO elle MPM et PCA pardon qui ces acronymes aujourd'hui bien connus ont permis de financer par des ressources locales affectées pesant sur le monde économique et monde touristique mais en concertation avec eux permettent que l'on ne prélève pas justement les ressources du système ferroviaire et confidences intelligemment de futures lignes à grande vitesse avec des projets ciblés.-- On a aussi eu réussi une grande réforme en France et se sont largement les régions qui le porte en pratique mais malgré, malgré, pardon les difficultés qu'ont été recensés sur les TER, les TER d'aujourd'hui il y a des difficultés ponctuelles, notamment dans les Hauts-de-France. Je le sais, je m'y suis engagé mais n'ont rien à voir avec ce qu'on a connu il y a 20 ou 30 ans, vous le savez bien parce que les régions ont investi réinvesti. Le tarif vous le rappeliez je crois Monsieur le Sénateur Tabarot dans notre débat l'autre jour le tarif que payent en moyenne les usagers français sur le prix du billet tout type de ligne confondus du train du quotidien à la grande vitesse.-- Et le plus faible d'Europe par le Luxembourg. C'est d'ailleurs peut-être un des débats que nous devons avoir, nous investissons en effet toutes collectivités publiques confondues, dont l'état dans une subvention très importante au ferroviaire. ferroviaire. Je sais qu'on a des débats sur les tarifs en ce moment. C'est d'ailleurs pour ça je remercie ceux qui l'ont souligné que par ma voix, l'État s'est engagé à donner une aide d'urgence non seulement bien sûr à l'Île-de-France mobilités parce qu'il y avait un besoin particulier mais aussi aux autres autorités métropolitaines organisatrices de transport à hauteur de 100 millions d'euros. Nous irons les débats pour la suite. Mais c'est très important pour faire face au coût de l'énergie, ne pas faire exploser les tarifs. Nous sommes ce pays collectivement qui subventionnons les usages du ferroviaire et les transports du quotidien, c'est une fierté et c'est très important et puis il y a des choses c'est vrai qui depuis longtemps. Où en ce moment fonctionne moins bien ou fonctionne mal, disons-le, pour essayer de le résoudre. Je pense évidemment, la question du réseau. Je l'ai toujours dit vous me l'avez entendu dire plusieurs fois dans cet hémicycle. Et il y aura encore des étapes à franchir, je ne me cache pas derrière le Conseil de l'orientation des infrastructures. Monsieur le sénateur, c'est plus large que cela. Le réseau ferroviaire. Oui là il nous avons collectivement un problème français. J'aurais aimé d'ailleurs parce que soyons honnêtes intellectuellement dans nos débats allant jusqu'au bout qu'on salue néanmoins que depuis 5 ans, 6 ans, pour être très précis, vous voyez je suis honnête on a réinvesti augmenter les crédits de régénération et de modernisation de notre réseau ferroviaire, c'était indispensable. On était à moins de 2 milliards d'euros par an 2015 donc j'entends les critiques et les contestations sur les 2,9 milliards d'euros par an prévus dans le contrat de performance. Il a un mérite, c'est qu'il nous met à un niveau qu'on n'avait pas atteint depuis plus de 30 ans. Et que en plus ils prévoient une sur 10 ans. Faut-il aller plus loin j'reviens dans un instant. Oui. Est-ce que cette proposition de résolution à l'Avantage de mettre l'accent sur ce point. Oui je le reconnais. Sur ce point précis, mais disons que cet effort est en train d'être en partie compensée rattraper et que nous devrons franchir des étapes supplémentaires. Je n'ai pas beaucoup entendu que on était dans un état de clochardisation lorsqu'on était à moins de 2 milliards d'euros par an. Il y a encore moins d'une décennie. Donc soyons justes, soyons honnêtes, pour être plus efficace dans nos réponses. Je pense aussi que oui sur aujourd'hui certains trains du quotidien. Nous avons des difficultés particulières. J'ai évoqué les coûts de l'énergie, l'État fait cette aide exceptionnelle, c'était important. Ça n'est pas négligeable. Et oui, nous avons parfois des situations très particulières. J'ai mentionné l'Île de France, j'ai mentionné, Les Hauts de France, c'est pour ça d'ailleurs qu'avec le président de région, Xavier Bertrand, je me suis rendu à Lille, j'ai discuté avec lui, j'ai demandé à la SNCF un plan exceptionnel de rattrapage des recrutements face aux pénuries de conducteurs, il commence à se mettre en place, nous allons essayer de l'accélérer encore en mobilisant tous les moyens, cela a parfois été moquée sur certains, je l'assume parce que nous sommes dans une période difficile, faire appel à Lyon une retraitée faire face aux pénuries temporaires. Il faut mobiliser tous les moyens, être créatif est innovant comme cela a été dit et répondent plus structurellement pénurie de conducteurs qu'on connaît partout, ce n'est pas une problématique de ce gouvernement ou de l'État, nous les connaissons les collectivités locales le savent bien, dans les recrutements de conducteurs de bus de conducteurs de métro et je m'engage aussi dans cette politique d'attractivité et de recrutement renforcée en Île-de-France comme ailleurs. Alors oui, nous avons un budget ferroviaire qui reste important et je le rappellerai pas en détail les chiffres évoqués il y a quelques jours à peine sur le projet de loi de finances pour 2023, 2 ou 3 simplement. 85% des crédits que. Le Sénat a voté vendredi dernier sur le programme consacré aux transports sont consacré précisément aux transports collectifs et ferroviaire. Donc il n'y a pas le choix qui se porterait massivement sur la route ou sur l'avion, c'est 85% du budget du ministère que je défends. Au total, si l'on additionne l'Agence de financement des infrastructures. La Société du Grand Paris. Le budget qui est directement dans le programme que j'évoquais. Nous avons un total de 12 milliards d'euros d'effort national de l'État consacré aux transports cette année c'est un niveau plus important que l'an dernier le plus de 10%. Et là c'est plus de la moitié de cet effort collectif qui est consacré au transport ferroviaire. Donc je veux aussi qu'on rappelle ces réalités alors que doit-on faire pour améliorer. Répondre. Un certain nombre de points qui ont été soulevées. D'abord cette priorité au réseau. Je l'ai dit, c'est un signal. Prenons-le comme tel. Pour atteindre ce niveau symbolique également le 3 milliards d'euros dans la régénération du réseau ferroviaire et sa modernisation. La fille portera dans son vote souhaite du budget dans quelques jours, 100 millions d'euros. Au-delà du contrat de performance pour 2023 vous me direz, il faut aller peut-être encore plus loin. D'abord j'indique que SNCF réseau le PDG Matthieu Chabanel pourrait en témoigner, indique lui-même qu'on ne peut pas absorber de toute façon en travaux. Ça n'est pas magique des sommes qui s'additionnent trop rapidement, donc c'est un signal utile concret pragmatique et puis nous aurons aussi sur la base du rapport du CO il mais plus largement la question d'un investissement supplémentaire dans le réseau, ça n'est pas fini, c'est un débat je ferai des propositions avec le gouvernement et Christophe Béchu en début d'année et nous en rediscuterons donc je ne dis pas que ce contrat de performance est une religion qu'il ait un tabou ou un totem. Je dis simplement, prenons le sur ce qu'il a une amélioration que nous amplifions pour 2023 et qui sera rediscuté ensemble politiquement et budgétairement. Dans les semaines et les mois qui viennent. Nous avons aussi à donner une priorité aux transports du quotidien. Je suis sûr, je, je suis revenu, pardon, sur les mesures d'urgence. Je veux dire un mot du RER métropolitains. Nous allons parler vendredi je ne serai pas trop long mais ils sont évoquées également monsieur le sénateur Lahellec dans votre proposition. C'est d'abord pas de la communication de la science fiction mais une réalité. J'ai avec le région Jean Rottner. La prison de la métropole. L'Eurométropole de Strasbourg Pia Imbs ce ce matin même lancé symboliquement ça fonctionnera à partir de ce 11 décembre le RER métropolitains à Strasbourg, qui est un effort conjoint financier d'investissement de l'État de SNCF réseau de la région de la métropole qui va permettent d'avoir une augmentation extrêmement significative des circulations autour de la métropole de Strasbourg. Donc ça montre la voie. Et nous avons déjà étudié un certain nombre de projets de RER de RER métropolitain une dizaine. C'est ce qu'a évoqué le plan de la République. Hé oui ce dodo, cela doit être une priorité. Cofinancé co-construite, État et collectivités, dans les années qui viennent. C'est un projet d'une décennie. Certains sont plus mûrs que d'autres et nous aurons aussi, je le redis comme je l'ai dit à l'instant sur les sociétés de projets pour la ligne à grande vitesse à inventer des modalités de financement nouvelles, pour ne pas aller prélever sur des transports qu'on doit aider déjà aujourd'hui des ressources qui sont rares ou un satisfaisante ou partiel et donc imaginer des outils comme le souhaitait le projet sera aussi une partie. Le ce débat que nous aurons dans les mois qui viennent à partir du rapport du conseil d'orientation des infrastructures. Je veux revenir plus spécifiquement puisque ces points ont été évoqués. Non seulement la proposition mais dans plusieurs interventions sur quelques axes qui sont sensibles et importants. J'ai le sénateur Dacbert à développer les chiffres. De manière précise. Donc je vais essayer de ne pas être répétitif, mais insisté sur quelques points le fret ferroviaire.

jeune réduction année après année, de la part modale du fret ferroviaire. Je me suis engagé personnellement et c'est encore un dossier en cours difficile nous y arriverons à préserver. Un opérateur fret SNCF qui est essentiel, nous sommes en train de gagner collectivement avec les opérateurs de fret ferroviaire, pas seulement la SNCF la bataille du report modal si difficile. Pour laquelle la France a été si critiqué tous gouvernements confondus nous augmentons pour la première fois depuis plus de 20 ans, depuis 2 ans la part du fret ferroviaire dans le fret total dans ce pays, c'est une réussite que je ne maîtrise en rien qui est collective. Il y a une stratégie nationale du fret qui a été porté par le gouvernement précédent. Que je m'engage à poursuivre, j'ai donné quelques indications. Ce ne sont pas des montants négligeable, 170 millions d'euros par an. Chaque année, jusqu'à 2024 garantie sur différents dispositifs dont la de wagons isolés. C'est essentiel 250 millions du plan de relance. Au total, c'est un plan, un milliard d'euros. Vous l'avez dit, monsieur le sénateur Dagbert qui est mobilisée qui se déploie et je le dis, je le confirme, nous prolongerons les aides jusqu'à prévu pardon actuellement jusqu'à 2024 jusqu'à 2027 jusqu'à la fin du mandat si le Parlement confirme ses crédits parce que je pense que c'est important de donner cet engagement et cette visibilité pour ne pas perdre ce sursaut dans le fret ferroviaire, notamment dans le transport combiné, que nous avons gagné ensemble depuis quelques années et qu'il demeure évidemment fragile et évidemment à consolider. La question des petites lignes a été évoquée. Nous en parlions là aussi dans le débat budgétaire, elle est essentielle là également. Il est vrai qu'il y a eu des fermetures de petites lignes. Pendant.-- Plusieurs décennies. Il est vrai aussi que nous sommes en train, collectivement, là encore, car c'est forcément un partenariat, État et région en particulier d'inverser la tendance. Je rappelle les grands chiffres en 2 mots. Le Premier ministre Jean Castex à l'époque avait beaucoup insisté sur ce point, remis des crédits inciter la SNCF a signé des conventions et il y a déjà 8 protocole État régions là encore toutes sensibilités politiques confondues qui ont contractualisé et qui ont permis, sur 9000 kilomètres, qui avait été identifié dans ce plan de petites lignes de contractualiser sur déjà plus de 6000 kilomètres. Et l'État. A doublé, triplé pardon les financements consacrés annuellement au financement au cofinancement des petites lignes sur la période 2022 1022, ses 550 millions d'euros. Nous sommes aujourd'hui à 200 millions d'Europe 1 et ce sera confirmé prolongé dans la prochaine génération de contrat de plan État-Région qui sera conclue au cours de l'année 2023. J'invite là encore si on veut être cohérent. Toutes les régions qui n'ont pas choisi cette démarche contractuelle proposée ouverte par l'État. La porte reste ouverte à s'engager à cofinancer. Avec nous la réouverture ou la préservation de petites lignes.-- Un mot sur le train de nuit qui a été aussi évoquée comme un élément là encore sur lequel on doit je pense réinvestir sur laquelle il y a eu parfois pendant des décennies, disons-le aussi franchement des reculs c'est exact avec la transition écologique avec un nouvel appétit pour le train, il y a sans doute. Une volonté.-- Collectif plus importante de se réengager sur le train de nuit, il n'y avait plus de de ligne en 2021, nous en avons déjà rouvert de, comme vous le savez. En 2021 2. Les deux lignes Paris-Nice et Paris-Tarbes-Lourdes et il y a aujourd'hui, je le disais encore vendredi une discussion qui devra repasser par des discussions parlementaires et budgétaire pour les commandes de matériel roulant, certaines sont déjà engagés pour les lignes existantes, je rappelle que pour Paris-, Briançon et Paris-Rodez-. Toulouse le matériel roulant et déjà en cours de rénovation et le sera entièrement d'ici la fin de l'année 2023, ces 50 millions d'investissement de l'État et pour le reste, il faudra une commande industriels et budgétaires supplémentaires sur la carte des nouvelles des nouvelles lignes de tram oui pardon, qui se sont qui seront rouvertes au-delà des deux qui ont été déjà réouverte en 2021. Je crois là aussi qu'on illustre un tournant à amplifier sans doute à consolider certainement que nous portons, que le gouvernement précédent et ce gouvernement défendent en matière d'accessibilité, de développement du train dans toutes ses modalités, y compris fret. Petites lignes trains de nuit et segments du ferroviaire, qui avait été parfois.-- Successivement par les différentes majorités différentes gouvernements oubliés négligés ou cassé. Et puis je veux revenir sur la question des tarifs que j'évoquais, brièvement, je le dis là aussi ça fait partie des fiertés française, nous sommes le pays où on aide le plus l'usager.-- Par une prise en charge publique à avoir recours aux transports publics si bien d'ailleurs que nous sommes le pays. Où il y avait eu le moins longtemps un effondrement des recours aux transports publics pendant la crise de la Covid. Une partie des mesures tarifaires que prennent nos voisins vise aussi à refaire à faire revenir les gens dans les transports publics là où en France nous avons malheureusement plutôt. Difficultés à satisfaire toute la demande et des trains, des métros, des bus qui, pour les raisons que j'évoquais sont aujourd'hui malheureusement bondés.-- Nous avons pris là aussi pour ce qui concerne l'état, le gouvernement en donnant. Des orientations claires à la SNCF des mesures que j'assume. Nous sommes dans une période de très forte inflation de très forte hausse des coûts de l'énergie néanmoins et c'est un effort de l'entreprise publique de ses activités de l'ensemble de ses salariés. Un bouclier tarifaire qui a été mis en place par la SNCF. l'augmentation moyenne des tarifs et des protections pour ceux qui sont les plus exposés qui ont des abonnements parce qu'ils utilisent le train régulièrement, notamment pour le travail. Nous avons gelé ses tarifs et pour le. Qui est aussi un mode de développement de transports pardon et de mobilité, plus social, qui concerne beaucoup de jeunes où beaucoup de familles qui ont moins de moyens. C'était très important aussi de prendre ces mesures. Donc pour résumer, je prends cette proposition de résolution comme un appel.-- Comme une volonté d'aller plus loin. Je ne prends pas dans les interventions et dans quelques éléments de cette proposition. Ce qui reviendrait à faire.-- En quelque sorte un discours de déclinisme ferroviaire. De flagellation collective, je le disais, je sais que ça n'est pas votre intention à monsieur Lahellec, mais je le perçois à certaines interventions ainsi je le prends comme une exigence. Prendrait que le gouvernement il sera pas favorable, mais je crois qu'on doit reconnaître aussi les efforts qui sont engagés depuis plusieurs années qui seront poursuivis que je suis prêt sur certains points, notamment la question du réseau à amplifier ce sera difficile parce que gouverner c'est choisir, y compris sur le plan budgétaire, mais il faut le faire en responsabilité dans nos échéances qui arrivent, dont le rapport du Conseil tentations d'infrastructures mais pas seulement. La négociation n'surtout au contrat de plan. Les discussions que nous aurons sur le réseau et je crois qu'ensemble dans cet esprit, nous avancerons. Merci beaucoup. Merci monsieur le. Ministre. Vos réponses très complètes. Nous allons procéder au vote sur la proposition de résolution.---- Comme je vous l'ai dit les interventions des orateurs Valais. Explications de vote, je mets donc aux voix cette proposition à main levée qui vote pour. Qui vote contre.-- Qui s'abstient.-- Cette proposition de résolution et donc adopté. Bravo, chers collègues. Mes chers collègues, je vais lever la séance prochaine séance jeudi 8 décembre donc demain à 10h 30 pour l'examen de la proposition de loi visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation et à interdire le démarchage de ses titulaires, la séance est levée. Bonne soirée chère collègue et bon appétit.